La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 10 avril 2025 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation. Je n'en vois pas. Le procès verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Henri Thor qui fut sénateur de l'Ardèche de 1980 à 2008. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la Commission mixte paritaire, chargée d'abord d'un texte sur les dispositions restantes en discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafique et de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée. La conférence des présidents a décidé que ces textes feraient l'objet d'explications de vote communes. La parole est à madame Muriel Jourda, rapporteur pour les Sénats de la Commission mixte paritaire. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres je crois qui arrivent effectivement. Mes chers collègues, quelques mots effectivement sur la lecture de ces conclusions de commission mixte paritaire sur le narcotrafique pour parler de cette situation de manière générale. Vous vous rappelez tous que la commission d'enquête, qui avait été mise en œuvre en novembre 2023, à l'initiative du groupe Les Républicains, mais qui a donné lieu à un travail transpartisan, puisque le président en était Jérôme Durin et le rapporteur Étienne Blanc, avait permis de mettre en valeur à quel point le narcotrafique n'est pas une simple suite d'infraction qui troublerait l'ordre public, mais bien une série de comportements qui portent atteinte aux intérêts entiers de la Nation. De sorte que, après que cette évidence a été mise en valeur par ce travail, les mêmes auteurs, Jérôme Durin, mon co-rapporteur au nom duquel je m'exprime également à l'instant, et Étienne Blanc, ont déposé une proposition de loi sur laquelle nous avons eu l'occasion de travailler et qui traitait, port par pan, de l'intégralité des sujets qui devaient être soulevés et qui devaient donner lieu à modifications législatives pour que nous puissions lutter efficacement contre le narcotrafique. Ce travail a été fait ici, il a été fait de manière transpartisane et je rappelle que ce texte avait été voté à l'unanimité. Il a été fait également à l'Assemblée nationale et nous avons réussi, après de multiples discussions, mais qui ont été fructueuses, à trouver un accord sur l'intégralité des points de ce texte. Le temps qui m'est imparti ne permet pas de mettre en avant la totalité de ces points. J'en mettrai peut-être trois en avant. Le premier, c'est le fait que nous ayons pu décider d'un parquet. le parquet national qui va lutter contre la criminalité organisée, que l'on appellera désormais le PNACO, un parquet unique qui va coordonner l'action des autres parquets sur la criminalité organisée et sur le narcotrafique. Cela est nécessaire si nous voulons arriver à maîtriser l'hydre du narcotrafique qui s'est abattu sur la France comme sur bien d'autres pays. Ce parquet qui sera opérationnel je l'espère en janvier prochain, c'est ainsi en tout cas que nous avons fixé la date avec je crois l'accord de monsieur le garde des Sceaux qui acquiesce, ce parquet permettra effectivement de lutter efficacement. Nous avons, et c'est un autre point je vais chronologiquement vers l'instruction, aussi changé le régime à la fois des demandes de l'unité mais surtout des mises en liberté. La mise en liberté d'un narcotrafiquant est un enjeu absolument crucial pour ce narcotrafiquant. Pourquoi ? Vous savez qu'en France, lorsqu'on est prévenu ou accusé et que l'on est détenu, on est jugé dans des délais impartis qui font qu'effectivement une décision de justice s'intervient. Dès lors que l'on est libre, et bien cette décision peut... ne pas intervenir malheureusement au regard de l'état d'encombrement de nos juridictions en France. Il fallait donc que cette espèce de guérilla procédurale qui est mise en œuvre aujourd'hui par les narcotraffiquants soit freinée par des dispositions qui ne sont pas attentatoires au droit de la défense mais qui permettent de façon objective de ne plus pouvoir soulever des moyens procéduraux qui sont des moyens soulevés de mauvaise foi et obtenir ainsi la mise en liberté de personnes qui ne devraient jamais sortir de prison avant d'être jugées toutefois. Le dernier point que je souhaiterais apporter, c'est l'incarcération. C'est l'issue. Cette issue, elle est importante. Nous avons beaucoup aussi travaillé sur ce sujet. Dans l'intervalle, nous ne l'avons pas vu au Sénat, mais l'Assemblée nationale, M. le garde des Sceaux, a proposé que des quartiers de lutte contre la criminalité organisée soient mis en oeuvre. Nous avons retravaillé ce point car nous étions favorables sur le principe avec nos collègues de l'Assemblée nationale, ce qui nous permet d'obtenir, me semble-t-il, un système assez équilibré dans lequel la décision du ministre qui permet d'avoir recours à ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée soit régulièrement réinterrogée tous les ans, de façon à ce que cette décision ne soit pas trop attentatoire non plus aux libertés individuelles. C'est un équilibre qui a été trouvé et qui me paraît bon. Voilà quelques points sur lesquels je souhaitais donner quelques éléments d'explication. Il y en a d'autres, bien sûr, dans ce texte, d'autres que nous avons déjà vus en séance, tous ensemble, et sur lesquels nous avons trouvé un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Il me paraît important que ce texte, qui a été adopté ici à l'énumité, voie une conclusion similaire. aujourd'hui au moment où nous lisons les conclusions de la Commission mixte paritaire, car je crois que c'est d'une seule voie que les parlementaires... Le gouvernement et les ministres qui sont là se sont beaucoup impliqués sur ce sujet, doivent parler face à l'hydre du narcotrafique de façon à ce que nous puissions efficacement lutter contre cette contre cette criminalité organisée qui s'abat sur la France avec son cortège de menaces, de corruption, de violence. Nous devons apporter une réponse qui soit commune, qui soit forte, qui soit unanime. J'espère que aujourd'hui encore cette même unanimité nous réunisse aujourd'hui dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Monsieur le Ministre Merci cher Amélie, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci au travail fait par les parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée nationale et en Commission exparitaire pour ce texte si important. pour nos magistrats, nos forces de l'ordre, pour l'ensemble de notre pays, pour lutter contre le narcotrafique. Merci tout d'abord évidemment aux auteurs de la proposition de loi, M. Blanc et M. Durin, même si une fois accouché, si je veux dire la proposition de loi, les pères peut-être considèrent que le bébé a grossi en nombre d'articles et peut-être a même été modifié mais modifié et enrichi avec votre accord je crois monsieur le rapporteur tant sur le parquet national criminalité organisé et non plus le parquet national anti stupéfiants que sur les dispositions très importantes que nous mettons et je vais rester évidemment au point de l'autorité judiciaire au service de nos magistrats notamment nos magistrats spécialisés Mais aussi, et vous l'avez dit vous-même dans votre rapport, monsieur le rapporteur ici au Sénat, des articles qui ne sont pas des cavaliers puisqu'il y avait quand même un certain nombre de dispositions pénitentiaires en fin de votre proposition de loi, des articles qui ont été très largement enrichis pour créer le nouveau régime carcéral, inspiré de l'article 43 bis. italien qui prévoit dans ce régime carcéral avec je l'espère demain les prisons de haute sécurité, donc la première le 31 juillet prochain à Vendane-le-Vieille et puis la deuxième le 15 octobre prochain à Condé-sur-Sarte, les lieux où nous allons enfermer les 200 premiers narcotrafiquants les plus dangereux, rampant ainsi avec une tradition pénitentiaire française qui consiste à classer ou à catégoriser les détenus selon leur statut dans la justice la détention provisoire, maison d'arrêt, les gens condamnés pour peine, prison pour peine, pour qu'effectivement nous puissions regarder la dangerosité des personnes et pas simplement leur statut dans la justice, puisqu'avant d'un levier, nous avons prévu d'y mettre 70% de gens qui sont en détention provisoire. Un régime carcéral extrêmement difficile, c'est vrai, mais qui permet d'isoler les trafiquants et les narcotrafiquants du reste de la société pour qu'ils arrêtent de pouvoir diriger leurs points de deal, blanchir leur argent, commander des assassinats, menacer des directeurs de prison, des agents pénitentiaires, des magistrats, des policiers, des femmes et des hommes politiques, des journalistes, des avocats, comme on l'a vu encore très récemment à Nancy, et de pouvoir couper, ainsi comme les Italiens l'ont fait, le lien social qu'il y a entre les gens qui sont détenus et l'extérieur, et notamment le narcotrafique. Alors évidemment, même la présidente vous l'avait dit, ce régime carcéral extrêmement original, et encore une fois difficile, pose des questions, et j'ai souhaité que le travail que nous avons fait avec l'Assemblée nationale, mais je sais que c'était la même concorde ici qui s'est exprimée au Sénat, puisse se faire, d'abord avec le rapporteur ici, monsieur Durin, pour le groupe socialiste, et de manière générale, je crois, la gauche dans l'opposition au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale avec M. Vico. J'ai souhaité d'une part que le Conseil d'État soit saisi des dispositions carcérales que je leur proposais, puisque ce n'était pas le cas de votre proposition de loi. Et nous avons modifié à l'avergule près, selon l'avis du Conseil d'État positif, ce nouveau régime carcérale qui nous permettra je suis sûr de passer les fourches codines du conseil constitutionnel mais également je me félicite du vote très large à l'Assemblée nationale comme ici à l'unanimité mais il n'y avait pas encore ces dispositions carcérales et j'ai donc souhaité dans un esprit de compromis partant du principe que nous étions à deux ans d'enfermement selon ce texte à l'Assemblée nationale de tomber sur un an pour que le groupe socialiste puisse voter le texte je pense qu'effectivement un an renouvelable avec évidemment La possibilité de voir très rapidement les jouesses présentes du Conseil d'État lorsque nous prendrons les premières décisions est un bon compromis républicain qui nous permet de mesurer en quoi ce régime carcéral est à la fois une volonté de la Nation toute entière tout en respectant la dignité de toutes les personnes détenues.

très récemment par les prises à parties extrêmement nombreuses, des dizaines et des dizaines de faits, des voitures d'agents pénitentiaires, leur domicile qui est attaqué à la Kalachnikov au cocktail Molotov, les centres de détention eux-mêmes. On a voulu faire on va dire, barrière à ce régime carcéral en imaginant peut-être que l'administration pénitentiaire, déjà sous le coup de menace, déjà sous le coup des difficultés extrêmement fortes de leur métier, fasse grève ou empêche l'adoption de ce régime carcéral. Ça n'a pas été le cas. Les agents de soignance, de probation, d'administration pénitentiaire ont été courageux. Ils ont tenu malgré les difficultés un peu partout en France. Vous les avez soutenus. Mesdames et messieurs les parentaires, je vous en remercie. J'en remercie le Parquet national anti-théoriste et les forces de l'ordre sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. d'avoir interpellé une partie, en tout cas très importante, des personnes qui sont responsables de ces menaces. Aujourd'hui, la réponse du Parlement, comme demain à l'Assemblée nationale, sera une réponse aussi aux narcotrafiquants qui ont voulu nous faire reculer et reculer l'autorité de l'État. Dès le Conseil constitutionnel, qui se sera exprimé, puisque, manifestement, il sera saisi par vos collègues de la France Insoumise, si j'ai bien compris les gazettes, nous allons préparer les décrets, que nous travaillons en même temps que la loi aujourd'hui est discutée, Et je proposerai, madame la présidente de la commission des lois, comme je vous l'ai dit, que nous puissions vous soumettre les décrets pour qu'au mois de juin, nous publions les décrets qui concernent le monde carcéral que vous allez voter aujourd'hui, pour que le 31 juillet prochain, la prison de Vendée-le-Vieille puisse bien, dans ce nouveau régime carcéral-là, avec les 100 premiers narcotrafiquants, être la première des prisons de notre sécurité, de notre pays. Et c'est un point extrêmement important au moment où nous commémorons le 14 mai prochain le massacre d'Incarville et de l'assassinat des deux agents pénitentiaires tués lors de l'évasion de M. Ambra. Ce régime carcéral n'est pas complet et j'en m'en excuse auprès de l'Assemblée si je propose Deux amendements, mais qui sont en fait le même thème. Devant vous, la CMP, mais je m'en suis expliqué avec les parlementaires, puisqu'il me semble que dans la CMP, mais la présidente, je n'y étais pas, mais plusieurs témoins font un témoignage, comme dirait les magistrats, j'imagine. L'anonymisation des agents pénitentiaires, qui était prévue dans le texte, a été supprimée, je crois par erreur ou par difficulté, d'une longue et très et très fructueuse CMP. Donc avec le respect que je dois au Parlement, même si ce n'est pas la tradition du ministre que vous avez en face de vous, je proposerai deux amendements. Les deux concernent l'anonymisation des agents pénitentiaires pour qu'ils ne puissent pas mettre leur nom et leur prénom lorsqu'ils font leur travail d'agent pénitentiaire. Lorsqu'ils découvrent un téléphone portable en cellule, lorsqu'ils doivent prendre un certain nombre de dispositions, de mettre des gens par exemple dans un quartier disciplinaire, ils doivent mettre le nom le prénom de l'agent et donc évidemment ainsi subir des menaces personnelles sur leur famille, sur leur domicile et on retrouve qui sont ces personnes à l'extérieur et ça crée évidemment un climat d'insécurité extrêmement fort. Depuis très longtemps, ils demandaient l'anonymisation de la procédure en y mettant par exemple leur numéro de matricule comme nous l'avons fait tous ensemble en 2021 dans la loi que j'ai portée au ministère de l'Intérieur pour anonymiser les OPJ, les policiers qui faisaient les enquêtes sur les trafics de drogue notamment. Cette anonymisation qui a été prévue dans le régime carcéral de Vandaleuvel et de Condé-sur-Sarte a donc été supprimée par votre CMP, mais je crois en bonne intelligence que nous pourrions le revoter aujourd'hui. Et j'ai proposé, vu les difficultés que l'administration pénitentiaire connaît ces derniers jours, que nous ayons un deuxième amendement pour l'anonymisation générale. pour les maisons d'arrêt, pour tous les centres de détention, parce qu'il n'y a pas que dans les prisons de sécurité où l'administration peut être demandée. Ça peut être le cas de toutes les prisons, où évidemment l'agent met son numéro de matricule lorsqu'il fait son procès verbal. L'administration ou si jamais il devait y avoir une contestation, on puisse retrouver quelle est la personne qui, évidemment, a utilisé le pouvoir administratif qui était le sien sans mettre son nom et son prénom en pâture. Je pense que ces amendements peuvent être votés, me semble-t-il, très largement par votre assemblée, de bon sens, et c'est surtout un signe d'encouragement de l'administration pénitentiaire. Je veux dire Madame la Présidente, pour terminer par là, que oui, le Parquet National, et merci d'avoir trouvé un compromis sur la date, sera bien au 1er janvier au rendez-vous et nous pourrons, si vous le souhaitez, l'inaugurer ensemble. Ce sera une très bonne chose. Et oui, je pense qu'avec le travail que fait Monsieur le Ministre de l'Intérieur et le chef de FILA qui l'aura désigné, mais aussi les dispositions numériques et les dispositions techniques qu'il aura fait voter dans ces dispositions, nous aiderons à davantage interpeller à mettre fin à l'expansion du narcotrafique dans notre pays et à ne pas être comme d'autres pays qui nous entourent, la Belgique, les Pays-Bas. Aujourd'hui, dans la première fois, nous regagnons du terrain. Je crois que les attaques de prison des agents pénitentiaires le démontrent. Nous faisons pour la première fois extrêmement mal aux narcotrafiquants. On le doit au Sénat. On le doit à l'action de nos policiers, nos magistrats, nos greffiers, nos forces de l'ordre. Mais on le doit, me semble-t-il, à la nation tout entière qui, je l'espère, soutiendra ce texte ici et demain à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, chère Gérald, Madame la Ministre, chère Amélie, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et les Sénateurs, je crois qu'il y a peu de textes qui ont cette force-là et c'est un texte, j'ai déjà eu l'occasion de le dire le 4 février dernier, qui n'a rien de banal. Il n'y a rien de banal parce que c'est un texte vraiment, qui est un texte puissant, qui est un texte dans le domaine du régalien et qui est un texte qui vient du Parlement. c'est très très rare et ça fait très longtemps qu'un texte aussi important sur ce domaine régalien vienne notamment du parlement et d'une initiative sénatoriale. Je me souviens très bien l'origine, la commission d'enquête, les conclusions de la commission d'enquête, la reprise par Jérôme Durin et puis notre rapporteur de l'époque Etienne Blanc dans une PPL, et puis le vote à l'une annuité le 4 février. Bonne surprise aussi pour un vote à une très forte majorité à l'Assemblée nationale. C'était très loin d'être fait à l'époque, plus de 436 voix. C'était un vrai succès. un texte n'est pas banal parce qu'il est d'initiative parlementaire et d'initiative sénatoriale. C'est rare dans ce domaine et je voulais d'abord le souligner. Ce qui est rare aussi par les temps qui courent et dans la situation politique qui est la nôtre, c'est un texte très important à adopter dans Paris majorité, non pas au Sénat, à l'unanimité mais aussi à l'Assemblée nationale, ce qui veut bien dire qu'on peut transcender quand même l'éclivage partisan dès lors qu'on a des objectifs qui sont des objectifs qui concerne vraiment les intérêts fondamentaux de notre nation. Puisque le narcotrafic, vous l'avez, Madame la Présidente, indiqué tout à l'heure, c'est un mal qui est à la fois la cause racine de beaucoup de homicides, de cette hyperviolence que connaît notre société, mais à la fois qui est la cause d'un ébranlement de nos institutions, notamment, je pense, à travers les phénomènes de corruption. Et puis, je suis certain que c'est un texte qui marquera une rupture entre un avant et un après. La preuve, le ministre d'État, le garde des Sceaux vient d'en parler il y a quelques instants. Dans la matinée, nos forces de sécurité intérieures, sous l'autorité du PNA, du Procureur national antiterroriste, ont pu interpeller pas moins d'une trentaine de ce que j'appelle les narcos racailles. qui ont participé soit parce que c'était des petites mains ou soit parce que c'était des donneurs d'ordre à plus d'une centaine de faits qui ont visé précisément les établissements pénitentiels et aussi les domiciles de nos agents pénitentiels. Preuve que ce texte ce texte va déranger le milieu du narcotrafic. Nous leur avons déclaré la guerre et c'est la raison pour laquelle ils veulent aussi nous faire la guerre. Simplement avec le texte qui, j'espère, sera voté dans les mêmes circonstances, avec la même majorité, la même unanimité que le 4 février dernier, désormais nous avons un arsenal qui va tout changer. C'est pour ça que je dis qu'il y aura un avant et un après, puisque c'est l'Etat que nous allons totalement réorganiser. Le garde des Sceaux a parlé de la spécialisation de la chaîne judiciaire. Dans quelques semaines, je me rendrai à Nanterre où nous ouvrirons l'Etat-major qui va être chargé de la lutte contre la criminalité. Je vous rappelle que sur un même plateau, vous aurez les services de renseignement de quatre ministères, bien sûr le ministère d'intérieur, mais aussi celui de Bercy, mais aussi le renseignement pénitentiaire, donc la justice, et enfin la DGSE, ministère des Arnées. Donc sur le même plateau, vous aurez à la fois les services de renseignement et les services d'enquête, exactement comme nous l'avions fait pour l'État-major permanent, qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. Nous allons donc décloisonner l'État, L'information va circuler entre les ministères, entre les différents services, et en face de ces réseaux qui sont très structurés, qui sont très coordonnés, enfin nous aurons un État qui sera beaucoup beaucoup plus agile. Et puis une grosse mobilisation, une mobilisation nouvelle je crois, à la fois contre le blanchiment d'argent, mais aussi contre les phénomènes de corruption qui concernent aussi bien les emplois publics. Mais aujourd'hui, les emplois privés, nous n'avons voulu désigner aucune profession en particulier. Mais quand on voit la chronique médiatique, vous voyez bien qu'un certain nombre de procès, au moment même où je vous parle ici ou là, touchent à un certain nombre de professions, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient Et donc il fallait que, là encore, on ait un réarmement régalien contre le blanchiment, contre aussi ces phénomènes de corruption qui sont de plus en plus prégnantes dans la mesure où où les narcotrafiquants à la criminalité organisée charient des milliards et des milliards d'euros et de dollars. Et puis nous aurons aussi de nouvelles armes, des nouvelles armes pour nos services de renseignement, puisqu'aujourd'hui il faut adapter les nouvelles technologies d'interception, le satellite bien sûr, les algorithmes, mais ce sera un pas décisif que nous ferons et qui vont nous permettre d'avoir des nouveaux outils pour les services de renseignement qui sont au quotidien et qui luttent contre ces narcotraffiquants. Et c'est des criminels qui sont extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Et aussi un arsenal qui va nous permettre de donner, je pense à nos préfets par exemple. Et les élus vont être je pense satisfaits que les préfets par exemple puissent disposer d'un pouvoir d'interdiction de paraître sur un point de deal un narcotrafiquant. Qu'un préfet pourra se substituer à un bailleur social, à un bailleur privé pour faire les opérations d'exclusion du domicile et notamment dans un cas notamment de logement social. d'un arco archaïque qui est en train de pourrir la vie de l'ensemble de l'immeuble, faisant subir en réalité ses actes sur des habitants qui sont là, qui n'ont pas les moyens de déménager et qui doivent subir justement ce dérangement. De même que le préfet avait déjà des pouvoirs en matière de fermeture de commerce, notamment des débits de boissons. Mais nous allons étendre ces pouvoirs-là pour que des commerces qui sont aujourd'hui, on les sait parfaitement, des blanchisseuses, puissent être fermés. J'ai fait un certain nombre de déplacements. Je me souviens qu'à Belfort, le maire de Belfort me disait qu'il avait dû acheter pas moins de 30 commerces pour que ces commerces-là ne puissent pas retomber justement dans le trafic en devenant des blanchisseuses. Donc ce sera là encore important pour les élus d'avoir le soutien de l'État, le soutien de nos préfets. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, il y aurait tant de choses. Merci d'avoir compris à l'époque puisque c'était une initiative de la Commission et des auteurs de la BPL en matière de protection de notre personnel, notamment de ceux et celles qui peuvent avoir recours et qui posent les appareils, les techniques de renseignement. Nous avions donc ce dossier Corse qu'on appelle désormais le dossier distinct. Nous l'avons affiné progressivement. Nous l'avions soumise au Conseil d'État. Le Conseil d'État avait ratifié d'ailleurs les choix que nous avions fait ensemble, comme étant des choix qui permettaient l'efficacité de ce que nous recherchions, c'est-à-dire protéger notre personnel, sauver des vies humaines en réalité, sans atteindre nos grands équilibres constitutionnels, nos grands équilibres en matière de liberté publique. Voilà, en tout cas un immense merci. Je voudrais vraiment remercier celles et ceux qui ont participé à cette aventure, à tout ce parcours parlementaire, sénatorial, Jérôme Durin, Étienne Blanc, les sénateurs qui faisaient partie de la commission, j'en vois plusieurs ici, ceux qui ont porté la PPL et vous tous qui avez voté à l'unanimité le 4 février. J'espère que nous aurons ce même unanimisme. C'est important parce que non seulement nous aurons désormais des armes, un nouvel arsenal, mais plus encore nous avons une volonté. Je n'ai jamais dit, et personne ne l'a dit je crois au gouvernement, que ce combat contre les narcotrafiquants, contre la criminalité organisée, serait un combat facile. Et qu'en quelques semaines, qu'en quelques mois, juste après que le texte soit voté, nous parviendrions à éradiquer. à éradiquer. Je ne l'ai jamais dit. Je sais que ce sera long, mais on y parviendra. On y parviendra parce que désormais nous avons ces armes, cet arsenal, ce texte. On y parviendra parce qu'il y a désormais une volonté. C'est une volonté nationale, c'est la volonté des représentants du peuple français, quel qu'il soit, et notamment au Sénat, sur quelques sièges que vous siégiez et je pense que ça c'est fondamental ça donne une force à la république et à la france en tout cas merci d'avoir compris et merci de réserver vos votes comme le 4 février pour donner le maximum de force à ce texte Merci monsieur le ministre la parole est à madame amélie de montchalin ministre chargé des comptes publics Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Gardesso, cher Gérald, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, cher Bruno, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Sénatrices, Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler ici devant vous, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, et devant nos députés, la lutte contre le narcotrafique et contre la criminalité organisée, est une priorité absolue du gouvernement et le Premier ministre l'avait d'ailleurs souligné lors de sa déclaration de politique générale en rappelant combien chaque jour l'actualité nous montre l'intensité de la menace que constitue cette criminalité organisée. Vous savez mon attachement en premier lieu en tant que ministre des Comptes publics à la situation budgétaire de notre pays et nous ne pouvons pas tolérer cette perte de recette fiscale et le détournement d'argent public lié à cette criminalité. Mais je suis également, vous le savez, la ministre des douanes et plusieurs services de Bercy concourent à la lutte contre la criminalité organisée, aux premiers chefs desquels nous pouvons compter deux centrales du renseignement du 1er cercle, que sont la DNRED, direction de renseignement de la douane, et TRACFIN, mais également la direction générale du Trésor, notamment en matière de sanctions et de lutte contre la criminalité financière. Nous avons fait le vœu de ne pas avoir la main qui tremble face à ces criminels et de nous donner collectivement les moyens d'agir pour lutter contre ces trafics. C'est d'abord grâce à vous, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, madame la présidente, vous qui avez pris l'initiative de cette proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafique et je vous en remercie très sincèrement. C'est aussi grâce au travail collaboratif que nous avons pu avoir pour identifier les besoins des services et leurs contraintes et coller à la réalité du terrain pour penser un corpus législatif qui soit le plus adapté à cette menace nouvelle ou du moins nouvelle par son ampleur. Il vient ainsi récompenser le travail considérable qui est accompli par les services de Bercy dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et la criminalité organisée, le blanchiment et les flux financiers illicites. Je tiens, une fois encore, et ce n'est évidemment que mérité, à saluer la très grande mobilisation et l'engagement sans relâche, chaque jour, à chaque heure, de la douane, de traque-fin, de la direction générale du Trésor pour lutter contre ce fléau, qui collaborent avec les services évidemment de police judiciaire et l'autorité judiciaire pour inscrire leurs actions en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants et contre le blanchiment dans le cadre interministériel du plan national de lutte contre les stupéfiants. La proposition de loi permet de renforcer significativement les pouvoirs d'action de mon ministère pour entraver et bloquer les flux, la logistique et l'enrichissement financier des trafiquants. Je voudrais ici rappeler quelques mesures qui nous semblent particulièrement importantes à relever. D'abord, la création d'un dispositif de gel administratif des avoirs des narcotrafiquants, dit le GABAN, comme il était déjà possible de le faire en matière de terrorisme, pour bloquer l'accès aux financements en complément de l'action judiciaire dans les cas de fuite ou pour l'élargir aux actions des personnes de l'entourage, des personnes impliquées et aux structures écran. Ensuite, cette proposition de loi va permettre d'interdire aux fournisseurs de services sur actifs numériques de proposer des comptes anonymes ou des mixeurs de cryptoactifs qui, on le sait, sont des vecteurs majeurs de blanchiment des revenus issus des trafics de suffiants. Cette proposition de loi permettra également à traque fin d'avoir accès au système d'immatriculation des véhicules, le SIV, pour élargir leurs enquêtes patrimoniales. De plus, en élargissant la présomption de blanchiments douaniers aux évolutions technologiques, et notamment aux crypto-monnaies, nous pourrons mieux suivre tout ce qui concourt à opacifier les transactions financières. Cette proposition en loi également permettra aux lanceurs d'alerte d'adresser des signalements à trac fin. Grâce à vous, sur proposition du gouvernement lors des débats, plusieurs mesures visant à renforcer la répression du blanchiment et à entraver les criminels ont été adoptées. Néanmoins, je veux le dire ici, je regrette que certaines mesures très importantes pour les douanes n'aient pas pu être retenues à l'issue de la CMP, qui constituait pourtant de véritables avancées pour les douaniers. Je pense en particulier à la disposition qui devait permettre aux agents de la douane d'avoir accès systématiquement aux données de certains opérateurs privés dans les secteurs des transports et la logistique dont la portée a été très largement atténuée. Je pense également à la possibilité qui avait été votée je crois à l'unanimité nos deux chambres de permettre aux agents des douanes spécialement habilité de pouvoir appréhender des criminels en autorisant les visites domicilières après 21h sur ordonnance du juge des libertés de la détention dans les cas de flagrance visite qui était permise au sein des locaux d'habitation et hors flagrance pour les locaux qui ne sont pas à usage d'habitation Il y a donc tant encore à faire et j'appelle donc de mes voeux que nous ayons très prochainement la possibilité d'en discuter à nouveau car je sais votre attachement à nos douaniers, au travail qu'ils font et vous savez que leur implication au quotidien et leur rôle en matière de lutte contre les stupéfiants et de criminalité organisée est majeure. Je rappelle ici que 70% des stupéfiants qui sont saisis dans notre pays le sont par les douaniers. Je vous remercie donc une nouvelle fois pour l'ensemble de ce travail. Les progrès sont inédiables et la bonne nouvelle, c'est que nous avons encore du travail devant nous. Vous pouvez donc compter sur notre mobilisation aujourd'hui. Cette mobilisation est nationale. Le fléau, nous le combattons et l'action, nous n'arrêterons pas de la mener. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements présentés ou acceptés par le gouvernement, puis par un seul vote sur l'ensemble de chacun de ces textes. En conséquence, les amendements seront mis au voie, puis le vote sur les articles sera réservé pour chacun de ces textes. Nous passons à la présentation puis au vote des amendements du gouvernement sur la proposition loi visant à sortir la France du piège du narcotrafique et nous débutons à l'article 3 par un amendement numéro 6 présenté par le gouvernement. Excusez-moi,

C'est pas le bien, si je peux me permettre. Je pense que c'est monsieur le ministre de l'Intérieur, les fermetures administratives de commerce, si je peux me permettre. C'est rédactionnel, donc ce sera très bref. Et à quel avis de la Commission sur cet amendement du gouvernement ? Je mets au voie cet amendement numéro 6 avec un avis favorable de la Commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 6 est adopté. Nous passons à l'amendement 3. C'est une coordination rédactionnelle et ça permettra donc avec les présidents qui sont apportés de le rendre encore plus robuste en matière de constitutionnalité. Quel avis de la Commission ? Favorable. Un avis favorable du rapporteur pour la Commission. Je mets au voie qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 3 est adopté. Je place sur l'article 4bc avec un amendement numéro 5 du gouvernement. Je le présente ici parce que j'ai du mal à passer de l'autre côté. Merci Monsieur le Président. Il s'agit d'une levée de gages pour permettre de financer et de soutenir la disposition prise dans cet article. Merci Madame la Ministre. Quel est l'avis de la Commission Monsieur le Rapporteur ? Favorable. Je vais mettre au voie cet amendement 5 qui a reçu un avis favorable de la Commission, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 5 est adopté. Nous passons à l'article 15bis B avec un amendement numéro 1. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit, et fait du gros gélis pendant mon discours introductif, de pouvoir anonymiser ce qu'on appelle ici pseudonymiser le travail des agents pénitentiaires. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de ne pas savoir qui a fait quoi dans une cellule, mais de pouvoir mettre un nom de code, en l'occurrence numéro de matricule, pour que l'administration sache qui fait quoi, s'il devait y avoir recours, mais ne met pas le nom et le prénom des agents pénitentiaires lorsqu'ils font leur travail, parfois difficile, de discipline à l'intérieur des prisons. prisons. Le ministre, quel est l'avis de la Commission, M. L'Importer ? C'est un avis favorable, c'est un amendement qui concerne la pseudonymisation des agents de l'administration pénitentiaire. C'est un aspect qui est transversal à tout le travail de la Commission d'enquête, à toute cette proposition de loi. Et il se trouve qu'il manquait cette petite touche, cette petite pierre, et donc il nous paraît très important qu'on puisse, notamment dans le contexte particulier qu'on vit en ce moment, étendre ce régime aux agents de l'administration pénitentiaire. Monsieur le rapporteur, je mets au voie cet amendement 1 qui a reçu un avis favorable de la Commission. Qui est pour Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement est adopté. Passons à l'article 19, un amendement numéro 8 de la Commission. C'est un amendement de coordination. Quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement ? Il y a l'accord du gouvernement. Donc c'est un avis favorable. Je mets au voie cet amendement 8 qui est pour ? Qui s'abstient ? L'amendement est adopté à l'article 22, un amendement du gouvernement. Amendement rédactionnel sur des enjeux portuaires. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis favorable de la Commission, qui est pour ? qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est adopté. L'article 23 quinquesse un amendement numéro 2 du gouvernement. Monsieur le ministre. sur les prisons de haute sécurité. On en fait donc deux, en espérant que le Conseil constitutionnel retienne les deux. Merci Monsieur le Ministre. Quelle est l'avis de la Commission Monsieur Laporta ? Par Par cohérence avec l'avis favorable émis sur le précédent, nous émettons un avis favorable sur cet amendement. Je mets au voie cet amendement 2 qui a reçu un avis favorable de la Commission, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est adopté. L'article 26, c'est un amendement 4, rectifié bis Monsieur le Ministre. Oui, je Oui, je me fais par parole Monsieur le Ministre des Outre-mer pour une coordination ultramarine. Merci Monsieur le Ministre. Quelle est l'avis de la Commission sur cet amendement ? C'est effectivement l'amendement de coordination, c'est favorable. Je mets au bout à cet amendement qui a reçu un avis favorable de la Commission, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 9 de la Commission présentée par Mme la Présidente. Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle, comme vous pourrez le lire sur l'amendement. Donc c'est avec l'accord du gouvernement, donc c'est un avis favorable, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Donc je mets au voie cet amendement de la Commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Nous passons... Nous avons terminé. Aucun amendement n'a été déposé sur la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée. Nous passons donc aux explications de vote commune des groupes à raison d'un orateur par groupe. Nous débutons avec Mme Laura Darkos pour le groupe Les Indépendants, République et territoires. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres d'État, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, Les drogues menacent notre société, elles mettent en danger nos valeurs et sapent nos institutions, elles tuent nos enfants. Voilà ce que déclarait le Président Reagan en 1986 et s'alarmer alors de la prolifération de la cocaïne et d'une nouvelle épidémie, le crack. La tendance américaine d'hier est hélas devenue la nôtre aujourd'hui. Le marché de la cocaïne dans notre pays, avec plus d'un million de consommateurs réguliers, avoisine des 3 milliards d'euros. Tous nos territoires sont désormais concernés. Nous avons eu l'occasion de dire que la drogue tue, qu'elle n'est pas une infraction sans victime. Il y a bien sûr les décès liés à des surdoses ou la toxicité des produits, mais il y a aussi toutes les victimes des cartels. Les trafiquants menacent, extorquent, enlèvent, frappent, mutilent et assassinent. Enfin, la drogue joue un rôle dans certains passages à l'acte et provoque aussi des accidents. C'est le cas de 20% des accidents mortels sur nos routes. Nous n'oublions jamais que derrière ces petits sachets, il y a des victimes et des familles endeuillées. Les Etats-Unis sont à présent confrontés au Fentanyl, dont le prix est aussi dérisoire que les effets sont puissants. Cette nouvelle drogue a transformé les centaines de milliers d'Américains en véritables zombies. Beaucoup n'y survivront pas. Nous devons tout faire pour que cette situation ne devienne pas celle de la France de demain. La drogue est le terreau fertile de la criminalité et ceux qui soutiennent cette proposition de loi l'ont bien compris. Les mesures de ce texte, que notre groupe salue d'autant plus qu'il est issu des travaux du Sénat, visent ainsi à porter un coup d'arrêt à la criminalité organisée sur nos territoires. Lors de nos débats, certains ont pu douter de l'efficacité des dispositions proposées, tout en avançant l'idée que le meilleur moyen de lutter contre les trafics consisterait à renforcer les aides sociales. Ces jours derniers, tout le monde a pu constater qu'il s'était lourdement trompé. La violence des attaques portées contre les personnels pénitentiaires et les centres de détention traduent la pertinence des mesures envisagées. C'est bien parce que les trafiquants savent que la loi sera efficace qu'ils réagissent aussi violemment. Le groupe Les Indépendants tient à redire tout son soutien au personnel pénitentiaire, à nos forces de sécurité intérieures ainsi qu'à leurs familles. La République doit continuer à protéger ceux qui nous protègent. Force doit rester à la loi. En cohérence avec l'approche globale du texte, Un parquet national de lutte contre la criminalité organisé est institué. Il sera notamment chargé des crimes les plus graves comme les homicides ou l'organisation de réseaux criminels. A ce titre, nous saluons la création de l'infraction de concours à une organisation criminelle inspirée du droit pénal italien anti-mafia. Il s'agit d'une mesure pragmatique qui permettra la poursuite de tout individu appartenant à une bande ou à un gang. Les têtes pensantes des trafics veillent à se tenir bien éloignés du terrain et des points de deal. Néanmoins, grâce aux améliorations apportées au statut de repenti, ainsi qu'au développement de l'infiltration, les services vont accroître les renseignements dont ils disposent sur ces organisations. Les poursuites judiciaires pourront atteindre le haut de leur hiérarchie et être donc plus efficaces pour paralyser ces trafics. Plusieurs dispositions permettront également de fermer les établissements concurrents au blanchiment, mais aussi de geler les avoirs des trafiquants. A cet égard, le groupe les indépendants rappelle son attachement au caractère judiciaire des procédures. Ce n'est qu'à cette condition que l'autorité judiciaire peut remplir la mission qui lui est conférée par notre Constitution, être la gardienne de la liberté individuelle. Afin que la justice soit plus efficace, il vaut mieux augmenter son budget que promouvoir des procédures administratives, Madame la Ministre. Dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons, notre groupe a toujours affirmé que priorité devait être donnée aux régaliens. Le groupe Les Indépendants soutient l'objectif de lutte contre la criminalité organisée, particulièrement en s'agissant de la drogue. Nous voterons donc à l'unanimité en faveur de l'adoption de ces propositions. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux,

Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Madame la Ministre chargée des comptes publics, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Nous venons d'aboutir en commission mixte paritaire un accord que je qualifierai de ferme, lucide et responsable. Un accord ferme, clair, sans ambiguïté, La République reprend la main face aux narcotrafiquants, un accord qui marque sans conteste une avancée décisive dans la lutte contre le narco-banditisme qui gangrène nos quartiers, pervertit nos institutions et menace l'autorité de l'État. Je tiens d'abord à saluer le travail de la Commission d'enquête du Sénat à l'origine de cette proposition de loi et tout particulièrement Jérôme Durin et Etienne Blanc, grands artisans dans une démarche transpartisane de ce texte majeur et que je qualifierais d'historique, saluer également l'écoute du gouvernement, qui a su écouter, qui a su dialoguer et surtout tenir bon car il fallait beaucoup de courage pour porter ce texte ambitieux dans un climat souvent miné par l'idéologie ou encore ou encore le déni. Et le Sénat a su peser dans toutes les discussions, nous avons su obtenir des garanties et nous avons obtenu gain de cause. Ce texte, c'est d'abord et avant tout un signal. Un signal envoyé aux Français qui ne supportent plus l'impuissance publique. Un signal envoyé également aux trafiquants qui doivent comprendre que la République ne reculera plus. plus. des mesures chocs avec des mesures phares, nous passons d'une logique de tolérance à une logique de dissuasion. C'est une rupture et c'était une nécessité. soyons lucides, le trafic de drogue n'est plus ni un simple fléau sanitaire ni un simple fléau social. C'est un véritable système mafieux, structuré, militarisé, qui infiltre nos cités, notre économie, notre culture parfois. Il s'agit d'un défi d'autorité, d'un défi civilisationnel. L'accord trouvé En commission mixte paritaire, sur la loi contre le narcotrafique n'est pas un simple consensus parlementaire. C'est un signal politique clair, net et attendu. Attendu par tous les Français qui n'en peuvent plus de voir la République reculer face à des narcos de mafia qui dictent leurs lois dans nos rues, dans nos quartiers, parfois jusque dans nos institutions. Je le dis avec gravité, mais aussi avec une certaine fierté, cette loi incarne un tournant, un changement de paradigme, la fin de l'annévité, le retour de l'autorité. Ce texte consacre une ligne de fermeté que nous réclamions depuis des années, car il y a ceux qui parlent de liberté individuelle, individuelle quand il s'agit de consommer de la drogue. Moi, je préfère parler des mères de famille qui pleurent leur fils abattu dans un point de deal. Je parle des enfants qui traversent un hall d'immeuble infesté de guetteurs armés. Je parle de la République qui a été humiliée, qui a été agenue. Nous avons tenu la ligne. Cette ligne qui assume l'ordre, qui assure la sécurité, la souveraineté, Une ligne qui ne s'excuse pas, qui ne relativise pas, qui agit. Il n'y a pas de République sans courage. À ceux qui s'inquiètent de la fermeté du texte, et ils sont peu nombreux au Sénat, je leur réponds que la vraie violence, c'est l'inaction. Et à ceux qui nous accusent de vouloir faire peur, je réponds oui. Il faut faire peur. Il faut que les trafiquants aient peur. Peur de la justice, peur de la prison, peur de perdre ce qu'ils ont volé à la République. Il faut que la peur change de camp. Ce texte n'est pas une fin, c'est un début, un socle, un acte de reconquête, reconquête de nos quartiers, de notre souveraineté, de notre pacte républicain. La République est de retour. Elle parle fort, elle frappe juste et elle ne tremblera plus. Nous, les Républicains, nous voterons bien évidemment ce texte avec détermination, car il n'arcarne ce que nous devons à la France, la volonté de protéger, la force de rétablir l'ordre et la fierté d'être exigeants. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame Marie-Laure Finérat-Hort pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur les Ministres, Madame le Rapporteur, Monsieur le Rapporteur, Chers collègues, Depuis délustre, une guerre fait rage sur le territoire français. Une guerre qui fait de nombreuses victimes, souvent collatérales. Une guerre sournoise, souterraine qui se passe à l'abri des regards. Une guerre qui n'est pas classique avec des chars et des bombes. Une guerre menée par des réseaux organisés, puissants qui infiltrent nos quartiers, nos écoles, nos familles. Il nous revient aujourd'hui de doter la France d'un nouvel arsenal législatif à la hauteur des enjeux pour mieux agir en première ligne de cette guerre. Vous le savez, la Commission mixte paritaire qui s'est réunie le 10 avril dernier a été conclusive. Face aux conséquences graves qu'aurait l'inaction dans ce combat, que nous partageons tous sur ces bons, Nous nous réjouissons que nous ayons trouvé un compromis sur ce texte et qu'il puisse rapidement aboutir. Au Sénat, nous avons défendu une approche ferme, réaliste et cohérente face à l'ampleur du fléau qu'à le narcotrafic. Je me félicite que le texte issu de la CMP préserve le travail que nous avons mené dans cet hémicycle. Je pense notamment à la création d'un Parquet national anti-criminalité organisé qui permettrait d'apporter des réponses judiciaires plus cohérentes et centralisées. Il en va de même pour le gel administratif des avoirs des narcotrafiquants, qui offrira au pouvoir administratif une action complémentaire aux procédures existantes en matière judiciaire. Aussi, je pense à l'article 15-terre, car j'avais déposé au nom de mon groupe un amendement visant à activer à distance les appareils fixes connectés sous le contrôle du magistrat. Ce développement des techniques d'enquête est indispensable afin de lutter efficacement et contre le narcotrafique Je souhaite saluer ici le centre des responsabilités dont en fait preuve des députés en adoptant ce texte à une large majorité. A mon sens, il est indéniable que la navette parlementaire a permis d'enrichir ce texte et les ajouts en provenance de l'Assemblée nationale sont nombreux et bienvenus. Je pense entre autres à l'article d'Hister, qui renforce des sanctions à l'encontre des trafiquants impliquant des mineurs dans leur réseau. C'est une avancée que je salue, car elle répond à une réalité tragique que nous connaissons bien. Mais comme je l'ai déjà dit ici, le texte reste silencieux sur la question de la prévention, pourtant essentielle pour protéger durablement nos jeunes. Dans les territoires ultramarins, comme la Guyane, que j'ai l'honneur de représenter dans cet hémicycle, le narcotrafique est une menace quotidienne. Il gangrène nos territoires, déstabilise notre jeunesse. Comment espérer gagner cette guerre, quand tant de jeunes n'ont d'autre choix que d'avaler des boulettes pour payer des loyers en retard ou soutenir leur famille ? La Guyane, désormais rejointe par la Martinique et la Guadeloupe, est devenue, malgré elle, un passage obligé pour les trafiquants. Aussi, je tiens à réaffirmer avec la plus grande fermeté qu'il est nécessaire que le gouvernement assume pleinement ses responsabilités en matière de contrôle aux frontières. Nous le savons, en dépit des contrôles renforcés au départ, des mules parviennent toujours à atterrir dans les aéroports parisiens. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à l'État. Il est urgent d'installer des scanners à Orly et à Roissy. Il s'agit d'une mesure simple, concrète, attendue de longue date et déjà mise en place par nos voisins belges et hollandais pour des liaisons très spécifiques. Cette avancée permettrait de briser un maillon essentiel de la chaîne logistique des trafiquants. Malgré ces quelques réserves, vous l'aurez compris, mon groupe soutient largement les progrès apportés par ce texte pour sortir la France du piège du narcotrafique. Enfin, je veux redire toute ma fierté d'avoir modestement apporté mon concours à l'élaboration d'un texte qui fera date. C'est avec fierté que j'ai mené ce combat aux côtés d'Etienne Blanc et Jérôme Durin depuis les travaux de la Commission d'enquête pour doter la France d'un outil à la hauteur de la lutte contre les narcotrafiquants. Et c'est pourquoi le groupe RDP votera en faveur de cette proposition. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre chargée des Comptes publics, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le rapporteur, Madame la présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Je souhaite souligner que cette proposition est une manifestation de la qualité de l'initiative parlementaire particulièrement sénatoriale. Par la co-construction et le dialogue entre les chambres et avec le gouvernement, sur la base d'un travail important de fonds issus de la commission d'enquête menée par Étienne Blanc et Jérôme Durin, que je salue, nous arrivons à la fin de la procédure législative avec un texte conséquent très majoritairement accepté. Sur le fond, il n'est plus nécessaire, après les nombreux débats qui ont animé notre Parlement, de rappeler la prégnance du sujet abordé par cette proposition de loi. Je prends pour témoignage l'écho qu'elle a reçu dans le débat public et médiatique. Les Français, leurs élus, les professionnels du droit, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie et les pénitentiaires connaissent désormais trop bien la réalité que représente un narcotrafique d'ampleur et du quotidien. Le rapport duquel fut lancé cette initiative faisait la lumière sur l'étendue géographique de la problématique qui n'est plus réservée au centre urbain, mais touche maintenant fortement le monde rural. Le trafic de drogue ravage tout sur son passage, désespoir des jeunes enrôlés aux vies des victimes de la violence des bandes. C'est pourquoi il faut saluer que le législateur puisse rendre plus efficace les moyens répressifs de la lutte contre le trafic de drogue. Mais parce que le trafic de drogue est désormais un fait de société, la répression ne suffira pas elle seule à régler le problème. Il faut renforcer également notre ambition en matière de prévention indispensable à la réduction de la consommation et donc au trafic. Plus globalement, le narcotrafique se nourrit. de la vulnérabilité sociale, économique, financière ou sanitaire de certains citoyens. Des outils cruciaux doivent être développés en matière de cohésion sociale, de protection de l'enfance, d'éducation, d'insertion et de réinsertion. La lutte contre le narcotrafique est un combat pour une société meilleure. Elle concerne et mobilise tous les citoyens. pas seulement les forces de l'ordre et la justice, mais également les assistants sociaux, le monde associatif, les soignants, les élus locaux. La majorité des dispositions de la composition de lois fait l'objet d'un large consensus transpartisan et entre les chambres. Parquets spécialisés, nouveaux régimes carcérales d'isolement, mesures repressives et outils pour les enquêteurs comme leur enseignement algorithmique ou la surveillance à distance sont parmi les mesures attendues et nécessaires. Je prends en acte que la Commission mixte paritaire a entériné la suppression de l'article 8R qui permettait l'accès des services de renseignement au contenu des messageries chiffrées. Elle a également conclu au maintien de l'article 16 bis autorisant les dispositifs de surveillance dans les lieux privés ainsi que des dispositions concernant le procès verbal distinct. Ces mesures doivent appeler à la vigilance, tout comme l'application du dossier qu'offre, qui devra être évaluée pour s'assurer que l'atteinte au droit de la défense est proportionnée. Bien que je me satisfasse du consensus trouvé à l'endroit de l'article 16, n'oublions pas qu'il constitue une atteinte importante au droit fondamental et fragilise ainsi l'équité du procès et, in fine, la justice elle-même. Or, la justice a besoin d'être forte aujourd'hui plus que jamais et doit pour cela être fondée sur le respect des droits. Il en va de même pour les forces de l'ordre qui se doit confier des pouvoirs importants dérogatoires aux droits communs à l'image du droit d'exception antiterroriste. L'exercice de ces prérogatives doit s'accompagner de moyens humains et financiers à la hauteur pour garantir un cadre de travail serein qui limitera les risques de non-respect du droit, d'erreur ou d'abus. En définitive, le groupe RDSE s'inscrit à l'unanimité en faveur de cette proposition de loi dont nous espérons qu'elle portera ses fruits pour lutter contre ce fléau du narcotrafique. La satisfaction de ce travail accompli ne doit pas nous voiler la face sur le chemin qui reste ensemble à parcourir. Merci. La parole est à madame Isabelle Floren pour le groupe Union Centriste. Monsieur le Président, messieurs, madames et messieurs les ministres, madames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les conclusions de la Commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafique sont sans nul doute le fruit d'un bon accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle reste dans la lignée du consensus qui s'est dégagé sur ce texte ici au Sénat le 4 février dernier et valide le travail accompli par la commission d'enquête sénatoriale présidée par Jérôme Durin et dont le rapporteur était Étienne Blanc. Nous ne pouvions pas objectivement rester inactifs face à l'ampleur des changements de méthode et de comportement des trafiquants de drogue. Comme l'a déclaré dans la presse M. Philippe Marna, l'ancien directeur de la lutte contre la criminalité organisée, les responsables des trafiques sont avant tout des logisticiens qui adaptent en continu leur mode opératoire à la réponse policière et douanière. Mais au-delà de cette flexibilité technique, l'usage de la violence et la volonté de tuer sont devenus monnaie courante si j'ose user de cette expression face au terrible nombre de victimes directes et indirectes qui sont désormais touchées par les agissements des nervis obéissant aux ordres meurtriers de leurs chefs. Dans cette course folle et effrayante où tout semble permis, notre pays est particulièrement exposé car il est à la fois un large bassin de consommation et un pays de transit, voire de rebond, vers des pays lointains où les prix des stupéphans, notamment celui de la cocaïne, sont très élevés, tel l'Australie, très distante de la France. Heureusement, l'engagement de l'ensemble de nos forces de l'ordre, de nos magistrats et du personnel judiciaire qui les entourent, que je tiens à saluer ici, est tel que nous faisons face vaillamment. Mais nous devons leur permettre de s'adapter, car nous sommes donc entrés dans une ère nouvelle. Le texte qui ressort de la CMP est multidimensionnel, combinant réponse immédiate et stratégie de long terme tout en cherchant un équilibre entre efficacité répressive et respect des libertés individuelles. Les mesures clés qui ont été adoptées ont pourtant fait l'objet de nombreux débats depuis des années. L'une des questions centrales est de savoir si les règles prises en matière de lutte contre le terrorisme pouvaient être transpose à la répression du trafic de drogue. Aujourd'hui, l'adoption de ce texte permettra d'apporter une réponse claire et positive à cette interrogation. Ainsi, un parquet national anti-criminalité organisé à l'instar du parquet national anti-terroriste va voir le jour en janvier 2026. Il en va de même avec la création de quartiers de haute sécurité pour les gros trafiquants et l'instauration d'outils de coercition contre les filières de blanchiment de l'argent et de la drogue. Deux autres innovations attendues depuis longtemps ont été également adoptées. Il s'agit de la réforme des repentis par la création d'une réduction de peine pouvant atteindre les deux tiers pour les collaborateurs de justice et de la création d'une nouvelle infraction, dite concours à une organisation criminelle. Des points de tension ont été résolus, enfin, entre nos deux assemblées. Ainsi, les fermetures administratives d'établissements participants au blanchiment de l'argent ne seront que du ressort exclusif du préfet. Les maires n'auront pas cette compétence, évitant ainsi qu'il soit l'objet de pression. La durée maximale de l'isolement carcéral un quartier de haute sécurité a été également réduite de deux ans à un an renouvelable. Enfin, la disposition controversée obligeant les plateformes à communiquer les correspondances a été abandonnée. Ce texte répond à des impératifs sécuritaires via un système de limitations proportionnées répondant en cela à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui appelle à ce que les restrictions de liberté publique soient nécessaires, adaptées et proportionnées. Pour terminer, je voudrais dire qu'en adoptant ce texte, nous allons montrer notre détermination à lutter contre le crime organisé. Nous allons également réaffirmer que l'État de droit est plus fort que les mafias.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Nous connaissons désormais bien la réalité et les conséquences du trafic de drogue. Dans ma ville, Marseille, ces habitants sont hélas souvent les premières victimes. Si nous savons l'horreur de cette gangrène mafieuse, nous ne pouvons ignorer qu'elle prospère sur la misère. Pourtant, la France, septième puissance du monde, Nous comptons plus de 9,1 millions de pauvres, soit plus de 14% de la population. Et alors que ces mafias sanguinaires exploitent de plus en plus d'enfants, dans notre pays, un enfant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Les plus précaires, les plus fragiles sont toujours les premières victimes de ces mafias. Et pourtant, alors que les enfants de l'aide sociale à l'enfant sont particulièrement exposés à cet esclavage, oui, j'ose le mot, la puissance publique défaillante fait des économies sur leur dos, les abandonnant aux mains de ces criminels. Ce que je souhaite exprimer ici, mes chers collègues, Alors que nous apprêtons à adopter définitivement cette proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafique, c'est que ce piège est multidimensionnel. Et lutter contre ce narcotrafique, c'est aussi lutter contre les causes de ce chaos que nous organisons en laissant la pauvreté prospérer, les inégalités sociales et économiques exploser et en abandonnant les plus précaires. J'espère que l'intérêt que nous portons sur ce texte sera étendu à un réel combat pour plus d'égalités, sans quoi notre combat sera vain. Si la sécurité est un droit fondamental que l'Etat se doit d'assurer, elle ne peut se faire sans un système plus égalitaire. Et à ce titre, une réelle politique globale de santé publique pour lutter contre la consommation de drogue est aussi primordiale. Sans ces efforts, la loi que nous votons aujourd'hui ne permettra pas de lutter réellement contre le trafic de stupéfiants et contre ces mafias. Toujours par souci de cohérence, je souhaite aussi attirer notre attention sur notre justice qui reste bien moins financée que chez nos voisins européens et plus particulièrement sur le juge des libertés et de la détention. Afin de mieux protéger les habitants de ce pays, cette proposition de loi inscrit dans notre droit des mesures privatives de liberté individuelle. La recherche d'équilibre entre nos droits fondamentaux conduit, dans un état de droit comme le nôtre, à mettre en place des verrous et des garanties de contrôle. A ce titre, nombreuses sont les dispositions de cette loi qui font reposer ces contrôles sur le juge des libertés et des tensions. Pourtant, alors qu'au fil des lois, on ne cesse de faire reposer sur les épaules de ces juges toujours plus de responsabilités, en leur demandant d'y répondre toujours plus vite, les moyens mis en place pour leur permettre d'exercer correctement ces missions sont défaillants et ne répondent pas ne répondent en rien aux besoins immenses. La justice française est paupérisée. Or, sans moyens et conséquences supplémentaires, les juges des libertés de la détention ne pourront pas exercer leur mission. Le contrôle indispensable qu'ils exercent ne pourra alors plus garantir le respect des droits fondamentaux. L'état de droit n'est pas qu'une idée, qu'un idéal. Il doit être une réalité pratique pour laquelle nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il soit effectif. Enfin, ce texte nous appelle à la plus grande vigilance. Nous touchons ici aux droits fondamentaux et nous devons prendre garde toujours à trouver un équilibre indispensable. La création des quartiers sécurisés en prison par l'article 23 de cette proposition de loi présente des risques que nous souligne également la défenseur des droits. Nous devons en effet mesurer ce qu'implique une telle disposition et rester vigilants. Ensuite, la mise en place de peine complémentaire d'interdiction de vol pour les mules interceptés et condamnés pourrait avoir des conséquences graves sur des personnes déjà précaires et en situation de quasi-esclavage. Enfin, l'article 22 instaure de nouvelles mesures relatives à la lutte contre le trafic de drogue dans les ports. Or, mon groupe et moi-même avons à cœur depuis le début de l'étude de ce texte de nous assurer de la sécurité des travailleurs de nos ports, mais aussi de la préservation de leur liberté fondamentale. Si des garanties ont été instaurées, nous restons vigilants quant à la mise en application de ces contrôles accrus. Ainsi, malgré ces mises en garde émises et la vigilance importante que nous continuerons à avoir sur le respect de notre état de droit, Notre groupe convaincu que la lutte contre les mafias et le trafic de stupéfiants s'intègrent dans un projet de développement économique, social, démocratique et populaire votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Guy Benaroche pour le groupe écologiste Solidarité des territoires.

Monsieur le Président, messieurs les ministres d'État, messieurs les auteurs et rapporteurs, chers membres de la mission de la formation sur le narcotrafique, chers collègues, nous voilà arrivés au bout du chemin législatif pour cette proposition de loi issue des travaux de notre assemblée. Ces travaux qui, dans leur approche, avaient recueilli l'unanimité, car les recommandations étaient claires, de la lutte contre le blanchibar à la réorganisation de notre arsenal pédale, mais aussi avec un volet sur la prévention forcément indispensable. L'idée n'était pas d'être méchant avec les méchants, mais de taper au portefeuille et de s'attaquer au haut du spectre. Le rapport de notre commission d'enquête sénatoriale comprenait de nombreuses recommandations, 35, dont beaucoup ont été reprises, afin en fait de changer de doctrine et de ne pas viser que le consommateur et les petites mains des réseaux. Réseaux qui génèrent de gigantesques profits par la vente de stupéfiants, mais opèrent aussi dans les trafics d'armes, le racket, la traite des êtres humains, le proxénétisme. De cette unanimité, que reste-t-il dans ce texte issu de la CMP ? Cette globalisation des groupes organisés au-delà de la vente de drogue a été prise en compte en spécialisant nos moyens de justice au travers d'un parquet national non limité au sol stupéfiant, mais pour l'ensemble de la criminalité organisée. Notre groupe salue cette vision à la juste échelle de ces nouvelles mafias et de la nécessité d'y accorder une attention particulière. Nous alertons quand même sur la dérive possible de centralisation excessive, mais nous devons être conscients que ces criminalités se retrouvent sur l'ensemble du territoire, en zone urbaine comme en zone rurale. Notre groupe s'associe à la volonté nouvelle de s'attaquer au haut du spectre, au blanchiment, à la corruption. C'est bien la raison qui nous a poussé en première lecture, malgré certaines réserves, à voter le texte. Car le constat premier de la Commission d'enquête, c'est aussi celui de l'échec de politique des places nettes des opérations XXL. Plus de saisies, plus de personnes en prison et pourtant un trafic qui continue d'augmenter. Reste que ce texte, aussi ambitieux soit-il, la suite question primordiale en suspens. Quels sont les moyens réels qui seront affectés par ce gouvernement pour mettre en œuvre vite et efficacement ces avancées ? Il y a quelques années, nous avions créé une Jules-Alcaud. Je ne ferai offense à personne en disant que la machine n'a que trop peu fonctionné, en raison justement d'un manque de soutien autant politique que matériel, financier en ressources humaines. Là, nous allons voter et prendre des dispositions qui coûtent de l'argent et qui nécessitent de nouveaux moyens humains dans un contexte où il semble, en tout cas on nous le dit, que nous n'en ayons pas les moyens avec l'état dans lequel se trouve nos finances publiques. Il y a du bon doc, mais il y a aussi des mocs. Nous regrettons donc que rien n'apparaisse dans le texte sur le volet prévention, sur l'urgence d'en faire une grande cause nationale, à l'attention des consommateurs d'une part, mais aussi d'autre part des personnes en grande précarité, qui sont la cible privilégiée des trafiquants pour devenir les petites maies de ces réseaux, le lumpet prolétariat de cette industrie. Rien sur les mesures d'information pour éviter l'entrée dans la consommation, rien sur le parcours de soins, sur la prise en charge des addictions, sur l'intérêt de légaliser ou de dépénaliser certains usages. Aucune mesure donc de politique de santé publique. Rien non plus sur le volet économique et social pourtant discuté dans la commission d'enquête, levier majeur de la lutte contre le narcotrafique dont a très bien parlé Jérémie Bakki. Rien sur la politique de la ville, rien sur la lutte contre les précarités, sur l'insertion par l'école et le travail. Enfin, rien sur l'accompagnement et le traitement social des victimes du darko trafic et de leurs familles. L'autre volet important est l'introduction de dispositions qui nous paraissent bien trop gênantes. Si nous accueillons favorablement la suppression d'accès aux messageries cryptées, certaines mesures nous apparaissent bien trop attentatoires aux libertés. C'est donc avec déception que notre groupe constate une sorte de phagocytage de la loi par les deux ministres d'État, M. Retailleau et Darmanin. La porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, déclare en conférence de presse post-conseil des ministres au sujet des attaques inacceptables contre les lieux de détention, je cite une réaction du milieu sur les décisions courageuses de M. Retailleau et Darmanin prises sur le narcotrafique et explique qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des ordres dispositions et dispositifs mis en place par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, proposés par une PPL du Sénat, ont été votés. Pas plus tard que jeudi dernier, Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, se félicite aussi que cette loi, issue de sa commission d'enquête sur l'ordre agrographique, n'ait de sans-droit de tirage et du vote définitif à venir. Je rappellerai juste que la création de cette commission a été demandée en premier lieu par trois sénateurs qui sont écologistes et de gauche et issus des Bouches-du-Rhône, Marie-Arlette Carlotti, Jérémy Boiky et moi-même. Dans la même conférence de presse, il se félicitait que la loi augmente les pouvoirs du préfet pour l'interdiction de paretes, pour la fermeture des blanchisseuses et en se substituant aux bailleurs pour expulser des logements sociaux et les trafiquants. Notre groupe voit en cela aussi le détournement politique regrettable de l'objectif de la loi, puisque rien dans ces mesures, contestables constitutionnellement, ne s'attaque au haut du spectre. Et en plus, je dirais que ces mesures ne figurent pas dans les travaux de la Commission d'enquête sénatoriale. Le consensus du Sénat sur celui de la Commission d'enquête n'est plus là, alors que ce texte aurait pu rester transpartisan grâce à sa volonté aux réelles mesures qu'il porte pour s'attaquer vraiment aux organisations du narcotrafique et à leurs dirigeants. Tout comme pour la loi immigration, nous ne pouvons voter une loi qui manifestement comprend des mesures non-constitutionnelles. Nous répétons le danger que représente cette méthode qui cherche à écrire des mesures d'affichage pour rejeter la responsabilité vers le Conseil constitutionnel de censurer des mesures présentées à tort comme des outils naturels. Pour toutes ces raisons, notre groupe geste s'abstiendra. Merci. La parole est à monsieur Jérôme Durand pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Nous sommes aujourd'hui réunis pour la lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire qui a permis à l'Assemblée nationale et au Sénat de se mettre d'accord sur une version consensuelle de la proposition visant à sortir la France du piège du narcotrafique. Ce texte, finalement, c'est peut-être en léger décalage avec ce que vient de dire mon collègue Guy Benaroche, essentiellement le texte du Sénat, moins l'injonction pour richesse inexpliquée, plus les amendements voulus par le gouvernement dans une configuration assez originale, ça a été dit par le ministre Retailleau, et qui est plutôt à l'honneur de nos institutions, de notre Parlement et de cette Chambre ou de quel Sénat. Permettez-moi d'exprimer d'abord la position du Coupe socialiste écologiste et républicain sur le texte qui nous est proposé. Par rapport au texte que nous avons voté à l'unanimité le 4 février dernier, je note plusieurs motifs de satisfaction. D'abord, la suppression de l'article 8R qui avait été introduit contre l'avis des rapporteurs de cette Chambre et notamment par la présidente Giordano Giordano Giordano Giordano. Il nous semble que c'est une suppression qui est bienvenue. Cet article inquiétait en effet bon nombre d'observateurs et défenseurs des libertés publiques. Il nous semblait qu'il n'était pas de bonne méthode d'introduire dans un texte par la voix d'un amendement issu de l'hémicycle une mesure aussi lourde. Et d'ailleurs je constate que toujours dans la sphère du renseignement, la limitation de l'extension du renseignement algorithmique au seul haut du spectre répond aux interrogations qui ont pu émerger. L'article relatif au procès verbal distinct. constitue à n'en pas douter un des sujets qui a été les plus sensibles dans ce texte. Les réécritures successives de ce dispositif ont été éclairées par l'avis du Conseil d'État. Elle me semble avoir permis de trouver un juste équilibre entre les droits de la défense, nous y avons beaucoup travaillé ici à la Commission des lois, et le besoin de protéger l'efficacité des techniques spéciales d'enquête pour lutter contre la criminalité organisée. À qui majeure du texte, la création du Parquet National Anticriminalite Organisée, entérinée pour début 2026, le 4 ou le 5 janvier, je ne me souviens plus, permet la création d'un chef d'orchestre qui correspond au vœu de la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider. Le PNACO sera systématiquement informé des dossiers pris en charge par les GIRS, ce qui lui permettra de faire jouer son pouvoir d'évocation pour le haut du spectre et disposera d'un lien privilégié avec les services de renseignement du 1er siècle. J'en viens maintenant à l'enjeu sensible des prisons. Les propositions du garde des Sceaux ont interrogé à gauche. Je dois rappeler qu'elles n'avaient pas été proposées à la sénat en première lecture. C'est un peu l'organisation de notre travail, cette démarche complément d'apport qui nous a conduits à ce texte final. Au groupe socialiste, écologiste et républicain, nous sommes la gauche fière de défendre l'héritage de Robert Badinter qui, vous vous en souvenez, avait contribué à la fin des quartiers de haute sécurité. nous revendiquons également le fait d'incarner une gauche responsable pleinement consciente des nouveaux enjeux propres à l'adaptation de la criminalité organisée au milieu carcéral. La commission d'enquête avait elle-même mis le doigt sur le danger qui pèse sur les prisons et sur les membres d'administration pénitentiaire que nous voulons assurer de notre plein soutien. La Commission mystoparitaire a décidé de réduire à 12 mois la durée de la décision d'affectation dans ses quartiers de lutte contre la contre la criminalité organisée, telle qu'elle avait été proposée initialement par le garde des Sceaux, et en accord d'ailleurs dans le cadre d'un travail avec le ministre. Cette évolution est très chère aux parlementaires socialistes et elle va, selon moi, lever un certain nombre d'inquiétudes et de craintes qui ont été exposées par les opposants à cette mesure. Sur les prisons, je veux revenir sur la terrible actualité que connaît notre pays. Tout au long de la commission d'enquête, nous nous sommes interrogés. Exagérons-nous la menace ? Est-ce que finalement ce qu'on nous dit est vraiment conforme à la réalité ? Est-ce que nos interlocuteurs n'en font pas un peu trop ? D'ailleurs, quand on a rendu nos conclusions, il y avait quelques sarcasmes, des doutes. Aujourd'hui, je crois que plus personne dans ce dans ce pays ne doute de la gravité, de la réalité, de la menace qui pèse sur le pays en raison du narcotrafique. Cette loi que nous allons voter permettra de réduire le déséquilibre des moyens que nous constatons souvent dans la lutte contre la criminalité organisée qu'il s'agisse des policiers, des douaniers, des gendarmes, des magistrats et parfois des élus locaux aussi. Elle permettra beaucoup cette loi, elle ne permettra pas tout. Il appartient à notre société de s'interroger sur son rapport à la drogue. Est-ce qu'on en fait assez sur la prévention ? Ça a été dit par d'autres orateurs. Est-ce que la répression de la consommation est une solution indépassable en ce qui concerne certaines substances ? Les consommateurs malades sont-ils suffisamment accompagnés ? Ce sont des questions qui méritent d'être abordées dans la sérénité et loin du combat partisan. J'espère que notre Chambre pourra y contribuer avec le même regard constructif qu'elle a porté sur les aspects répressifs présents dans ce texte. Un texte que les sénateurs socialistes voteront, vous l'aurez compris, en pleine responsabilité. Merci, chers collègues. Conformement à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre en voie l'ensemble de la proposition de loi ordinaire visant à sortir la France du piège du narcotrafique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission expéritaire, modifié par les amendements du gouvernement et de la commission. Je suis saisi d'une demande de scrutin public sur ce texte par le groupe Les Républicains. Le scrutin est ouvert.

demande à voter. Le scrutin est clos. 341 votants, 325 exprimés pour 325. La proposition de loi est adoptée. Conformément Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi organique, fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisé dans la rédaction résultante du texte élaboré par la Commission mixte paritaire. Je rappelle qu'en application de cet article, le Sénat statue par un seul vote sur l'ensemble du texte. Au terme de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. 341 votants, 341 exprimés. Pour 341, la proposition de loi organique est adoptée. Je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour CG au sein de la Commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition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 L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire. Une demande de la Commission de la Culture, d'Education, de la Communication et du Sport. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Ce texte est examiné sur la procédure de législation et de commission prévue au chapitre 14 bis du règlement du Sénat. La parole est à monsieur Max Brisson, rapporteur de la Commission de la Culture, de l'Education, de la Communication et du Sport. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, le moins que l'on puisse se dire est que la propulsion de loi de Laurent Laffont que nous allons voter cet après-midi est à plusieurs égards dérogatoire à la doctrine que nous sommes fixées sur les restitutions d'œuvres d'art dans le cadre de l'engagement de longue date sur le sujet de la Haute-Assemblée. Quand nous avons en effet, avec mes collègues Catherine Morin de Sailly et Pierre Ousoulias, recommandé dès 2020 que les engagements politiques et diplomatiques à la restitution de telles ou telles oeuvres ne précèdent pas la consultation du Parlement. Nous avons également préconisé l'intervention systématique d'un conseil national chargé d'une expertise scientifique préalable aux temps politiques. Une forme de consensus s'était même nouée un temps sur la mise en pause des lois d'espèces qui pouvaient nourrir le sentiment d'une forme de fée du prince pour privilégier la construction d'un cadre législatif général. Sur la restitution du tambour parleur Didier Ayokoué, demandé par la Côte d'Ivoire il y a six ans, rien n'a été fait pour que cette méthode soit respectée. Pas d'expertise préalable de conseils scientifiques, pas de loi cadre et pourtant, la France est engagée par la foi de son président de la République à satisfaire à cette demande dès 2021. Or, depuis cette date, aucune portée juridique concrète n'a été donnée à l'engagement que notre centre des responsabilités nous impose pourtant aujourd'hui de tenir. Et c'est bien parce que la Commission de la culture du Sénat depuis des années travaillé la question des restitutions d'une initiative transpartisane portée par Laurent Laffont, son président, a pu intervenir pour pallier cette carence. Alors pourquoi, mes chers collègues, accepter de déroger à nos principes ? Parce que nous pouvons parfaitement appréhender l'origine de l'œuvre, son histoire, son entrée dans les collections publiques françaises, son parcours. Didier Ayokoué est un tambour à fente de l'ethnie hachante, arraché à sa communauté d'origine par l'administration coloniale il y a plus d'un siècle. Cet instrument aujourd'hui exposé au musée du quai Branly Jacques Chirac n'est pas un tambour ordinaire. Par ses dimensions, puisqu'il mesure plus de 3 mètres 50, par ses qualités esthétiques qui ont conduit à ce que sa présence au palais du gouverneur de Bergerville soit signalée au Musée de l'Homme par l'écrivain Paul Morand en 1929, par sa fonction au sein de l'ethnie hachane qu'il utilisait comme instrument de communication servant à annoncer des événements et à transmettre des messages, notamment sur la progression de l'armée coloniale française. Sa place dans la communauté à Tchad était centrale, au point qu'il était considéré comme une entité spirituelle partie intégrante de ce peuple. Nous vous invitons également, mes chers collègues, à déranger parce que son absence au plongée aurait pu créer des difficultés entre notre pays et la République de Côte d'Ivoire. Il eût été tout à fait regrettable que les excellentes relations que la France entretient avec la Côte d'Ivoire se trouvaient altérées par l'absence de traduction concrète des engagements pris par le chef de l'État en 2021. Cela ne sera pas, heureusement, le cas. Et permettez-moi de saluer en tribune son Excellence M. Maurice Bordaman, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France et ancien ministre de la Culture. M. Mamadou Touré, ministre la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service édique. Et M. Ibrahima Diabete, président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. L'inertie que nous avons connue ces dernières années était d'autant plus étonnante que la demande ivoirienne était parfaitement légitime compte tenu des conditions dans lesquelles le tambour a été intégré aux collections françaises, également tout à fait exemplaire au regard des préconisations de notre Commission sur la méthode des restitutions. Car ce que nous n'avons pas encore intégré dans notre droit a été fait de manière spontanée par les acteurs de terrain ivoiriens et français dans le cadre d'un projet muséal à la forte dimension scientifique et partenariale auquel la France apporte un appui opérationnel et financier. Ce projet vise en effet à adapter le Musée des civilisations de la Côte d'Ivoire à la conservation. et à l'exposition du tambour. Il tente également à la construction d'une histoire du tambour incontestable d'un point de vue historique et partagé entre nos deux pays. Son achèvement, prévu pour le mois de juillet, permettra une réappropriation de son patrimoine par la Côte d'Ivoire en même temps qu'une analyse de son passé colonial par la France. L'exemplarité de cette démarche, conjuguée à l'importance des investissements consentis par notre pays, doit donc nous conduire à répondre dans les plus brefs délais à la demande de restitution de la Côte d'Ivoire. Grâce à vous Madame la Ministre, la conclusion d'une convention de dépôt en novembre dernier a constitué un signal positif. Il est cependant impératif d'aller plus loin et de rendre à la Côte d'Ivoire la pleine et définitive propriété du tambour, parce qu'elle suppose de déroger, au principe d'inaliénabilité des collections publiques, cette opération nécessite l'intervention du gélateur télé, l'objet de l'article unique de cette proposition de loi. Pour la suite, car il est certain désormais que le mouvement de restitution ira à son profondissant. Les réserves du Sénat sur la méthode aujourd'hui suivie pour restituer des oeuvres d'art restent entières, comme nous l'avons fait lors de notre réunion du 9 avril. J'exorde le gouvernement à travailler en lien avec notre Commission pour définir de manière concertée les principaux éléments d'une éventuelle loi cadre. Dans cette attente, je vous invite, mes chers collègues, à suivre la position unanime de la Commission en vous prononçant pour le retour du tambour-parleur Gigi Ayokoué sur son sol d'origine. Ce faisant, nous répondrons à l'attente légitime de la communauté hachiane et au-delà de toute la nation ivoirienne. Nous veillerons également en responsabilité à ce que la parole donnée par la France se traduise en hâte. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, cher Laurent Lafont, Monsieur le Rapporteur, cher Max Brisson, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Nous nous réunissons cet après-midi autour d'un texte important dans la continuité d'un travail entamé depuis plusieurs années déjà. Je voudrais à nouveau saluer l'engagement de la Commission des affaires culturelles du Sénat et de son président Laurent Lafont, qui en matière de restitution ont joué un rôle déterminant, ainsi que son rapporteur cher Marcus Brisson, puisque nous souhaitons même aller plus loin désormais. Le Sénat, de manière transpartisane, s'est emparé de ce sujet essentiel à l'apaisement des mémoires et contribue à une véritable prise de conscience collective. Je souhaite également saluer la présence de M. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Maurice Mandaman, et le ministre Mamadou Touré, présent ici dans les tribunes. Dans ce travail, le ministère de la Culture a également su prendre ses responsabilités, d'abord avec la loi cadre que vous avez rappelé du 22 juillet 2023, sur les biens spoliés du fait des persécutions antisémites survenues entre 1933 et 1945, ensuite avec les travaux en cours déjà menés ou déjà menés sur les restes humains. À ce titre, la loi du 26 décembre 2023, portée par la sénatrice Morin d'Esailly, a permis la publication d'un décret le 2 avril dernier autorisant le transfert de trois crânes sac à lave des collections françaises à la République de Madagascar et je peux vous dire qu'ils en étaient très heureux lors de notre dernier déplacement avec le président de la République. Je souhaite saluer son travail de très longue date sur ce sujet. Je pense également au rapport et à la proposition de loi du député Marion sur la restitution des restes humains ultramarins. Alors aujourd'hui, nous examinons un texte portant sur la restitution du tambour parleur à Chan à la République de Côte d'Ivoire. Cette proposition de loi s'inscrit plus globalement dans une démarche très chère au Président de la République, telle qu'il l'a définie dans son discours de Ouagadougou en 2017. Cette démarche est celle qui vise à renouveler, à renforcer nos relations avec le continent africain, que ce soit par la restitution de biens culturels ou plus largement par la circulation des oeuvres entre la France et ses partenaires africains. Cet engagement s'est d'ailleurs déjà illustré à travers la loi du 24 décembre 2020, relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Cette politique de restitution répond à des enjeux de politique étrangère et est d'ailleurs de plus en plus prise en compte dans les enceintes diplomatiques à l'Union africaine, au G20 ou encore à l'UNESCO. Elle répond également à un enjeu de réparation qu'il faut mentionner comme tel. Réparation s'agissant de peuples qui ont pu être privés de l'accès à leur patrimoine et à ce qui fait partie intégrante de leur mémoire. Nous poursuivons donc aujourd'hui ce cheminement avec la proposition de loi qui nous occupe concernant la restitution du tambour parleur à la République de Côte d'Ivoire. Ce texte est le résultat d'un travail commun. La restitution avait été actée en 2021 par le président de la République et son nomologue, le président Alassane Ouattara. Depuis, un travail a été mené conjointement afin que ce tambour puisse retrouver son pays d'origine et, à nouveau, le ministère de la Culture s'y est pleinement engagé. Je veux saluer aussi les travails des équipes du musée du quai Branly Jacques Chirac et du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. N'oublions pas que le dialogue scientifique est constitutif du processus de restitution de biens culturels tels que nous le concevons avec nos partenaires africains et bien au-delà. Leur engagement a permis d'aboutir de façons pragmatiques à une double solution, le dépôt et la restitution. Le 18 novembre dernier, j'ai donc signé avec mon homologue ivoirienne la ministre Françoise Remarque une convention de dépôt. C'était une première étape pour garantir dès que possible le retour du tambour à Abidjan selon le calendrier de fin des travaux et de réouverture du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Il s'agissait aussi d'envoyer un signal clair, volontariste, à nos partenaires ivoiriens et non de contourner le circuit législatif. Parallèlement, votre engagement sur ce sujet a abouti au dépôt d'une proposition de loi au Sénat, un texte qui nous permet désormais d'avancer sur le chemin de la restitution L'article unique de cette proposition de loi a donc dérogé, au principe, je vais me lancer cher Max Brisson, inaliénabilité, des collections nationales prévues par le Code du patrimoine. Cette proposition de loi, qui est une proposition de loi d'espèce, marque une avancée importante. Nous devrons à l'avenir poursuivre notre dialogue concernant l'élaboration d'une loi cadre relative aux restitutions. C'est un chantier dont nous devons nous saisir ensemble. Je l'ai dit en commission il y a quinze jours, j'y suis pleinement favorable. Et les échanges que j'ai eus encore à Madagascar aux côtés du Président de la République nous renforcent dans cette conviction. je sais que c'est un texte très attendu par la Chambre haute et moi je peux vous dire que nous sommes prêts. Cependant, au vu des enjeux qui entourent ce texte, ce débat ne pourra se faire que dans un cadre apaisé, vertueux et qui exprimera la volonté de la représentation nationale de faire droit aux demandes de restitution de ses partenaires étrangers. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ouvrir la porte à une instrumentalisation des débats. J'attends la confirmation. J'y veillerai à travers la consultation des groupes représentés au Parlement et que je souhaite engager dès à présent sur ce dossier. Enfin, cette proposition de loi et la restitution du tambour parleur s'inscrivent dans la perspective de la réouverture du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire qui devrait avoir lieu d'ici la fin 2025. A travers l'appui que la France apporte à sa rénovation et aussi à sa modernisation, ce musée incarne notre ambition en matière de politique de restitution. Elle s'accompagne d'un dialogue scientifique, comme je l'ai évoqué. Elle s'accompagne également d'une démarche de coopération muséale et patrimoniale. Le partenariat avec la Côte d'Ivoire illustre parfaitement les différentes dimensions de notre approche. Alors, mesdames et messieurs, cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui témoigne de la volonté de la France d'écrire une nouvelle page de notre histoire partagée avec l'Afrique. Cette page, nous l'écrivons conjointement avec le Sénat, sa commission des affaires culturelles et le travail approfondi que vous avez mené nous permet désormais de franchir cette nouvelle étape qui est une étape importante, essentielle et qui, j'en suis sûre, continuera aboutira évidemment à l'adoption du texte de cette loi cadre que nous attendons tous. C'est pour l'ensemble de ces raisons que vous pouvez compter sur mon soutien plein et entier sur ce texte. Je vous remercie. Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Ruel pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues et vous, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et Monsieur Mamadou Touré, Ministre de Côte d'Ivoire, en tribune. Saviez-vous qu'au XXe siècle, le peuple ébrier Hatchan se servit du tambour-parleur Jiji à Yokuei pour avertir grâce à un langage tambouriné de dangers dont celui de l'arrivée de l'administration coloniale venue réquisitionner les membres de la communauté pour le travail forcé ? Le retour prochain sur ces terres d'origine de ce tambour sacré, datant de la fin du XVIIIe et confisqué en 1916, est donc hautement symbolique, mais pas que. Revenons un peu en arrière sur cette humultueuse histoire. Réclamé en 2019 par le président Ouattara, le président de la République française annonce sa restitution lors du sommet France-Afrique du 8 octobre 2021. Puis pendant trois ans, rien ne se passe, rien. Jusqu'à faire désespérer les autorités ivoiriennes de revoir un jour le précieux instrument. Et ce, faute au report successif du vote d'une loi cadre sur la restitution de biens culturels, j'y reviendrai. C'est donc à la faveur d'une loi d'exception que nous sommes réunis aujourd'hui pour autoriser la restitution tant attendue du Didi à Yokuei. Loi d'exception par sa forme, mais aussi exceptionnelle par les effets qu'elle emporte. La restitution du Didi à Yokuei à la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique. de réappropriation du patrimoine, de sauvegarde des mémoires, de découverte pour les jeunes générations de leur histoire, de leur culture, de consolidation d'une identité culturelle. L'intégration espérée du Didier Ayokoué aux collections ivoiriennes s'est accompagnée d'une formidable revitalisation du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, dit MCCI. avec la réhabilitation du bâtiment principal, le réaménagement des espaces qui accueillent plus de 15 000 oeuvres, la formation des équipes, le développement d'une stratégie de médiation culturelle. Actions qui ont été soutenues notamment par l'AFD et Expertise France. Aucun doute à avoir sur les conditions d'accueil de qualité qui sera réservé au Tambour sur ces terres ancestrales. Ce retour et les aménagements du MCCI ouvrent aussi la voie pour les 148 objets du patrimoine réclamés encore par la Côte d'Ivoire. Leur institution symboliserait une étape clé dans le renforcement du partenariat culturel et patrimonial entre nos deux pays. Pour ces raisons, Je me prononcerai bien évidemment en faveur de cette proposition de loi. Cela étant dit, je souhaiterais vous livrer, chers collègues, quelques-unes de mes réflexions mûries, entre autres par mon expérience ivoirienne et plus largement africaine. La première. Le caractère arbitraire et aléatoire de ces restitutions est la proportion infime des objets rendus, moins d'une trentaine sur les 150 000 biens africains que conservent les 230 musées français. A cet égard, je crois que la France gagnerait à s'inspirer de ses voisins européens dont la politique en matière de restitution a gagné en souplesse au cours de ces cinq dernières années. ni de rendre distinctement ni au gré de nécessité diplomatique. Il faut bien évidemment organiser scientifiquement les travaux d'examen de restitution et établir une méthodologie permettant de déterminer la provenance, la circonstance de la première acquisition, etc. et de s'assurer des conditions d'exposition, de mise en valeur, de conservation de conservation de l'œuvre transférée. Ma seconde réflexion concerne bien sûr Madame la Ministre, l'absence de loi cadre. Madame la Ministre, un projet de loi cadre avait été rédigé en 2023 par votre prédécesseur, Madame Abdoul Malak, mais n'avait pas survécu aux critiques légitimes du Conseil d'État. Aux yeux des juges, les motifs de restitution évoqués dans le texte, à savoir la conduite des relations internationales et à coopération culturelle, ne justifiaient pas une dérogation au principe d'inaliabilité des collections publiques. La sortie de la dominalité publique doit en effet être impérativement motivée par un intérêt public supérieur ou par un motif impérieux. Ces motivations auraient pu simplement être ajoutées au texte, reproposé par la suite pour validation au Conseil d'État. Vous n'en avez pas fait une priorité, nous imposant donc de légiférer à postériorité à posteriori, d'annonces de restitution déjà actées. Ces solutions de fortune ne sauraient constituer une poétique cohérente culturelle, garante de l'intégrité de nos collections publiques et respectueuse pour nos partenaires africains. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des travaux engagés par la Commission de la Culture du Sénat sur le sujet des restitutions d'œuvres d'art. Nous pouvons nous féliciter de cette expertise et de ce travail transpartisan permettant de faire émerger cette question de manière sereine au vu des enjeux qu'elle contient. Cette PPL vise à répondre à la demande de restitution du tambour Gigi Ayokwe par les autorités ivoiriennes en 2019. En 2021, le président de la République s'est engagé à satisfaire cette demande, mais le processus juridique de sortie du tambour des collections publiques n'a pas été enclenché depuis. considérée comme une entité spirituelle par les communautés hachans à qui il appartenait, ce tambour parleur confisqué en 1916 était un outil de communication servant à prévenir des dangers, à mobiliser pour la guerre et pour la guerre et a été un outil de communication très utile, notamment lors de la conquête coloniale. Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'une coopération muséale et diplomatique étroite entre la France et la Côte d'Ivoire. Il est donc nécessaire de satisfaire cette demande de restitution afin de préserver la forte relation bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. que j'ai pu d'ailleurs constater directement lors de mes déplacements et que je salue, ainsi que M. l'ambassadeur, sur le plan culturel, diplomatique, de l'enseignement ou du développement. J'en profite pour saluer également le travail de coopération muséale engagé entre la France et la Côte d'Ivoire afin d'adapter les infrastructures du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire à la conservation, à l'exposition du tambour. Ce projet a pu se réaliser grâce à l'appui sous la houlette du MCCI de nos agences comme l'AFD Expertise France ou encore des entreprises françaises d'ingénierie culturelle. Permettez-moi de souligner le rôle essentiel de ces agences dans notre politique de coopération internationale et d'aide au développement, ici dans une optique de développement de politiques culturelles durables. Cette approche partenariale fondée sur sur l'échange de savoir-faire et de respect des identités permet de renforcer le lien entre patrimoine et développement. Ainsi, le lancement du processus de restitution a débuté le 18 novembre 2024 par la signature par les ministres de la Culture des deux pays d'une convention de dépôt, c'est-à-dire un prêt de longue durée renouvelable, permettant de préparer le transfert du tambour dans les prochains mois. Notre Commission a jugé que cette solution provisoire n'était pas adéquate compte tenu d'une part des engagements pris par la France et d'autre part des investissements fournis dans le cadre de la coopération muséale mise en oeuvre. une intervention législative était nécessaire. Et je salue ce texte. Pour conclure, je rejoins les conclusions de la Commission sur la nécessité absolue de travailler à une loi cadre sur les restitutions. Nous ne pourrons pas continuer à légiférer au cas par cas. Nous avons besoin d'un cadre juridique permettant de respecter le principe d'inaliabilité des collections publiques tout en s'adaptant aux enjeux de notre temps. Le groupe RDPI votera donc évidemment en faveur de cette proposition de loi et pour finir je tenais à saluer l'engagement du gouvernement qui poursuit ici la dynamique initiée par le discours du président de la République à Ouagadougou en 2017 et confirmé par les récentes restitutions à la République du Bénin et au Sénégal. Merci. Merci. La parole est à monsieur Bernard Fialer pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues, Le groupe RDSE votera ce texte de restitution d'un bien culturel à la Côte d'Ivoire, comme nous en avons débattu en commission. Je partage entièrement les propos du rapporteur Macron aussi, je n'y reviendrai pas, et permettez-moi de profiter de l'occasion qui nous est donnée pour revenir sur une réflexion que nous pouvons mener sur le statut et la patrimonialité des biens culturels. L'inaliénabilité des biens culturels est issue de la Révolution française qui voulait sauvegarder dans le patrimoine national des biens dont la royauté pouvait jouer à son gré. Aujourd'hui, reconnaissons que c'est l'inaliénabilité de la dimension culturelle des biens que nous voulons garantir. On atteste d'ailleurs les différentes restitutions et les conditions que nous exigeons de ces transferts de propriété. Nous pourrions envisager l'attribution de ces biens culturels à un patrimoine mondial de l'humanité. Ces biens culturels sont inestimables et ne peuvent être négociés. Leur provenance peut prêter à discussion et soulève parfois des disputes historiques sur les us et coutumes en vigueur à l'époque de leur acquisition. Le débat que nous avons eu sur le terme de restitution avec sa connotation culpabilisante ou de retour avec une appréciation purement géographique n'intègre pas l'apport culturel de l'acquereur qui a parfois sauvé de l'oubli, de la négligence ou même de la destruction de ses biens culturels. Ils deviennent un bien culturel par le regard porté par leur acquisition. un bien devenu culturel relève du patrimoine mondial de l'humanité. Les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres. La Convention de 1972 n'intègre pas les biens culturels matériels. Elle concerne les lieux patrimoniaux et, depuis 2003, le patrimoine immatériel de l'humanité. Ne conviendrait-il pas de faire évoluer cette Convention pour l'élargir aux biens culturels matériels ? Ce patrimoine mondial de l'humanité pourra alors se répartir entre les lieux d'origine de certains biens culturels qui revêtent une dimension essentielle à l'identité d'un peuple ou d'un territoire, et c'est le cas du tambour Jiji Aoké, dont nous parlons aujourd'hui, ou alors il peut séjourner dans des musées pour alimenter un dialogue interculturel. Consacrer l'inaliénabilité culturelle d'un bien plutôt que sa propriété ne serait-il pas un progrès pour l'humanité que nous sommes en droit d'attendre la contribution de la culture ? Ce progrès dans le domaine culturel pourrait même éclairer une réflexion à mener sur la propriété d'autres biens. réflexion qui serait bien utile dans une période d'agression territoriale et prédation de richesses naturelles. C'est le rôle de la culture d'ouvrir les esprits et de stimuler l'émergence de concepts qui pourraient rendre notre monde plus beau et plus fraternel. C'est l'honneur de notre culture nationale d'initier cet avancé vers un patrimoine mondial qui intégrerait les biens culturels avec les sites et lieux patrimoniaux et le patrimoine immatériel de l'humanité. bien. La parole est à madame Catherine Morin de Saillie pour le groupe Union Centriste. Monsieur le Président, Madame les Ministres, mes chers collègues, le présent texte visant à restituer le tambour par l'heure d'Yidi Ayokoué à la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la lignée de plusieurs textes, autres textes d'initiative sénatoriale et d'un travail de fond réalisé par notre commission de la culture. M'exprimant pour le compte de notre groupe union-centrise, je tiens à rappeler à quel point celui-ci a été de longue date, moteur d'une réflexion devenue nécessaire alors que ces 20 dernières années les demandes se sont faites de plus en plus pressantes. Les pays anciennement colonisés, retrouvant le chemin de leur histoire et le besoin de renouer avec leur passé, de valoriser leur culture et leur identité et aussi en faire un atout de développement. La mondialisation et le travail d'institutions internationales comme l'UNESCO ou l'ECOMOS ont contribué, elles aussi, à une meilleure connaissance et reconnaissance des cultures de tout à chacun et ont relayé ces besoins. Madame la Ministre, nous saluons l'engagement de votre Prédécesseur, Imad Abdulmalak, qui reconnaissait le travail pionnier du Sénat et proposait en 2022 de mettre en œuvre un triptyque législatif, un premier texte pour la restitution des biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites, un deuxième déjà engagé en réalité par le Sénat pour la restitution des restes humains et enfin un troisième pour les biens culturels. Après l'adoption de lois d'espèces, celles sur le retour de la Vénus autentote à l'Afrique du Sud et des têtes mauries à la Nouvelle-Zélande, puis la loi de restitution des 26 oeuvres à la République du Bénin et le sabre d'El Hajj Omar Tal au Sénégal dont j'étais rapporteur, nous avions insisté, tout banc confondu, sur la nécessité de disposer d'un cadre général et d'une méthode garantissant pour les parties prenantes l'authenticité et la rigueur de la démarche. que nous avions moyennement apprécié que le Parlement, garant des collections nationales, seule habilité à permettre une dérogation au principe de leur inalinabilité, ait été mis plusieurs fois devant le fait accompli d'annonces de restitution avant même d'avoir pu mesurer leurs biens fondés. Un contournement des procédures par ailleurs contre-productifs, y compris pour les pays demandeurs. Depuis 2022, Les deux premières lois CAD se sont concrétisées. La loi du 23 juillet 2023, relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, rapportée par notre collègue Béatrice Gosselin. Puis la loi du 27 décembre 2023 que j'ai portée comme vous le savez avec mes deux collègues. Elle permet désormais la restitution de restes humains réclamés par des états étrangers appartenant aux collections publiques. Je me réjouis qu'elle ait trouvé sa première application concrète, Madame la Ministre, avec la restitution des crânes Sakalava à Madagascar. J'espère maintenant l'aboutissement rapide du dossier australien. Cela fait plus de dix ans que l'ambassadeur d'Australie était venu me trouver. Reste également aujourd'hui établir une liste claire des restes humains restituables présents dans nos collections publiques. Nous mesurons l'ampleur de la tâche, bien sûr, et l'importance des moyens humains et financiers nécessaires. Maintenant, l'article 2 de la loi doit enfin s'appliquer concrètement. Une réponse rapide doit être apportée à la Guyane et à l'association Modico pour le retour des restes humains Calinas. Aussi, sans plus attendre, nous avons déposé avec Pierre Ousoulia et Max Brisson un texte très simple qui permettrait non pas de traiter toute la question ultramarine au demeurant nécessaire, mais au moins déjà cette légitime demande, nous aurions occasion d'en reparler. Le troisième texte de loi se fait lui aussi attendre, d'où la proposition de notre président Laurent Lafont que nous allons voter aujourd'hui et qui permet d'honorer l'engagement pris par le président de la République en 2021. Notre rapporteur Max Brisson a très bien exprimé le bien fondé de la restitution de cet objet qui revêt une grande importance culturelle et spirituelle pour la communauté ivoirienne à Tchènes dont je salue chaleureusement les représentants ce jour parmi nous. Madame la Ministre, nous espérons donc que l'adoption du présent texte soit l'occasion de relancer et d'achever un processus législatif dont l'aboutissement représenterait un véritable progrès sur un sujet hautement sensible au carrefour de la culture et de la diplomatie. Nous sommes prêts ici au Sénat pour ce dernier texte, au contenu duquel nous avons déjà travaillé et surtout été atroitement associés avec mes collègues. Vous comprendrez donc notre impatience. En conclusion, j'insisterai sur le fait que si la restitution des biens culturels et des restes humains participe au renouvellement des liens de la France avec certains Etats étrangers par le dialogue des cultures, elle n'épuise pas le champ des coopérations nécessaires et fructueuses, telles étaient les préconisations de notre mission d'information avec Pierre Ouzoulia et Max Brisson qui souhaitaient que nous vélions à la circulation des œuvres, aux résidences croisées, aux expositions communes. Fort de mon expérience, je peux vous dire que la restitution des têtes mauries à la Nouvelle-Zélande a davantage été le début d'une nouvelle aventure, qu'interdit certes à une histoire abominable, mais aujourd'hui expliquée, racontée, mais en même temps a permis l'émergence de nouveaux projets scientifiques et culturels à rapprocher nos peuples, nos cœurs et nos cultures. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Président Pierre Ouslian pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur l'ambassadeur, D'où viens-tu, quitte à créer ? Le tambour est matière pour les artistes qui le sculptent, son pour les physiciens, divin pour les croyants. Pour ces derniers, au cancement, est-il tambour ? Le tambour est énergie, puis vibration, laquelle devient son émot, et finalement, phrase venue de Dieu, il explique comment le Verbe est né. Ainsi s'exprimait Georges Niangoramboua, ethnologue ivoirien, spécialiste des instruments de musique traditionnels d'Afrique de l'Ouest et de la mémoire sonore africaine qui posa les bases de la drumologie, la science du langage tambouriné. En 1958, le Musée de l'Homme lui confia une mission ethnographique en Côte d'Ivoire pour tenter de déterminer l'origine l'usage phonique et la fonction religieuse du tambour rafante appelé Jiji Ayokwe, le tambour panthère. L'enquête qu'il mena auprès de la communauté des Tchamans des Bijans raviva le douloureux souvenir de la perte de ces objets et provoqua des cris d'effroi et de colère de ceux pour qui il conservait un prestige symbolique et une fonction initiatique dont ils avaient été privés. Le calme revenu, la communauté décida d'adresser une supplique au président ivoirien Félix Oufuette-Boigny pour qu'il demande à son homologue français, le président Charles de Gaulle, la restitution du pression-tambour. Ce fut sans doute l'une des toutes premières demandes de restitution. Symbolique ce tambour, l'est à plus d'un titre. C'est une oeuvre d'art d'une grande force, réalisée par le sculpteur Bien Gui. C'est aussi un instrument de communication dont les messages pouvaient être entendus à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est enfin un objet rituel qui est indispensable aux cérémonies de l'organisation politique traditionnelle des Tchamans, fondée sur le système des classes d'âge dit APAZA. Comme de nombreux biens culturels africains, ces multiples fonctions échappent aux catégories trop étroites de l'art occidental. Cette pluralité de sens a été détruite par l'appropriation coloniale et le transfert dans un musée. Sa restitution ne permettra pas de les restaurer. Il demeurera le témoin d'une tradition perdue. Comme le dit Guy Diagois, le chef bidjan d'Atécoubet, je le cite, « Tous ceux qui avaient le savoir-faire, qui sculptaient le tambour de génération en génération, sont partis avec leur connaissance. La langue tambourinée, elle-même, n'est plus comprise. Aokwe a lancé son dernier message en 1916 pour prévenir de l'arrivée de la troupe qui s'est emparée de lui. Ce tambour est également représentatif de la violence physique et symbolique exercée sur les populations ainsi que des difficultés à en déterminer aujourd'hui les circonstances exactes Sa saisie par l'administration coloniale en 1916 est avérée, mais les raisons de ce vol demeurent incertaines. Georges Niagora-Boura en cite deux versions divergentes. Il fut probablement déposé à Bains-Gerville, chef-lieu de la colonie, avant d'être convoyé à Paris et conservé définitivement par l'Humaisée d'ethnographie de Paris le 1er mars 1930. En 1958, la mission ethnographique suscita une première demande de restitution que l'on pourrait considérer, avec un brin de malice, comme réitéré par le gouvernement ivoirien le 10 septembre 2019, soit plus de 60 ans plus tard. La République française, par la promesse de son président, s'était engagée en 2023 à un rapatriement rapide. Nous sommes en 2025 et il fallut l'an passé la mission en Côte d'Ivoire d'une délégation de la Commission de la Culture du Sénat pour que ce dossier connaisse enfin un dénouement heureux. Une nouvelle fois, il revient donc au Sénat de jouer un rôle décisif dans une restitution. Historiquement, Madame la Ministre, c'est ici au Sénat que cette cause fut plaidée pour la première fois et je rends un image appuyé au travail fondateur de notre collègue Catherine Morin d'Esaïe qui, bravant la ferme opposition de l'institution muséale et l'habileté obstructive des ministères de la culture successif, déposa en 2008 une proposition de loi permettant le retour des têtes Maori. Depuis, deux lois cadres ont été votées quatre cadres ont été votés. Nous attendons toujours la troisième qui devrait nous éviter de voter dans l'urgence de nouvelles lois de circonstance. En commission et de nouveau ici, Madame la Ministre, nous avons entendu votre engagement à nous transmettre rapidement ce texte. Madame la Ministre, nous sommes prêts à l'examiner sans tarder. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Mathilde Olivier pour le groupe écologiste Solidarité et territoire. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, chers collègues. La restitution n'est pas une faveur, c'est un droit. Ces mots de l'universitaire et commissaire d'exposition sénégalaise Engo Neffal doivent résonner aujourd'hui dans le cadre de nos débats. Le bien culturel dont il est question, le tambour-parleur ou Jiji Ayo-kwe, n'est pas seulement l'une des nombreuses pièces que compte le musée du quai Branly. Il est le stigmate sensible d'une histoire longue, douloureuse et encore vive. celle de la domination coloniale, de la dépossession et du mépris culturel systématique. Pendant des décennies, la France a construit une part de son prestige en pillant les terres, les richesses et les symboles des peuples qu'elle prétendait entre guillemets « civilisés ». La Côte d'Ivoire, comme tant d'autres nations africaines, a subi cette histoire dans sa chair, dans ses institutions et plus encore dans sa mémoire. La restitution dont il est question aujourd'hui dans cet hémicycle est un signe de bon sens, que je souhaite saluer au nom du groupe Ecologistes Solidarité et Territoires. Alors que ce bien est officiellement réclamé depuis 2019 par le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, il est satisfaisant que cette demande soit mise à l'ordre du jour six ans après. Mais mes chers collègues, nous en sommes toutes et tous conscients, l'enjeu aujourd'hui est bien plus grand. Les restitutions aux comptes-gouttes, qu'il s'agisse du tambour-parleur, des trésors royaux d'Abomé ou du sabre avec fourreau, dit Eladj Omar Thal, opéré au cours de ces cinq dernières années, sont insuffisantes. Emmanuel Macron s'était engagé à l'occasion du discours de Ouagadougou en 2017 à ce que, d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Rappelons simplement qu'à l'heure actuelle, 90 à 95 % du patrimoine africain se trouve en dehors du continent. En 2023, les deux premiers textes du paquet législatif sur la restitution des restes humains et des biens culturels spoliés pendant la guerre par les nazis ont été adoptés sous l'impulsion de l'ancienne ministre de la Culture, Madame Rima Abdulmalak, et de nos collègues ici au Sénat. À l'époque, le gouvernement et les forces en présence dans cet hémicycle s'y étaient engagées. Ces deux premiers textes devaient être suivis d'un texte sur la restitution des biens culturels. Nous le savons tous ici, le texte est prêt. Il est sur votre bureau, Madame la Ministre, depuis des mois déjà. Alors je vous le demande, où en sommes-nous ? Pourquoi cette loi cadre a-t-elle si subitement disparu des radars de l'ordre du jour ? Madame la Ministre, chers collègues de la majorité sénatoriale et du Soc le commun, il est de votre responsabilité d'accorder vos violons et qu'enfin, cette loi soit mise à l'ordre du jour. à la fois pour tenir les engagements que vous avez pris et parce que je pense que nous serons tous d'accord ici, nous ne pouvons pas avancer sur la question de la restitution des biens culturels par loi d'espèce et à coup en fonction de bonnes volontés diplomatiques. Nous avons besoin d'un processus définissant des critères clairs permettant de définir la spoliation coloniale et par conséquent de faire la différence entre les acquisitions légitimes et illégitimes. de la mise en place d'un cadre pour les commissions scientifiques chargées de déterminer la provenance, le contexte de l'acquisition ou de la spoliation des biens culturels, et d'une définition de quand, comment et à qui les biens culturels seront rendus. Partout en Europe, de l'Allemagne au Pays-Bas, en passant par la Belgique, les États débiteurs d'un passé colonial se sont engagés dans ce travail mémoriel. Ne soyons pas à contre-courant de l'histoire, qu'attendons-nous ? Le principe d'inaliabilité des collections publiques est un principe important, permettant de sortir du marché des biens culturels et de les protéger. La restitution répond quant à elle à des enjeux extrêmement forts historiquement, socialement et culturellement. Nous devons donc concevoir la restitution comme une dérogation aux principes d'inaliabilité fondamentale au processus de réparation et de travail de mémoire que nous devons conjointement mener avec les pays et peuples colonisés. C'est la condition à une collaboration avec les États qui développent des infrastructures muséales d'ampleur comme nous l'avons vu lors du déplacement de la Commission culture du Sénat en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ces œuvres revêtent une signification majeure pour les peuples qui en ont été spoliés. le démontrent la restitution des trésors royaux du palais d'Abomé au Bénin et leur exposition à Cotonou qui a attiré en un temps record des dizaines de milliers de Béninois. Il faut que les Ivoiriens puissent enfin, eux aussi, avoir accès à leur patrimoine culturel. Nous le savons, la mise sur pied d'une politique de restitution des œuvres indiments issues de la colonisation ou des guerres est indispensable pour l'avenir de nos relations. Ce que nous faisons n'est que l'occasion pour la France de réparer et de réinventer sa relation avec l'Afrique, comme le rappelait très justement le philosophe et historien camerounais Achille Mbembe. Le travail de réparation et de mémoire que nous devons accomplir en tant que nation à l'égard des pays que nous avons colonisés par le passé ne peut se satisfaire d'une loi d'espèce à l'image de celle dont nous discussionnons aujourd'hui. Le groupe Ecologie, Solidarité et Territoires votera en faveur de cette proposition de loi relative à la restitution d'un lien culturel à la République de Côte d'Ivoire et demande plus largement à enfin mettre à l'ordre du jour cette loi cadre tant attendue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, c'est un honneur de m'exprimer aujourd'hui sur cette proposition de loi transpartisane relative à la restitution du tambour DJI-Yokuei à la République de Côte d'Ivoire. Et de le faire devant M. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, de son excellence, M. Maurice Kouakou, bandamane, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, de M. Ibrahima Diabaté, président du Conseil national de la jeunesse et d'une délégation ivoirienne, accompagné de notre conseiller élu des Français de l'étranger à Abidjan, monsieur Baptiste Heinz, que je chaleureusement. Cette proposition de loi fait suite aux déplacements que nous avions effectués en Côte d'Ivoire. En septembre dernier, avec le président Laurent Lafont, et nos collègues Max Brisson, Cédric Vial, Jean Ingré et Mathilde Olivier. À cette occasion, nous avions rencontré la ministre de la Culture ivoirienne, madame Françoise Remarque, qui avait renouvelé officiellement la demande de restitution du tambour Jiji Ayukwe. Nous avions aussi effectué une visite du chantier du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, actuellement réaménagé en vue d'accueillir le Tambour. Ce fut l'occasion de constater la formidable mobilisation des acteurs ivoiriens et français engagés dans le processus de restitution et les moyens et les moyens financiers et humains déjà investis dans la coopération culturelle et muséale entre nos deux pays. C'est donc de façon unanime que nous avions décidé à notre retour de déposer cette proposition de loi. Il s'agit d'abord de tenir l'engagement de la France puisque le président de la République avait confirmé à l'occasion du sommet Afrique-France de 2021 que le Tambour avait vocation à être restitué à la Côte d'Ivoire. Il n'était plus acceptable que le processus de déclassement du Tambour soit au point mort depuis trois ans. Ces retards suscitent l'incompréhension en Côte d'Ivoire et dans la diaspora ivoirienne de métropole. Il s'agit aussi de réparer une faute morale. Le dji-dji ayokwe est un objet sacré du peuple hachang. Ce n'était pas qu'un instrument de musique servant à produire des sons, c'était aussi un instrument de résistance. Il était censé donner des informations sur le positionnement des ennemis dans la forêt et l'on dit qu'il servait à prévenir les villages lorsque les colons français venaient réquisitionner les populations pour le travail forcé. Or, ce tambour parleur fut réduit au silence en 1916, lorsque l'administrateur colonial Marc Simon le dérobât à la communauté Bijan. Pendant 15 ans, en guise de représailles, il fut déposé dans les jardins de sa résidence, dans de piètre condition, exposé aux intempéries, ce qui l'a grandement détérioré. La restitution du DJI au Quai n'est donc pas qu'un acte administratif ou juridique. C'est un acte moral, de justice, de réparation et de reconnaissance de la vérité historique. Par cet acte, nous, les représentants du peuple français, rendons à leurs propriétaires le tambour parleur, mais nous reconnaissons aussi le témoignage de la domination et des violences coloniales qu'ils constituent. Nous avons pu constater, lors de notre voyage, que la restitution de ce bien culturel faisait l'objet d'un travail remarquable de formation et de mise en récit historique en lien avec la communauté Hatchant. Nous aimons-t-on le souhait que ces restitutions de biens culturels, encore trop peu nombreuses, fassent l'objet d'un travail historique et pédagogique approfondi dans notre pays aussi et qu'elle serve de support à un meilleur enseignement de notre histoire coloniale. Cela aussi contribuerait à créer les conditions du pardon, de la colonisation, pour reprendre l'expression utilisée la semaine dernière par le président de la République en déplacement à Madagascar. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons cette proposition de loi avec conviction et parce que c'est le devoir de notre assemblée d'honorer la parole de la France. Merci, la parole est à madame Laura Darkos pour le groupe Les Indépendants, République et territoire. M. le Président, Mme la Ministre, M. l'Ambassadeur, M. le Président de la Commission, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi pour la restitution du tambour-parleur Gigi Ayokwe à la Côte d'Ivoire. Cette restitution répond à une attente de longue date de la communauté Hatchan, communauté d'origine du tambour-parleur, pour laquelle celui-ci est sacré. Elle relève aussi d'enjeux diplomatiques, culturels et juridiques. Au-delà, cette restitution participe de la consolidation de notre relation à la société civile et à la jeunesse ivoirienne. En ce sens, je tiens à saluer l'initiative transpartisane qui a mené à cette proposition de loi, et en particulier le travail de nos collègues Laurent Lafont, Max Brisson, Catherine Morin de Sailly, Pierre Ousoulias, Yann Chantrelle, Jean Ingré, Mathilde Olivier et Cédric Vial. Sur le plan diplomatique, cette restitution est prioritaire. La Côte d'Ivoire, pays ami avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, l'attend depuis des années. Confisquée en 1916 et conservée dans des collections françaises depuis 1930, ce bien est réclamé par sa communauté d'origine depuis des décennies. En 2019, la Côte d'Ivoire a fait une demande officielle en ce sens. La France s'y était engagée à y donner suite lors du sommet Afrique-France de 2021. La restitution n'a pourtant toujours pas eu lieu, alors que le Sénégal et le Bénin, eux, ont bénéficié de presse d'opérations de restitution il y a peu. Sur le plan culturel, cette dernière est essentielle. Depuis 2022, plusieurs opérations préparatoires ont été menées à cet effet par le Musée du Quai Branly. Celui-ci a accueilli la communauté Hatchan pour une cérémonie de désacralisation préalable à la restitution. Une coopération muséale d'ampleur a aussi été mise en place avec le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement et Expertise France. Cette restitution fait aussi écho au renforcement de nos relations avec la société civile ivoirienne, en particulier sa jeunesse. De nombreux projets réunissant nos deux pays ont déjà vu le jour, comme le HUB franco-ivoirien pour l'éducation, rendre le tambour parleur au peuple ivoirien contribue aussi ainsi en ce sens à ces initiatives destinées à la jeunesse ivoirienne. Le 7 juin 1978, l'appel d'Amadou Matar Ambo pour, je cite, « le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable » a marqué les esprits. Il y rappelait à quel point certains biens culturels participent de la mémoire collective de leur peuple d'origine. Pour cette jeunesse ivoirienne qui aspire à mieux connaître ses racines, la restitution dont nous débattons aujourd'hui revêt une dimension particulière. A nous d'agir pour que la France honore cet engagement. A cet effet, le groupe Les Indépendants salue la restitution du tambour à la Côte d'Ivoire, dont je rappelle la légitimité, la nécessité et l'urgence au regard du retard que nous avons déjà pris. Néanmoins, nous regrettons que cela ne se fasse pas au travers d'une loi cadre, comme l'a répété beaucoup de mes collègues. En effet, afin de procéder à cette restitution, le présent texte prévoit une dérogation à l'article L451-5 du Code du patrimoine qui consacre le principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises. Cette méthode, si elle se justifie pleinement par le contexte, présente des écueils. Si nous continuons de procéder à des restitutions via des dérogations au principe d'inaliénabilité, alors nous réduisons la portée juridique de ce principe pourtant essentiel. Ce principe tire ses racines de l'ancien régime. Il a été consacré par la Cour d'appel de Paris en 1846, la Cour de cassation en 1896, le Conseil d'État en 1932 et pour les collections des musées publics par la loi du 4 janvier 2002. Ce principe protège notre patrimoine. Il ne doit pas être traité avec légèreté. Or, à l'automne 2018, les collections publiques françaises comptaient au moins 88 000 objets provenant d'Afrique subsaharienne. Parmi eux, certains devront être restitués à leur pays d'origine. C'est un fait. Ferons-nous des lois de dérogation à chaque fois ? Cette méthode n'est souhaitable ni pour les peuples africains ni pour nous. Nous avons besoin d'une loi cadre. La question de la restitution des biens culturels aux pays africains est posée depuis plusieurs années. pouvoir plusieurs décennies. En 1982, déjà le ministère des relations extérieures français chargait Pierre Cognam de former un groupe de travail à cet effet. Un nouveau rapport paru en novembre 2018 et réalisé par Félix Nsart et Bénédicte Savoie dresse un constat exotif et sans appel sur ces enjeux. La société civile s'est aussi emparée à juste titre de cette problématique qui appelle une réponse à la hauteur. Et bien évidemment, je salue particulièrement les travaux depuis de nombreuses années de mes collègues Catherine Morin-Decahie, Max Brisson et Pierre Ousoulia sur ce sujet. En définitive, le groupe Les Indépendants apporte tout son soutien à cette proposition de loi et salue le travail mené par nos collègues. Il insiste néanmoins sur la nécessité qu'une vraie loi cadre sur ces enjeux soit adoptée à terme. Je vous remercie.

Leur présence est importante, elle témoigne aussi de l'importance que revêt le retour du tambour pour la Côte d'Ivoire. que nous réjouir de ce texte d'aujourd'hui et du très large consensus et d'une unanimité autour de ce retour. Nous avons à travers ce texte corrigé une anomalie, anomalie entre l'attente forte en Côte d'Ivoire, l'attente qui était accompagnée de travaux dans le Musée des civilisations et d'un partenariat tout à fait exemplaire entre les historiens et les scientifiques ivoiriens et français, et l'attente d'un véhicule législatif permettant ce retour. Avec ce texte, avec cette loi spécifique, cette anomalie est désormais corrigée. Moi je voudrais d'abord remercier les parlementaires Tout ce qui ont pris part à ce texte, en particulier ceux qui ont composé la délégation transpartisane, ce qui montre aussi que la diplomatie parlementaire permet d'obtenir des résultats, je tiens à le souligner. Ça lui est bien sûr Catherine Morin de Sailly qui mène sur la question des restitutions à un travail de longue date auquel se sont associés Max Brisson et Pierre Ouzouyas pour faire en sorte que le Sénat, sur ce sujet-là, soit une vraie référence. Remercier aussi Madame la Ministre qui a tout de suite réagi quand nous sommes venus la voir notre tour de Côte d'Ivoire pour accélérer le processus de restitution à travers cette loi spécifique. Merci de votre écoute et de votre intervention tout à fait utile pour avancer sur ce sujet. Nous avons bien noté votre annonce sur la loi cadre. Elle nous paraît, vous l'avez compris mais je le dis aussi, tout à fait indispensable pour avancer. Nous l'attendons de longue date. Sachez qu'ici, vous trouverez dans cet hémicycle un lieu de dialogue serein, constructif, pour avancer sur ce sujet. Et bien entendu, s'il venait au gouvernement la bonne idée de commencer le travail parlementaire sur cette loi cadre ici au Sénat, nous en serions tout à fait heureux. Merci Monsieur le Président. Je mets au voie la proposition de loi relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La proposition de loi est adoptée. Je vais suspendre Je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur l'intelligence artificielle. La parole est tout d'abord à l'orateur qui a demandé ce débat, en l'occurrence Monsieur Stéphane Piennoir, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Monsieur Piennoir. Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il ne se passe désormais plus une seule journée sans que l'on évoque le sujet de l'intelligence artificielle. Les médias, bien sûr, en parlent abondamment, des experts nombreux sont consultés dans les différents colocs. Elle donne aussi lieu à des débats quotidiens sur les lieux de travail dans les écoles, dans les universités et jusque dans le cadre familial. On dit beaucoup de choses, parfois exactes, souvent approximatives et superficielles. On anticipe le pire ou le meilleur avec, me semble-t-il, un manque de nuance et surtout de compréhension. L'IA est à la fois omniprésente et insaisissable. Elle fascine et inquiète en même temps. C'est pourquoi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et la délégation à la prospective, qui ont l'un et l'autre récemment travaillé en profondeur sur l'IA avec des approches très différentes, ont demandé conjointement ce débat. Christine Labarde, présidente de la délégation à la prospective du Sénat, qui conclura ce débat, nous souhaitions que le Sénat puisse discuter avec le gouvernement en séance publique des orientations que notre pays doit prendre sur un sujet devenu hautement stratégique. Pour l'Office, le rapport récemment publié était une commande du plus haut niveau parlementaire à l'occasion du 40e anniversaire de l'Opex, puisque les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont conjointement décidé de travailler sur les nouveaux développements de l'IA, à l'heure du déploiement donc incroyablement rapide de l'IA générative notamment. Je salue en particulier le travail approfondi de nos deux collègues co-rapporteurs, Patrick Chaise qui posera une question tout à l'heure et Corinne Narasiguin qui est retenue me semble-t-il aujourd'hui, et vous engage à lire ce rapport un peu ardu, certes, mais essentiel pour comprendre ce que peut et ce que ne peut pas faire l'IA. Il évoque aussi les différentes problématiques soulevées par l'IA qui transforment nos sociétés, nos économies, mais aussi les rapports de force politique et géopolitique. La puissance des entreprises technologiques américaines, Google, Microsoft, Amazon, Meta, auxquelles j'ajoute Nvidia, est désormais bien connue de tous. L'aspiration de la Chine à devenir leader mondial dans le domaine d'ici 2030 apparaît à travers des annonces régulières et fortes. Dans ce contexte, le défi pour l'Europe et notamment pour la France est celui de la souveraineté numérique afin d'éviter de devenir une pure et simple colonie numérique. L'Union européenne mise aujourd'hui sur sa régulation, mais contrée la domination de la Big Tech américaine, appelle au développement d'acteurs français et européens réellement puissants. Lors du sommet de l'intelligence artificielle qui s'est tenue en février dernier à Paris, une coalition de plus de 60 entreprises européennes a été créée pour traduire dans les faits l'urgence d'une réaction européenne forte. Madame la Ministre, vous pourriez nous indiquer tout à l'heure où en est cette initiative, quelles visions et quelles stratégies l'Europe et la France ont-elles déterminées et mises en place depuis ? Y a-t-il un plan d'action précis et financé, vous semble-t-il encore possible, de se placer dans cette course effrénée où chaque mois compte ? Cette stratégie européenne apparaît d'autant plus nécessaire que les manipulations politiques et les atteintes à la sécurité à grande échelle créées à partir de l'IA prennent une ampleur chaque jour plus importante. Les équivalents européens de l'Opex ont d'ailleurs consacré leur dernière réunion à ce sujet, IA et démocratie, et j'ai pu constater à cette occasion les vives inquiétudes partagées par nos collègues. Plus insidieuse encore est la domination culturelle que les systèmes d'IA permettent. Dominés par des acteurs anglo-saxons, ceux-ci risquent non seulement d'accentuer fortement l'hégémonie culturelle des États-Unis, mais aussi, plus grave, de favoriser une forme d'uniformisation cognitive en appauvrissant la diversité culturelle et linguistique. Il est urgent d'avoir des systèmes d'IA entraînés avec des données en français et construits autour de nos valeurs. Madame la Ministre, comment le gouvernement s'est-il emparé de cette priorité, notre exception culturelle régulièrement invoquée dans les discours, est cette fois-ci réellement en danger et les évolutions sont de plus en plus rapides Comment garantir que l'IA s'aligne sur nos valeurs, respecte les droits de l'homme et les principes humanistes ? Par ailleurs, dans le domaine scientifique, l'IA recèle de vraies promesses en s'intégrant à toutes sortes de disciplines. Elle ouvre des perspectives immenses comme en témoignent quelques exemples, les exemples de la génomique ou de la création de jumeaux numériques. Ces avancées permettront de résoudre, j'en suis sûr, des problèmes complexes et d'accélérer les découvertes. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas anodin que les prix Nobel 2024 de physique et de chimie soient revenus à des chercheurs en IA. Les bénéfices de ces technologies nécessitent donc une adaptation de nos politiques de recherche. Et là encore, Madame la Ministre, vous pourrez nous dire les mesures prises pour aider nos scientifiques à s'emparer et à disposer de ces outils pour développer et accélérer certaines de leurs recherches. Alors, des tas de promesses ont été faites au cours des dernières années, il faut le dire, des moyens financiers à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, la création de 9 pôles d'excellence en IA, la formation jusqu'à 100 000 personnes, mais l'exécution n'est pas au rendez-vous, nos mesures ne sont pas suffisamment coordonnées et surtout souffrent d'une absence de pilote, comme l'a récemment souligné la Cour des comptes. Madame la Ministre, vous êtes l'une des premières au monde à avoir dans l'intitulé de votre poste les mots intelligence artificielle. Mais avez-vous pour autant l'autorité et les moyens nécessaires pour piloter cette politique stratégique ? Avez-vous autorité sur les services ministériels et notamment ceux de Bercy, qui négocient dans le cadre européen la politique de l'IA ? Êtes-vous en contact direct avec vos homologues qui ont une vision proche des nôtres ? de la nôtre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie ou l'Espagne. Un rapport récent, celui de Philippe Aguillon et de Anne Bouvereau, parle de cette nécessaire coordination nationale et européenne. Il propose un investissement massif de 27 milliards d'euros sur cinq ans pour la formation, la recherche et le développement d'un écosystème robuste en IA. La baumilisation de telles sommes paraît complexe dans le contexte budgétaire actuel, mais avez-vous néanmoins retenu quelques mesures préconisées ? Vous l'aurez compris, notre principale interrogation concerne la stratégie de notre pays en matière d'IA pour aujourd'hui et pour demain. Et je le redis, il y a urgence. C'est l'aspect qui faisait l'objet des toutes premières recommandations de l'Office. S'y ajoutez quelques-unes que je vous livre. D'abord une indispensable régulation mondiale de l'IA actuellement éparpillée entre différents organismes. Il nous semble essentiel essentiel que l'Union Européenne prenne rapidement le leadership sur cette question. Elle a déjà commencé évidemment à élaborer un cadre juridique pertinent en lien étroit avec l'OCDE. Deuxièmement, l'Office estime prioritaire d'accompagner le déploiement de ces technologies dans le monde du travail, de prévoir l'impact précis qu'elles auront avec des outils d'IA qui sont déjà présents et veillent des inquiétudes. Enfin, et cela nous semble majeur, il faut former les élèves, les écoles, les collégiens, les lycéens, les étudiants des universités et former plus largement le grand public la connaissance du fonctionnement de ces technologies, des conséquences et des risques notamment de manipulation, nous paraît essentiel. Voilà, mes chers collègues, les axes principaux que je souhaitais évoquer pour introduire ce débat, donc je ne doute pas qu'il sera particulièrement riche et intéressant. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. La parole est à madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs, vous l'avez très bien posé, plus un jour ne passe sans que nous entendions parler d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, deux Français sur cinq disent l'avoir déjà utilisé. Orlia n'est pas qu'une innovation technologique de plus. Elle modifie une façon de produire, de décider, de comprendre le monde et donc, inévitablement, de gouverner. C'est bien pour ça d'ailleurs que la France s'est dotée d'un ministère de l'IA, comme nous avons pu nous doter le moment venu d'un ministère des postes, des télécommunications, du numérique. C'est parce que cette technologie est si puissante qu'il nous faut mettre les moyens pour la gouverner. Je salue le travail des parlementaires et bien sûr celui de l'OPEX qui a rendu un rapport très complet, je ne dirais pas si ardu, sur l'IA qui me semble absolument nécessaire pour que nous puissions nous approprier les défis qui sont devant nous avec cette technologie. Car oui, nous ne sommes pas simplement confrontés à une nouvelle technologie, nous faisons face à une redistribution profonde des pouvoirs économiques, scientifiques, cognitifs. Et dans ce moment, ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement notre compétitivité, c'est notre capacité collective à orienter le progrès, à lui donner un sens, à rester maître de nos choix. L'intelligence artificielle cristallise tous les défis du XXIe siècle. La souveraineté, la démocratie, la transition écologique, l'éducation, la justice sociale, et elle nous oblige à répondre à une question essentielle. Qui décide et au nom de quoi ? Giuliano d'Ampoli, pour ceux qui peut-être ont lu l'heure des prédateurs, compare les responsables politiques à Moctezuma face à Cortez, fasciné, dépassé, impuissant. Face à un pouvoir qu'ils ne comprennent pas, ils en sont réduits à vouloir impressionner par les apparences ces nouveaux maîtres du monde en les recevant dans les salons dorés de leur ministère. La comparaison est excessive, mais elle touche un point sensible. Oui, nous, politiques, nous avons parfois du mal à suivre la vitesse du progrès technologique. Oui, une poignée d'acteurs économiques concentre aujourd'hui une puissance inédite. Mais non, la puissance publique n'est pas condamnée à l'impuissance. Notre action est claire, développée, encadrée, orientée, corrigée, agir. C'est pour cela que l'IAT est un sujet politique et c'est pour cela que le gouvernement en a fait une priorité de son action. Le gouvernement agit pour faire de la France une championne de l'IA. C'est le fruit du travail que nous menons depuis 2018 avec la toute première stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui a permis d'investir plus de 2 milliards et demi d'euros sur toute la chaîne de la recherche à l'entreprise. En recherche d'abord, nous avons 14 médailles field, des talents qui nous sont reconnus dans le monde entier, que nous avons renforcés avec le lancement de 9 clusters IA partout sur le territoire, Arene, Sofia, Nancy, avec un budget de 360 millions d'euros dédié à former près de 100 000 personnes par an d'ici 2030. Nous avons développé notre capacité de calcul publique avec Jean Zay, notre calculateur. Nous avons attiré les meilleurs centres de recherche mondiaux, les plus brillants du monde, de DeepMind à OpenAI. Ces centres ont essaimé, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 startups, dont bien sûr Mistral AI, Hugging Face ou encore Ackemia, dans le domaine de la santé. Ces startups sont reconnues dans le monde entier et elles nous permettent d'être dans cette course mondiale et d'offrir une troisième voie entre les États-Unis et la Chine. En février dernier, vous l'avez mentionné, s'est tenu le grand sommet pour l'Action sur l'IA, un événement d'ampleur mondiale ici, en France. Il a marqué une nouvelle étape décisive. Pour la France, d'abord, ce fut l'occasion de lancer la troisième étape de notre stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et de lancer le comité interministériel de l'IA sous l'égide du Premier ministre. Ce comité répond à certaines de vos interrogations car vous avez raison, l'IA n'est pas seulement un enjeu économique mené par les ministères de Bercy et les administrations de Bercy qui nous appuient sur le développement de politique publique sur cette question mais bien un enjeu imminemment interministériel. Le Premier ministre nous a mobilisés chacun sur nos périmètres respectifs pour avancer et coordonner cette stratégie de l'intelligence artificielle et répondre à ce rapport que vous avez mentionné d'avril 2023. L'ampleur du sujet, les moyens sont donc bel et bien mis et nous sommes, je vous le garantis, bien tous à la tâche pour avancer. Ce sommet a aussi été l'occasion d'annoncer 109 milliards d'euros d'investissement pour développer l'IA et ses infrastructures nécessaires à la puissance de calcul ici en France. Pour l'Europe, c'est près de 200 milliards d'euros d'investissement qui ont été dévoilés pour réaffirmer notre ambition d'innovation. Et pour le monde, nous étions attendus. Nous étions attendus pour fixer un cap à cette gouvernance mondiale dont vous avez parlé aussi dans votre rapport. Gouvernance mondiale pour orienter cette technologie avec des actions très concrètes. La création de la fondation Current AI dotée de 400 millions d'euros pour financer des IA d'intérêt général, la signature d'une coalition mondiale pour une IA durable ou encore la déclaration commune que vous avez citée qui rassemble 62 pays pour une IA inclusive et éthique. Dorénavant, l'enjeu crucial dans cette course, c'est l'adoption. Ma priorité, c'est de faire de la France une championne de l'IA, mais bien pour permettre à chacun de s'en en parler. C'est une des conditions de la compétitivité de notre économie. C'est surtout une nécessité pour construire une société inclusive dans laquelle l'innovation bénéficie à toutes et tous. L'IA transforme déjà nos vies. Je l'ai observé partout en France. À l'hôpital à Bourg-en-Bresse, c'est un médecin qui détecte une embolie pulmonaire À l'école, à Quimper, c'est un lycéen dyslexique qui, grâce à un surlignage automatique, comprend enfin ses cours. Dans une ferme, dans les Ardennes, c'est un agriculteur qui arrose moins, récolte plus. Dans les bureaux de Bercy, c'est un agent de la DGFIP qui peut mieux cibler ses dossiers. Et dans les Maisons France Service, comme à la mode Cervelex, c'est un agent qui répond plus facilement aux usagers. Dans le monde du travail, elle facilite la prise de notes, la rédaction, accélère la rédaction de contrats, optimise les plannings, simplifie les démarches administratives. Pour autant, elle suscite toujours certaines craintes chez nos concitoyens. Et n'est pas utilisée par toutes et tous. La question d'âge, d'abord, quand 7 jeunes de 18 à 24 ans sur 10 utilisent l'IA quotidiennement, ce chiffre tombe à moins de 2 sur 10 pour les plus de 60 ans. En entreprise, 5 petites et moyennes entreprises sur 100 seulement utilisent l'IA au quotidien, quand c'est près de 35% des grandes entreprises. Et les études sont unanimes. À l'échelle du pays, nous ne sommes pas en avance en matière d'adoption. Or, l'IA ne serait un progrès qu'à condition de ne pas être réservé à une minorité. J'ai fait de ma priorité d'en faire un outil d'émancipation, un moyen de résorber la fracture numérique. Et c'est pourquoi nous organisons des milliers de cafés partout sur le territoire. Et parce que l'adoption réussie se fera en guidant notre jeunesse, dès la rentrée, des cours seront intégrés en quatrième et en seconde pour aider les élèves à utiliser l'IA, mais surtout à la comprendre et à développer leur esprit critique. Pour finir, je voudrais aussi parler de la nécessité de comprendre, d'orienter l'IA sans entraver l'innovation. Répondre aux risques, aux défis que nous avons à affronter en face en créant un institut qui permet de mieux comprendre ces modèles et en s'appuyant sur la réglementation européenne. Oui, l'Europe régule. J'entends souvent les railleries qui disent que l'Europe régule. Mais en matière d'intelligence artificielle, nous avons décidé de façon déterminée, en européen, que ce ne soit pas la loi du plus fort et de nous noter d'un texte qui nous permet de déterminer les usages anodins anodins et les usages strictement interdits comme une IA qui déterminerait l'orientation sexuelle de toutes les personnes dans cet hémicycle. En Europe, nous n'en voulons pas. L'IA française, l'IA européenne n'est pas subie, elle est innovante, performante, compétitive, fidèle à nos valeurs. C'est bien ce qui fait sa puissance, une tech au service de l'humain et de notre prospérité. Je vous remercie. Le gouvernement dispose pour répondre d'une durée équivalente. Le gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de répondre à une réplique éventuelle pendant une minute. L'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute. Je rappellerai si nécessaire. La parole pour la première question est à Mme Marie-Laure Finérat-Hort du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, les chers collègues. À ce jour, trois rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ont déjà abordé l'intelligence artificielle. Le dernier analyse les technologies actuelles et les grandes tendances à venir. Parmi les enjeux sociétaux, culturels et parfois juridiques, notamment en matière de droit coutumier au local, figure la reconnaissance, la traduction et la restitution de nos langues régionales patois, créoles, langues autochtones. Avec environ 15 millions de locuteurs dans le monde, les langues créoles représentent un enjeu sur lequel la France peut se positionner en tête, notamment en Europe. En France, près de 2 millions de personnes parlent quotidiennement des créoles à base lexicale française. Plus de 80% à La Réunion, plus de 70% aux Antilles. En Guyane, les créoles guyanais et haïtiens forment un lien linguistique partagé entre les différentes communautés. Conformément à la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de de 2005, un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité. Je salue d'ailleurs ici le travail initié par les associations ultramarines grâce auquel une épreuve de créole est proposée au bac partout en France depuis 2011. Interrogée sur le créole, l'IA reconnaît ses limites faute de données suffisantes contrairement aux français ou à l'anglais. Les créoles encore aujourd'hui à l'étude linguistique pour préciser leurs constructions et pour lesquelles l'apprentissage de l'écrit progresse nécessite une attention particulière pour éviter les approximations ou pire des clichés nuisibles à notre imaginaire collectif. En s'appuyant sur ces talents académiques et littéraires, notamment ultramarins pour constituer un socle de données structuré, la France peut faire réunionner le créole à travers l'IA, créant ainsi des ramifications à tous niveaux, en renforçant les liens entre les générations, de part et d'autre entre l'Hexagone et les Outre-mer, mais aussi des liens entre l'Europe et ses régions ultrapériphériques. En somme, des liens entre la France des cinq océans et le monde. Madame la Ministre, pouvez-vous me dire comment l'État entend s'emparer de ce défi qui permettra une meilleure compréhension et diffusion de notre culture plurielle ? Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, je vous remercie pour cette question. C'est une question fondamentale dans ce que je disais tout à l'heure. La question de développer nos intelligences artificielles européennes, c'est bien pour protéger nos valeurs et au centre de ces valeurs, la richesse de notre patrimoine linguistique est évidemment fondamentale. Nous avons lancé avec ma collègue Rachida Dati, le 20 mars dernier, un altédic qui vise exactement à faire ça au niveau européen, mettre en commun des moyens mais aussi des bases de données pour pouvoir avoir de la matière sur laquelle nos modèles vont pouvoir se déployer pour répondre à la richesse linguistique européenne et bien sûr la richesse linguistique française. Et donc avec les moyens qui seront développés, 88 millions d'euros pour ce projet, aurons les moyens de pouvoir avancer et répondre aux rapports que vous avez mentionnés. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Avec mon collègue Christian Bruyens, nous avons remis un rapport sur l'intelligence artificielle et l'éducation dans le cadre de la délégation à la prospective. Nous recommandions trois axes, un pour mieux accompagner les enseignants, le deuxième pour former à l'IA et favoriser l'émergence d'une culture citoyenne de l'IA, et un troisième sur l'évaluation et la poursuite de la recherche. Nous voulions garantir une évaluation indépendante des technologies d'IA mises à la disposition des enseignants et des élèves dans le cadre scolaire, créer un observatoire de l'IA à l'école permettant notamment la réalisation d'études de cohortes et de mieux comprendre en comprendre les usages, Et enfin, dans le cadre du du pilotage des politiques éducatives, mener une réflexion sur l'analyse à l'aide de technologies IA des données recueillies à l'occasion des évaluations nationales pour offrir, si ça s'avère pertinent, la possibilité de mieux les exploser. Parce que ces données sont quand même séquestrées par l'éducation nationale et c'est un véritable atout que l'on perd et dont on prive nos entreprises de tech qui sont assez performantes dans ce domaine. Merci Madame la Ministre. d'autant plus qu'on sait que les jeunes l'utilisent de plus en plus tôt et donc développer des outils pour accompagner non seulement les jeunes mais aussi les professeurs est nécessaire. Plusieurs réponses aux différents points que vous mentionnez. La question de la transparence est une question fondamentale. Je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure mais nous avons lancé à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ce qu'on appelle l'INESIA. C'est notre centre de recherche qui nous permet d'évaluer, de comprendre, de mettre de la transparence sur les modèles et nous pourrons lui confier un certain nombre de missions. Nous sommes en ce moment en train de définir la feuille de route et donc une attention particulière pourra être portée à l'éducation. Sur la question de l'Observatoire, il y a certaines choses en cours au niveau de l'OCDE afin de pouvoir bénéficier aussi de bonnes pratiques au niveau international. Et sur la question des outils que vous mentionnez à mettre à disposition des élèves et des professeurs, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un ami l'année dernière qui vise à recenser les différents outils qui pourront être déployés sur tout le territoire. Nous sommes en train de faire le bilan de cette première étape avec ma collègue, la ministre de l'Éducation. Et en train de préciser aussi dans les cours que j'ai mentionné mentionné pour les élèves de quatrième et de seconde, quelle sera l'approche, comment nous pouvons aussi... pouvoir apporter des réponses à toutes ces questions que se posent les élèves mais aussi les professeurs. Vous avez raison. Merci. Monsieur Fialer. même sur votre vigilance pour que l'on puisse utiliser et ne pas laisser séquestrer toutes ces données d'évaluation qui posent souvent des problèmes d'ailleurs aux enseignants qui doivent les faire, qui ont été d'ailleurs assez discutés et lorsqu'elles sont collectées elles servent à rien, rien n'en sort alors que c'est un réservoir extrêmement important de données qui peuvent permettre à nos entreprises qui sont assez performantes même au niveau mondial pour pouvoir faire des outils qui aideraient après nos élèves de culture française à faire des études en IA. Madame la Ministre, vous souhaitez... Très bien. La parole est à madame Catherine Morin de Saillie pour le groupe Union Centriste. Madame la Ministre, face aux opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, le risque c'est de voir comme pour le cloud se constituer une nouvelle hégémonie des big tech, accroissant un peu plus nos dépendances dangereuses. J'ai donc deux questions lors du sommet sur l'intelligence artificielle. Le Président de la République a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros. Comment ce plan se déclinera-t-il concrètement ? Va-t-on tirer les leçons du passé et admettre que les précédents plans n'ont pas permis de faire émerger un seul acteur de dimension internationale 80% des technologies utilisées en France sont américaines et les deux sols licornes sont majoritairement financées par les américains. Ensuite, je vous ai déjà interpellé au sujet du règlement sur l'IA. Ici même, il y a quelques semaines, Menemou n'avait pas répondu à mes questions qui portaient sur les dernières négociations du Code de Bonne Pratique. Plusieurs acteurs expriment leur colère face au poids disproportionné des Big Tech dans le processus de rédaction. Reporters Sans Frontières s'est d'ailleurs retiré des négociations puisqu'ont été évacués les enjeux informationnels. Les acteurs La Culture, soutenus par Rachida Dati, demandent eux aussi plus de garanties pour le respect des droits d'auteur et droits voisins. Quel est à vous votre position ?

il y a deux questions dont je tâche de faire la première et puis de basculer sur la seconde. La première, c'est la question de la souveraineté numérique. Vous savez, un sujet qui me tient fortement à cœur et qui pose une question qui va au-delà de l'intelligence artificielle. Je vous réponds sur les 109 milliards d'euros et puis nous aurons l'occasion de revenir sur la souveraineté numérique et technologique en général. Les 109 milliards d'euros d'investissements annoncés lors du Sommet pour l'action sur l'IA sont des investissements en infrastructures qui mélangent à la fois des consortiums de financeurs internationaux et nationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de suivi de ces projets et nous assurons de mettre en relation les entreprises françaises et européennes de datacenters pour qu'elles puissent créer des consortiums autour du financement de ces projets et créer une offre qui permette de répondre aux besoins de souveraineté. Comme vous le savez, la question des datacenters et de l'hébergement des données, l'approche qui a été la nôtre, c'est de s'assurer que nous avons une offre de cloud qui répond très très fort niveau de sécurité avec la certification Sectum Cloud et nous visons dans le même temps attirer ces moyens pour créer de l'infrastructure mais aussi continuer à soutenir avec la puissance publique la montée en puissance des acteurs européens du cloud et français notamment afin de pouvoir les accompagner à développer toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin. C'est pourquoi j'ai lancé la semaine dernière un appel à projets de plusieurs dizaines de millions d'euros sur cette question. Je vois le temps qui tourne, je passe sur le RIA. Les positions, vous l'avez dites, sont divergentes. Nous sommes encore dans une période de négociation. La Commission européenne n'a pas rendu les derniers arbitrages. Ma position est la suivante. Le règlement pour l'intelligence artificielle le Code of Practice et le modèle de transparence doivent rester fidèles à ce qui a été négocié, c'est-à-dire d'encadrer les usages et de permettre de pouvoir donner de la transparence sur les usages, notamment au risque. en respectant cet équilibre qui parfois est délicat à trouver, mais bien en s'assurant que les intérêts des petits acteurs, vous avez même mentionné les big tech, sont bien représentés. Je les rencontre très régulièrement dans mon ministère pour échanger avec eux sur leurs besoins et sur l'évolution de ce règlement pour l'intelligence artificielle et je serai très vigilante à ce que la voix de ces petits acteurs soit entendue et non pas seulement la voix des gros acteurs qui ont beaucoup de pouvoir de lobbying à Bruxelles. Concernant les droits d'auteur, Mais je pense que vous pourrez répliquer ensuite. Mme Morin de Sailly. Oui, Mme la Ministre, je crois qu'il faut vraiment investir, bien sûr, massivement, mais pour cela, la France doit vraiment mener une action concertée, volontariste, avec d'autres États membres de l'Union européenne. Il faut absolument revoir le plan Horizon 2030, construire une stratégie offensive et partager de soutien à la formation, la recherche et à nos entreprises, avec des programmes transversaux, financés inexistants aujourd'hui, grâce à des mécanismes innovants. Nos entreprises françaises et européennes doivent enfin compter sur le levier de la commande publique. L'action de l'État, désolé de le dire, en tant que prescripteur de la technologie, a été nulle et choquante. Encore récemment, l'enseignement supérieur avec Microsoft est au au mépris des dispositions contenues dans la loi SNED. Nous exigent désormais que cela chance. S'agissant de la mouture du texte IA, nous vous demandons urgemment de plaider vraiment pour la prise en compte des enjeux informationnels, des risques systémiques spécifiques et d'inclusion du droit à une information fiable et non trafiquée. Nous exigeons aussi l'arrêt du pillage actuel des données des journalistes

pour pouvoir trouver l'évolution dont on a besoin pour valoriser la richesse de notre patrimoine culturel dans l'heure de l'intelligence artificielle. Et nous y serons absolument attentifs, bien sûr. Vous souhaitez Je remercie la ministre pour sa réponse. Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux reprendre une partie des questions de ma collègue Catherine Morin de Sailly. Je les partage. Nous avions eu ensemble une première discussion le 10 avril, notamment sur la protection des droits d'auteur. Vous nous aviez dit à l'époque, et nous sommes tout à fait d'accord, qu'il fallait à la fois défendre le droit d'auteur, notre patrimoine, mais aussi notre capacité à innover. Tout le monde est d'accord avec ça. Il ne faut pas une réglementation prohibitive. De toute façon, elle ne pourrait pas être appliquée. En revanche, vous m'aviez dit à l'époque, nous ne sommes pas face à une question de transparence. Je vous cite. L'enjeu est bel et bien le modèle d'affaires. Je ne partage pas votre point de vue. Je pense au contraire que la transparence est quelque chose de fondamental. Il faut que les auteurs qui produisent des données sachent que leurs données ont été réutilisées par les GAFAM, il s'agit d'eux, largement, sans aucune rémunération. Ma collègue Catherine Morin de Sany l'a dit, il y a un pillage systématique structurelle, et qui est encouragée aujourd'hui par l'administration américaine. Il faut cesser notre irrednisme par rapport à ça et il faut absolument intervenir. Je vous l'avais dit à l'époque le 10 avril, ce matin, vous le savez, une agence américaine a envoyé un courrier à la Commission européenne pour lui dire que le code de bonne conduite qu'elle était en train de rédiger n'est pas satisfaisant. Les États-Unis, l'administration de Trump, refusera, refusent pour l'instant ce code de bonne conduite. Donc nous allons, c'est ma crainte, reculer sur la protection du droit d'auteur. Et pourtant, la directive était très peu contraignante sur le sujet, puisqu'elle parlait simplement, elle demandait aux plateformes de faire des efforts suffisants, des efforts suffisants pour respecter le droit d'auteur. Donc, je vous repose la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la protection du droit d'auteur ? Merci, cher collègue cher collègue président. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je remercie de me reposer cette question. Vous le savez, je suis attachée au droit d'auteur, j'ai eu l'occasion de le rappeler, nous avions déjà eu cette conversation c'est bien pour ça qu'on lance cette consultation avec ma collègue Rachida Dati. Il y a plusieurs moyens de vérifier ce que vous avez mentionné, notamment le droit à l'optaut et qu'il soit bien respecté. Et la question aussi de pouvoir donner l'information sur les données d'entraînement est bien sûr un des enjeux qui doit être discuté lors de la concertation mais je pense que la concertation doit nous aider à ne pas perdre de vue l'importance de trouver dans le modèle d'affaires comme je vous l'ai dit la dernière fois. le bon équilibre et nous permettre de trouver un enjeu gagnant-gagnant à la fois pour les auteurs et pour les innovateurs. ce n'est pas seulement une question de transparence et de modèle de transparence comme ceux qui sont discutés en ce moment au niveau de l'Union Européenne, mais bien aller plus loin et réfléchir ensemble grâce à cette consultation au modèle de rémunération. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Justine Sonnet pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. pas dire exponentiel, est en effet une révolution. Si la France ne veut pas louper ce tournant technologique, l'heure est à la décision et vous l'avez dit. Et pour ce faire, j'en appelle au nom du groupe écologiste au pragmatisme et à l'humilité. Au pragmatisme d'abord parce que face à des puissances mondiales tentées par la dérégulation sans limite, nous devons au contraire, avec nos partenaires européens, défendre un modèle régulé, souverain, transparent et respectueux des droits fondamentaux. Et à l'humilité ensuite parce que le développement illimité de l'IA dans toutes les dimensions de nos vies n'est aujourd'hui pas compatible, ni avec notre capacité de production électrique actuelle, ni plus généralement avec les limites planétaires. électricité aux terres rares liées à un coût écologique colossal. Et en complément des différents enjeux qu'a soulevé notre collègue Pied Noir en introduction, le secteur des data centers peu pouvoirilleurs d'emploi devrait voir sa consommation d'électricité doublée d'ici 2030. Il va donc falloir se fixer des priorités. J'en viens à mes deux questions Madame la Ministre. Quelles priorités comptez-vous fixer face aux risques réels de saturation du réseau électrique et ceux alors même que les besoins pour la transition énergétique vers les énergies décarbonées est en augmentation croissante ? Et enfin, quelles stratégies l'Etat compte-il adopter pour éviter les effets d'éviction par manque de disponibilité électrique sur le développement d'autres activités économiques et sociales plus pourvoyeuses d'emplois tels que la réindustrialisation ? Merci, je vous remercie pour cette question madame la sénatrice. Vous avez raison qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, la consommation énergétique des centres de données pourrait doubler d'ici 2026 et donc cela pose la question de comment nous réfléchissons à cet enjeu-là. La priorité qui est la nôtre, c'est déjà d'attirer les acteurs de l'intelligence artificielle et de donner aux acteurs de l'intelligence artificielle français et européens les capacités de s'entraîner en France parce que nous avons accès à une énergie décarbonée qui a un impact considérable sur la consommation de ces modèles. Mais c'est aussi et avant tout d'accélérer la recherche sur la question de la frugalité de ces modèles. mot pas très joli mais qui veut dire que nous sommes aujourd'hui au début de, enfin nous sommes pas au début mais nous sommes encore dans une phase où la recherche peut s'intensifier pour ces modèles et c'est ce que nous avons voulu aussi lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle avec la coalition pour une IA durable embarquer des acteurs, mettre les moyens pour faire avancer la recherche sur la question de la frugalité des modèles, avoir des plus petits modèles, avoir des data centers moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs d'eau. J'étais chez OVH la semaine dernière ou celle d'avant. Ils ont un système unique au monde qui utilise l'eau en circuit fermé pour pouvoir refroidir les data centers. Donc il y a encore beaucoup de recherche à amener pour s'assurer qu'on peut réduire et maîtriser cet impact des data centers et de l'intelligence artificielle. Et le ministère de la Transition écologique a d'ailleurs lancé des travaux pour définir ce que c'est qu'une IAF rugale sur toute la chaîne de malheur avec l'AFNOR et un AAP de 40 millions d'euros pour favoriser l'adoption de ces technologies par les collectivités.

d'intérêt général. Mais est-ce que finalement ce que l'on voit fleurir sur Internet, créer des oeuvres à la façon de Miyazaki, animer des photos d'être disparu ou choisir encore sa meilleure coiffure, qui va prendre énormément, énormément de place sur les data centers, sont-ils nécessaires ? Je pense qu'il va falloir également réguler les cas d'usage. ? Peut-être pour donner de la perspective, aujourd'hui on parle de 0,1% de la consommation, donc même s'il faut comprendre ces usages, les maîtriser, investir dans la recherche pour les maîtriser, l'enjeu du développement de cette technologie, de par nature parce que la technologie foisonne et que son usage est mis dans les mains de nombreux acteurs, sera multiple, divers avec des retours sur investissements énergétiques. si on peut le dire, variable. Pour autant, ça fait partie du cycle technologique de laisser chacun se l'approprier avec ses propres usages. Et je pense que pour accélérer l'adoption, c'est absolument fondamental. Maintenant, la question de la sensibilisation, encore une fois, de la compréhension. Et je crois qu'on fait un très bon travail d'ailleurs en France, médias, parlementaires, à pouvoir mettre le doigt sur ces enjeux écologiques et ce qui doit importer. Et dans la question d'ailleurs de l'éducation, Apprendre à mieux maîtriser cette technologie, à mieux prompter, c'est aussi s'assurer d'avoir des réponses plus efficaces et donc de moins dépenser en énergie. Donc tout va concorder pour accélérer en ce sens. ce sens. C'est dans la création des besoins que je suis inquiète parce que je ne doute pas qu'on ira effectivement vers des solutions qui te permettront d'utiliser moins moins d'énergie et de concentrer au maximum les data. Mais lorsque sur des jeunes, on va pouvoir les former aux UJAS et que sur internet, sur TikTok, on va les pousser à aller et jouer et créer ces besoins. Moi, je ne crois pas un seul instant que le courage politique sera en capacité d'amener d'amener à supprimer ces nouveaux divertissements qui sont en train de se faire et donc je crois réellement qu'il y a des décisions à prendre. il va falloir réellement réguler là-dessus parce que sinon ça deviendra un outil complètement ingérable et voilà, on aura que nos yeux pour pleurer une fois qu'on aura détruit toutes les ressources de ce monde. Merci, la parole est à la présidente Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En se dotant d'un règlement sur l'IA, l'Union Européenne, on le sait, a été pionnière avec une approche équilibrée. L'objectif était bien sûr que l'IA respecte les principes et les droits fondamentaux qui font lieu. Parmi les dispositions du règlement de l'IA, les obligations en matière de transparence, j'y reviens. s'avère absolument essentielle. Or, en termes concrets, et mes collègues Morin de Sailly et Osulias l'ont dit, cette transparence est loin d'être toujours effective. Et notamment dans le domaine culturel, elle est particulièrement lacunaire au point de porter préjudice à un principe auquel la France est séculairement attachée, qui est le droit d'auteur. Alors on a parlé du code de bonne pratique, La dernière version, vous le savez, publiée au mois de avril a braqué les ayants droits, qui estime à juste type qu'elle constitue un vrai recul par rapport aux précédentes moutures. Leur dépit est tel qu'ils songent même à claquer la porte des discussions en préférant un mauvais accord. finalement à une absence d'accord. Nous le savons, sur le droit d'auteur, la position de la France est décisive. Il faut absolument que le gouvernement ait une position très forte et non générale, en arrêtant d'arguer tantôt de soutien à l'innovation, tantôt de l'impérieuse nécessité de respecter le droit d'auteur. Madame la Ministre, Quelle est la position de la France dans les discussions actuelles relatives aux codes de bonne conduite ? Vous y avez déjà répondu mais j'aimerais que vous alliez plus loin. Quel niveau de transparence préconisez-vous ? Et quelle garantie apportez-vous aux ayants-droit avec quel mécanisme de juste répartition de la valeur ? Prenez-vous. Merci. Je vous remercie pour cette question madame la sénatrice. Ça me permet de revenir avant de repartir sur le droit d'auteur sur la première partie de votre question qui était sur la transparence pour les usagers finaux. Et donc bien vous rappelez que dans le règlement pour l'intelligence artificielle européen, l'article 50 émet des obligations de transparence. des modèles et en fonction des usages va même pour les usages au risque demander des audits préalables à la mise sur le marché des modèles d'intelligence artificielle et donc c'est un cadre ambitieux sur cette question de la transparence qui nous paraît fondamentale. sur la question du droit d'auteur peut-être donc revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure la question qui est devant nous ce n'est pas une question simple c'est de trouver un résumé suffisamment détaillé qui doit permettre à la fois aux ayants droit d'exercer leurs droits tout en maintenant le secret des affaires expliquer très clairement est une tension que nous tâchons de résoudre. Et moi je crois sincèrement au dialogue et à la consultation. Donc nous résolvons avec ma collègue Rachida Dattil à cette consultation que nous avons lancée officiellement la semaine dernière. Nous aurons l'occasion de réunir les deux écosystèmes pour créer ce dialogue et pour aboutir à une solution à laquelle, sincèrement, je crois, je pense que c'est un sujet difficile. Mais comme dans tout sujet difficile, si on prend du temps, si on écoute, si on dialogue, on trouvera une solution. Madame Robert, vous souhaitez... Oui merci de votre réponse Madame les Ministres. En fait j'ai lié la transparence à la question du droit d'auteur parce que tant que les ayants de droit ne pourront pas avoir accès à donner il ne s'agira finalement pas de reconnaître le droit d'auteur. Et la France a une responsabilité en la matière. Je pense qu'elle a une exigence. Je crois que c'est aussi l'histoire qui fait qu'à un moment, ce droit d'auteur beau marché fait partie intrinsèquement de notre histoire culturelle. Donc je crois qu'elle faut qu'elle soit exigeante et que la volonté politique soit vraiment au rendez-vous. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous souhaitiez répliquer à la réplique ? Oui, je suis alignée avec ce point. Il y a plusieurs moyens, ce que nous étudions en ce moment, que nous étudierons avec la consultation, mais je tiens aussi à rappeler que le droit d'auteur n'est pas extraterritorial et donc il faut que nous ayons des exigences des deux côtés, Madame le Sénateur Catherine de Seille le disait tout à l'heure, Morin de Seille le disait tout à l'heure. La question qui nous occupe avec l'intelligence artificielle, c'est aussi de ne pas reproduire les erreurs du passé et de ne pas tomber dans une dépendance technologique face à des acteurs extra-européens. Et donc nous voulons garder nos acteurs ici et donc trouver cet équilibre est absolument fondamental pour ce faire. Très bien. La parole est à monsieur Pierre-Jean Rochette pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci Président, Madame la Ministre et chers collègues. La course mondiale à l'intelligence artificielle ne se joue pas uniquement sur le terrain de l'innovation technologique mais aussi et peut-être surtout sur celui de l'adoption à grande échelle par les entreprises, les administrations et les citoyens. Si les États-Unis et la Chine sont en tête de la compétition en matière de recherche et de développement, de récentes analyses soulignent que la capacité à diffuser et à intégrer l'intelligence artificielle dans les usages quotidiens est un facteur tout aussi déterminant pour activer ce levier de croissance. La Chine, depuis longtemps perçue comme peu efficace en matière de mise en œuvre technologique, semble rattraper très rapidement son retard. Plus de 50% des entreprises utiliseraient déjà l'intelligence artificielle contre un tiers aux États-Unis. Il apparaît aussi et ainsi qu'en Chine, le secteur public, la consommation individuelle ou encore l'industrie manufacturière utilise désormais ces outils à grande échelle. Face à ces constats, il semble crucial de s'interroger sur les situations en France, sur la maturité de l'intelligence artificielle et de ses de ses usages dans notre société. Disposons-nous, la ministre, d'indicateurs clairs et récents permettant de mesurer l'adoption réelle de l'intelligence artificielle dans les entreprises, dont l'usage au quotidien de nos collectivités territoriales, de nos administrations, de nos concitoyens. Quels usages en font-ils ? Quelles sont les mesures de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle destinée à encourager son utilisation dans tous les pans de la société ? qui sera faite aussi à travers les logiciels qui seront proposés aux collectivités locales et notamment aux mairies où là je pense qu'on a un petit sujet de souveraineté, on doit peut-être accompagner nos collectivités locales à l'usage de cette intelligence artificielle qui peut être bien entendu un réel atout mais qui peut aussi être un gisement de données important à surveiller et devenir un sujet de souveraineté par de facto. Merci. Parce qu'on peut avoir les meilleurs labos de recherche du monde, on peut avoir les meilleures entreprises, mais si on n'utilise pas l'intelligence artificielle, alors on n'aura pas les gains de compétitivité, ni les gains pour les usagers et les agents et les employés que cette technologie permet. Donc je suis tout à fait alignée avec votre propos. Comment on fait ? Sous l'égide du premier ministre, je le rappelais pour la partie administration, avec le comité interministériel pour l'IA, nous avons demandé à chaque ministère de lister de quelle façon ils utilisent l'intelligence artificielle, quels sont les cas d'usage et comment ils peuvent passer à l'échelle et tous les ministères nous remettront ces feuilles de route intelligence artificielle au moment de Vivatec, donc dans un mois et quelques maintenant, dans lequel nous réunirons à nouveau le comité interministériel pour l'IA. Ils le font avec l'appui de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, afin de pouvoir avoir accès à un conseil technologique sur la capacité que l'on peut avoir de déployer ces solutions à l'échelle. Parce que quel usage c'est bien, mais on veut les déployer aussi à l'échelle. Pour la partie collectivité, collectivité, c'est une vraie question. Nous travaillons avec toutes les associations, France Urbaine, les Interconnectés, pour que ce travail qu'on peut faire au niveau de l'État puisse aussi bien sûr être porté au niveau des collectivités. Et ça fera partie aussi des choses sur lesquelles nous souhaitons avancer dans le cadre du plan du comité interministérieur. Pour la partie entreprise, plusieurs réponses. Suivre la diffusion de l'IA, bien sûr. On a certains sondages que je mentionnais tout à l'heure qui nous permettent de dire, par exemple, qu'aujourd'hui que 5% des PME utilisent l'IA quand c'est 35% pour les grandes entreprises. Et on s'appuie sur à la fois les CCI. On a signé avec les CCI une logique d'accompagnement qui vise à accompagner 20 000 entreprises dès cette année à l'utilisation de l'IA les plus petites et pas seulement les grandes entreprises. J'ai été la semaine dernière à un événement avec la CCI Paris. qui met en place de la formation, de l'accompagnement pour pouvoir accélérer. On a aussi un dispositif qui s'appelle IA Booster, qui est financé par l'État, qui vise à accompagner les plus petites entreprises et on travaille sur un observatoire, un portail qui permette à chaque entreprise de trouver en fonction des cas d'usage les solutions qui seront les plus pertinentes. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Chaz pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Chaz, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Beaucoup de choses ont déjà été dites, je vais essayer de ne pas faire de redites en vous posant plusieurs petites questions Madame la Ministre. Dans le contexte actuel où l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus central dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, comment pouvons-nous assurer une gouvernance efficace et éthique d'OLIA ? Quelles sont les principales problématiques à prendre en compte, telles que la transparence des algorithmes, la protection des données personnelles et la responsabilité des entreprises qui développent ces technologies ? Par ailleurs, quelles réglementations pourraient être mises en place pour minimiser les risques liés aux biais algorithmiques et à l'automatisation des décisions et comment impliquer les divers acteurs de la société, y compris les gouvernements, les entreprises et les citoyens dans ce processus de gouvernance ? Et enfin, Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits des individus ? Je vous remercie. Ça va être dur de tenir en deux minutes. Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour toutes ces questions. Nous aurons l'occasion d'en discuter autant que vous voulez après le débat avec chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Sur la question de la régulation, nous avons parlé du règlement pour l'intelligence artificielle de nombreuses fois, donc je n'y reviens pas. Sur la question de la gouvernance, ça me permet d'aborder un peu plus en détail. Au niveau français, la façon dont nous abordons la question de la gouvernance, c'est de s'appuyer à la fois sur l'Institut d'évaluation dont j'ai parlé, l'INESIA, pour nous permettre d'avoir accès à de la recherche de qualité pour comprendre l'intelligence artificielle, les modèles, comprendre les différents usages, de s'appuyer sur les citoyens avec les CAFEIA. on a lancé ce dispositif avec le Sénum, qui est la représentation structurée de ce mouvement citoyen, et avec les conseillers numériques pour pouvoir rester au plus proche du terrain, répondre aux interrogations de chacun. Et bien sûr, nous travaillons à l'implémentation du règlement pour l'intelligence artificielle, à définir quelles administrations auront en charge la mise en place de cette réglementation. Vous aurez de la visibilité là-dessus très prochainement. Sur la question internationale, parce que la gouvernance, nous pensons, doit être internationale, c'était aussi l'objet du sommet pour l'action sur l'IA. Pas seulement d'accélérer la feuille de route nationale, mais bien aussi d'impulser une dynamique internationale. Nous avons réappuyé notre soutien à ce qu'on appelle le PMIA, Partenariat Mondial pour l'Intelligence Artificielle, qui est maintenant adossé à l'OCDE et qui emporte plus de 60 pays pour définir une gouvernance mondiale. qui s'appuie sur ces centres de recherche d'expertise, donc on en a un en France, mais il y en a un aussi au Canada et un au Japon, pour pouvoir faire avancer ensemble, collectivement, de façon internationale, ces questions de gouvernance. C'est un projet qui est très important, qui a été d'ailleurs impulsé par la France en 2018 par le président de la République et par l'ancien Premier ministre Justin Trudeau, canadien, et que l'on continue bien sûr à fortement appuyer.

Ma question porte sur un enjeu de plus en plus central. Comment concilier la montée en puissance de l'intelligence artificielle avec celle du réchauffement climatique ? Nous assistons, vous le savez, depuis quelques mois à une explosion d'usage des intelligences artificielles génératives, notamment par le grand public. Qu'il s'agisse de créations d'images, de textes ou de contenus divers, la production automatisée atteint aujourd'hui des volumes impressionnants. Vous n'avez pas pu passer dernièrement à côté de ces créations numériques, ces avatars personnalisés, appelés starter packs, dont plus de 750 millions d'exemplaires ont été générés à travers le monde. Or, chaque génération d'image ou de contenu consomme de l'énergie, de l'eau, mobilise des ressources informatiques considérables et contribue à son échelle à l'empreinte carbone du numérique. Dans le cas précis d'un starter pack, c'est l'équivalent de 3 à 5 litres d'eau qui est nécessaire sans compter l'électricité consommée pour charger les appareils connectés, ni même les ressources dépensées pour, au préalable, entraîner et perfectionner l'IA. Cette frénésie d'usage pose une question, dans quelle mesure cette consommation est-elle soutenable à long terme, à un moment où notre société s'efforce de maîtriser sa consommation énergétique. Il est important d'encourager des usages responsables et prioritaires de l'IA en privilégiant son utilité concrète et en renforçant la sensibilisation aux bonnes pratiques. L'intelligence artificielle est aussi, comme vous l'avez rappelé Madame la Ministre, comme la ministre, un allié précieux dans la lutte contre le réchauffement climatique, optimisation énergétique des bâtiments, gestion intelligente des réseaux, modélisation du changement climatique, détection des pollutions. Des applications vertueuses de l'IA peuvent bien sûr être trouvées et développées. Ce constat se retrouve à la fois dans le dernier rapport du Césaire sur l'IA et dans le manifeste des intercommunalités de France sur l'IA, dans les axes stratégiques définis par le MEDEF pour le développement de l'intelligence artificielle et au cœur des sept principes de l'IA de confiance établis par le Conseil d'État dans un rapport paru en 2022. Madame la Ministre, quelles actions le gouvernement prévoit-il pour promouvoir une utilisation utile et responsable de l'IA et d'en faire un outil au service de la transition écologique ? Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour cette question et on entend bien, c'est la deuxième question sur ce sujet, l'importance qu'accordent nos citoyens à cette question et donc vous les représentez ces interrogations et c'est une bonne chose parce que je crois que ça montre ce qu'on veut dire quand on veut dire une IA à la française, une IA durable, on voit bien que c'est au coeur des préoccupations des Français. préoccupations des Français. Pour autant, je voudrais comprendre un tout petit pas de recul si possible, même si c'est une question fondamentale et qui sincèrement doit nous occuper. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça représente seulement 0,1% de la consommation. Quand des astronautes, par exemple, nous disent qu'ils ne veulent pas créer un starter pack parce que ça utilise de l'énergie, je les invite à s'interroger sur la consommation énergétique. d'un vol enfusé. Ceci étant dit, je pense que ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle c'est que bien sûr il faut prendre conscience de ses usages mais je pense que le plus gros risque c'est qu'on ait une population qui n'ose pas utiliser l'IA, qui se freine dans son adoption. parce qu'on voit bien à quel point elle va transformer tous les métiers, notre façon d'apprendre, notre façon d'interagir, d'échanger et donc il faut que l'on puisse faire de l'écologie notre allié et c'est ce qu'on peut faire en France parce qu'encore une fois on a une énergie bas carbone qui est parmi la plus compétitive du monde donc la réponse française à ce défi elle est par nature plus écologique et la réponse de l'intelligence artificielle c'est d'ailleurs que l'écologie est une amie de l'économie pour l'IA. Pourquoi ? Parce que qui dit plus petits modèles, et c'est là où on met notre recherche en ce moment, qui dit plus petits modèles dit aussi modèles plus économiques. Et donc tout le monde a à gagner si on investit non seulement pour avoir des IA qui s'entraînent ici avec notre énergie décarbonée, mais en plus des plus petits modèles qui auront un retour sur investissement plus grand pour les entreprises. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, et vous l'avez dit très justement, en plus l'IA peut nous permettre d'accélérer sur des des points fondamentaux de nos défis sur la transition écologique. J'ai rencontré des chercheurs qui ont gagné des années sur la recherche de matériaux pour remplacer le plastique. C'est ça aussi ce que permet l'IA. Et donc je crois qu'il faut qu'on trouve le juste équilibre. La prise de conscience, c'est très bien, c'est formidable, c'est ce qui fait, je pense, qu'on est très fiers d'être européens parce qu'on veut répondre à ces défis mais sans freiner l'adoption et surtout en accélérant sur la recherche de solutions. Merci Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur David Ross pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes tous convaincus que le sujet en débat ce soir, organisé à la demande de l'Opex, et je salue son Président Stéphane Piednoir, autour des enjeux de l'intelligence artificielle est essentiel pour l'avenir de notre pays, et ce à de nombreux égards. Comme l'a déjà signé le Président de l'Opex, un rapport de nos collègues Corinne Narasiguin et Patrick Chaise, je salue aussi par sa présence, avait déjà soulevé de nombreuses questions sur ce sujet. Ma collègue Sylvie Robert vous a interrogé madame la ministre concernant les questions relatives aux droits d'auteur qui inquiètent le monde culturel et mon collègue Adelzian vous questionnera quant à lui sur les enjeux de souveraineté. Je souhaitais pour ma part, compte tenu du temps de débat limité, vous interroger sur le volet formation-recherche. En effet, lors des questions d'actualité au gouvernement du 12 février dernier, j'ai interrogé la ministre d'État, Mme Elisabeth Borne, en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, quant au déploiement de l'IA dans le système éducatif français. Pourriez-vous nous informer, Madame la Ministre, quant au bilan des expérimentations au cours depuis la rentrée scolaire et les intentions ou directives opérationnelles pour la rentrée 2026 ? La création et l'usage de logiciels d'apprentissage développés et contrôlés par les autorités françaises me semble primordial afin d'assurer une formation adaptée à une volonté à terme d'une souveraineté nationale. De plus, Madame la Ministre, avez-vous d'autres ambitions qui pourraient être impulsées sur le temps scolaire, mais également qui pourraient être impulsées sur le temps hors scolaire ? Et de manière plus générale, Madame la Ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait essentiel de favoriser l'émergence de pôles de formation, de recherche et de développement, en particulier à proximité et en relation avec des centres de données numériques, afin de participer pleinement à une souveraineté numérique pour les générations à venir Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour cette question sur l'éducation qui est, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment fondamentale si on veut favoriser l'accessibilité de l'intelligence artificielle, ne pas créer cette fracture numérique et surtout créer un esprit critique de nos jeunes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. La question de la diffusion via l'éducation est absolument fondamentale. Deux ans, l'Education nationale a lancé un AMI qui, pour les usages, pour les outils d'intelligence artificielle destinés aux jeunes, a rassemblé un certain nombre de solutions. C'est par exemple une entreprise comme Nolège que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a d'ailleurs eu un prix, qui a été élu meilleur start-up des techs mondial parmi plus de 7000 candidats. et qui permet de transformer les supports de cours pour les rendre plus ludiques et donc de créer un intérêt accru pour les élèves. Donc on a recensé toutes ces solutions, on a fait l'éducation nationale, madame la ministre Elisabeth Borne a fait le bilan de ses premiers usages, c'est un bilan qui a été jugé très positif et c'est pourquoi le ministère de l'éducation nationale lancera à l'été sur le même système un AMI pour les professeurs, pour pouvoir aussi recenser les meilleures solutions solutions pour équiper les professeurs d'intelligence artificielle et les aider à adapter leurs cours et leurs méthodes pédagogiques pour les élèves afin d'être prêt dès la rentrée 2025, comme cela a été annoncé par madame la ministre Elisabeth Borne, que les élèves de quatrième et de seconde aient accès à des cours dès cette rentrée sur cette intelligence artificielle. Merci madame la ministre. Monsieur Ross, vous avez quelques secondes. Merci Madame la Ministre pour votre réponse qui rejoint un grand nombre de préoccupations qui sont d'ailleurs dans le cadre d'une PPL que je déposais. J'espère qu'on aura l'occasion dans cet hémicycle d'aller plus en avant sur ces sujets-là et à la fin d'assurer à notre pays une souveraineté numérique, une véritable IA, une indépendance assumée. Merci Madame la Ministre. Vous souhaitez compléter ? Je passe la parole à Madame Marie-Claire Carrégé pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sauf à courir le risque de dégâts potentiellement irréversibles, des décisions sur l'IA générative s'imposent à très court terme avant même l'entrée en vigueur du règlement européen. Des risques pour la démocratie et la confiance des rapports sociaux d'abord. Des images produites sur l'IA sont diffusées et reprises des milliers, voire des millions de fois sur les réseaux sociaux, le plus souvent depuis des comptes anonymes, dans un but de manipulation des esprits. Quantité de faux documents circule aussi avec une explosion des tromperies, par exemple à l'embauche avec de faux diplômes et de fausses preuves d'expérience, et aussi une fraude massive aux assurances avec des sinistres fictifs. L'article 50 de la IA qui imposera aux fournisseurs de systèmes d'IA que les contenus soient, je cite, marqués dans un format lisible par une machine et identifiable, mais identifiable par qui, comme ayant été généré par une IA. J'aimerais Madame la Ministre qu'il soit absolument clair que les fournisseurs d'IA et le modèle d'IA usage général doivent, devront systématiquement, systématiquement apposer un marquage général dans un coin des images et documents, une sorte de logo immédiatement visible par des yeux humains et non pas seulement par des machines. Il faudra aussi que le plus tôt possible les plateformes et réseaux sociaux se mettent en situation de détecter et d'afficher l'origine IA des publications. LinkedIn a récemment annoncé vouloir aller dans cette voie, il convient de tous les encourager à le faire. L'autre risque majeur concerne la santé avec la diffusion actuellement très rapide d'outils d'IA extra-européens permettant d'effectuer la synthèse de consultation médicale et de produire un récapitulatif du dossier médical. Ils ne respectent aucunement l'obligation d'un contrôle humain régulier par un professionnel de santé français. Ils peuvent permettre une exfiltration rapide de nos données de santé hors d'Europe et induire la perte de contrôle sur l'avenir de notre système de santé. Là aussi, quelles décisions comptez-vous prendre, Madame la Ministre, sans attendre l'entrée en vigueur de toutes les dispositions du Règlement sur l'IA pour faire respecter de strictes conditions de souveraineté et de contrôle humain ? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.

Vous avez raison, nous avons décidé en Européen, avec le règlement pour l'intelligence artificielle, avec l'article 50, d'exiger des obligations de transparence des contenus qui sont générés par l'IA. À l'époque, la France a activement soutenu le fait de pouvoir inclure ces mesures dans l'article 50 et aujourd'hui nous suivons avec attention l'élaboration des lignes directrices de certains articles 50 parce qu'à l'époque du RIA, les solutions techniques de marquage n'étaient pas encore complètement définies et donc il a fallu laisser libre à pouvoir évoluer la réglementation avec l'évolution de la technologie. On a fait le choix en Europe de se doter d'un cadre réglementaire au départ de la diffusion massive de cette technologie et donc il faut que ce cadre soit adapté. J'ai rencontré un certain nombre de solutions jusqu'aux Etats-Unis. Adobe travaille par exemple sur une solution sur cette question-là, mais quoi qu'il en soit, dans ces lignes directrices, il y aura bien la question de la mise en application de cette obligation de l'article 50 qui est absolument fondamentale pour créer de la confiance autour de l'utilisation de cette technologie. Pour autant, à mon sens, le marquage et la question de quel marquage sera défini bientôt, vous l'aurez compris, Mais le marquage ne suffit pas, il faut aussi qu'on se donne de capacités de détection pour anticiper. C'est ce qu'on fait avec le Péren, le pôle qui existe rattaché à trois ministères, qui est un appui à la régulation du numérique, qui nous permet avec des expertises techniques développées par l'État de pouvoir créer des modèles de détection. Ils m'ont montré l'état d'avancement de leurs travaux qui seront absolument fondamentaux pour pouvoir appuyer d'un côté le marquage et de l'autre la détection et donc créer cette confiance. Sur la question de la santé, je vois que j'ai plus que quelques secondes, mais la question que vous mentionnez fait finalement le lien avec le RGPD, au-delà même du RIA et la protection des données personnelles. Avec le ministère de la Santé, je tâcherai de pouvoir rentrer plus précisément dans l'objet que vous avez mentionné pour apporter des réponses précises. Mais oui, dans le RGPD, les cas que vous aurez mentionné ne sont pas autorisés et donc on y sera vigilants. Dans les processus d'innovation, il y a toujours des entreprises qui mordent un peu sur la ligne, mais on a une réglementation très claire sur la protection des données et sur l'intelligence artificielle et elle sera respectée. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Adel Zian pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme cela a été rappelé, les promesses, tout comme les risques de l'intelligence artificielle, sont immenses. Pour ma part, je souhaitais, comme l'a évoqué mon collègue David Rost, vous alerter sur le danger de notre décrochage En effet, dans cette course mondiale à l'intelligence artificielle, la France et l'Europe prennent du retard. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national numérique par la voix de son président, Gilles Babinet, qui parle, je cite, d'un déclassement en cours absolument certain. Face aux colosses américains comme OpenAI, Microsoft ou Google et aux ambitions fortes de la Chine, notre continent n'a à l'heure actuelle ni la puissance de frappe financière ni la stratégie industrielle cohérente pour peser. J'en veux pour preuve par exemple l'avance américaine et l'annonce du projet Stargate par la Maison-Blanche dotée de 500 milliards de dollars qui devrait nous alerter. Pourtant, en France, notre recherche publique continue de manquer de moyens et de nombreux talents encore, malgré tout, partent faire carrière dans les labos de la Silicon Valley. Alors oui, Madame la Ministre, les 109 milliards d'euros d'investissements annoncés en France sont à saluer, mais ce plan reste fragmenté, sans vision européenne coordonnée face aux empires industriels américains et chinois. L'Europe a mieux en effet, il faut le souligner, un cadre de régulation. Mais ce cadre doit maintenant s'accompagner d'une véritable ambition industrielle. Sans cela, nous resterons les consommateurs des technologies des autres. Nous ne sommes qu'au commencement d'une révolution technologique comparable à celle de l'électricité ou d'Internet. Et l'IA est amené à bouleverser notre économie, notre manière de produire, de soigner, d'apprendre. C'est donc avant tout, et j'insiste là-dessus, un enjeu de souveraineté, de démocratie, de civilisation. Si une IA souveraine peut poser des défis, ils ont été évoqués précédemment par mes collègues, éthique, politique, environnementaux, elle reste toutefois à porter de débats démocratiques, de régulation publique et de contrôle citoyen. Là où, à l'inverse, une IA conçue ailleurs, et on le voit avec les GAFAM, selon d'autres intérêts, s'impose à nous. De fait, notre dépendance technologique n'annonce pas un simple retard, mais une dépossession politique sur laquelle je voulais vous alerter. Alors Madame la Ministre, quelle stratégie de rupture la France, avec ses partenaires européens, compte-elle adopter pour sortir de cette dépendance, et en somme à quand, un véritable airbus de l'intelligence artificielle capable de structurer une ambition collective souveraine et durable ? Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que ça fait un moment qu'on est dans l'hémicycle et la question de la compétitivité et finalement de la réponse à l'enjeu de cette course dans l'IA n'avait pas été encore posée. Je pense que c'est bien ce qui doit nous occuper avant tout. Parce que toutes les autres questions auxquelles on a tâché de répondre et qui ont existé de la discussion jusqu'ici ne peuvent exister que si on a une réponse européenne, si on a une IA européenne. la seule solution pour pouvoir avoir une IA qui est fidèle à nos valeurs, pour pouvoir avoir une IA qui est plus frugale, pour pouvoir avoir une IA qui est à disposition des jeunes pour l'éducation. Et donc c'est bien ça, je crois, qui doit nous occuper plus que jamais. Là où je vous rejoins pas tout à fait, c'est que je pense pas qu'on soit dans cette situation de décrochage, preuve en est les différents index qui nous placent entre la troisième et la quatrième position au niveau mondial. Et sur les différents pans que vous avez mentionnés et que je reprends, le projet Stargate américain était très conséquent, 500 milliards d'euros. Pour autant, le projet que nous avons annoncé lors du sommet pour l'action sur l'IA, les 109 milliards d'euros sont peu ou prou, le même ordre de grandeur ramené à la population française, donc il n'y a pas à rougir il n'y a pas qui est mis en France en termes d'infrastructure qui est un des piliers de la stratégie de l'IA. Concernant la recherche, je l'ai mentionné tout à l'heure mais c'est un de nos atouts les plus fondamentaux. C'est pourquoi on a décidé de réinvestir dans la recherche avec les clusters IA partout sur le territoire. Neuf clusters, 360 millions d'euros qui visent à former 100 000 personnes par an d'ici 2030 et on fera toujours de cette recherche une priorité de notre action. Et concernant l'Europe, vous avez parlé de la réponse peut-être un peu décoordonnée européenne. Là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où lors du sommet pour l'action sur l'IA, ça a aussi été l'occasion pour l'Europe de rappeler sa stratégie InvestEI, 200 milliards d'euros sur toute la chaîne de valeurs des Gigafactory, à la diffusion de l'IA dans l'industrie. l'Europe a dévoilé il y a maintenant deux semaines le plan AI continent dans lequel on va consulter un certain nombre d'acteurs pour voir comment est-ce qu'on peut mieux se coordonner au niveau européen sur ces giga-projets. Mais il y a des moyens, il y a une vision, il y a une ambition d'innovation et pas seulement de régulation. Merci Anna la ministre. est à monsieur Christian Brien pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'intelligence artificielle elle alimente des angoisses irrationnelles autant que des attentes démesurées. Cette technologie nous semble à la fois omniprésente et insaisissable et alors que sa diffusion n'est encore que très très relative. Bref, l'IA est un phénomène d'une telle puissance qu'il nécessite donc au plus vite de se préoccuper de la formation de l'esprit critique de ces utilisateurs. Plus et mieux on comprendra le fonctionnement de ces solutions et moins on les subira. Et d'évident cela doit débuter à l'école, au collège, au lycée et c'est pourquoi mon propos porte sur l'enseignement scolaire. Nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté gouvernementale de définir une stratégie ambitieuse pour l'IA dans l'éducation. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous exposer quelques priorités, points essentiels de la dite stratégie, voire nous indiquer des échéances prévisionnelles de cette démarche ? Merci M. le Sénateur. J'ai eu l'occasion de rappeler que lors du comité interministériel sur l'IA présidé par le Premier ministre, chaque ministère a pu s'engager dans cette démarche de diffusion de l'IA dans son propre ministère. Madame Elisabeth Borne, ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé ses grandes orientations. Je la laisserai peut-être échanger plus en détail avec vous sur cette question si nécessaire, mais les grandes décisions qui ont été prises, c'est déjà de pouvoir, déjà d'ailleurs depuis deux ans, expérimenter avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ces solutions peuvent nous apporter pour faire plus de personnalisation dans la démarche d'éducation. C'est l'AMI dont j'ai parlé tout à l'heure qui a recensé un certain nombre de solutions. que l'on doit maintenant porter et que l'on porte dès cet été au niveau des professeurs donc s'assurer qu'on ne crée pas entre les professeurs et les élèves des élèves qui eux utiliseraient l'IA et des professeurs qui seraient plus en difficulté. J'étais la semaine dernière à Quimper dans un lycée et les professeurs utilisaient l'IA dans un bac pro service et restauration et un des professeurs on le sentait était beaucoup plus en retrait que l'autre donc on veut remédier à ça et mettre des outils dans les mains de tous les professeurs. Et puis la question de savoir comment l'IA, au-delà de l'Éducation nationale, s'inscrit dans toutes les formations. Mon collègue Philippe Battiste est aussi bien sûr en réflexion pour voir dans l'enseignement supérieur comment l'IA va pouvoir insuffler toutes les formations. Merci, M. Brouillard. Merci Madame la Ministre. Comme vous, le ministère de l'Education nationale évoque à juste titre, vous l'avez fait, l'indispensable préservation de la notion de souveraineté, de même qu'est primordial l'application de principes de précaution, plus encore pour ce qui touche à la jeunesse. Mais il convient tout de même de ne pas mettre en place toute une série de garde-fous qui seraient pour beaucoup illusoires, mais viendraient scléroser le développement de cette technologie et de ces applications. Il est évoqué dans la présentation de stratégie par Madame la Ministre de l'Education nationale des outils à même d'aider les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Très bien, mais il faut le dire, il existe déjà de nombreux outils de qualité, d'ailleurs promus par le ministère de l'Education nationale, mais ils sont malheureusement sous-exploités. Vraiment, il est donc surtout à mon sens nécessaire d'accompagner le corps enseignant pour que s'engage une véritable appropriation de ces outils. Disons-le, les usages de l'IA dans le système éducatif sont parfois trop normés pour offrir des possibilités de pédagogie différenciée adaptées aux capacités de l'apprenant. C'est bien dommage, car c'est d'abord en mieux valorisant l'IA auprès de ses personnels enseignants que l'éducation nationale favorisera l'émergence d'une vraie culture citoyenne de ce phénomène, et c'est fondamental. Merci Merci madame la ministre. Tout à fait, c'est la démarche qui est la nôtre qui est très importante, vous l'avez justement souligné et je dois dire d'ailleurs qu'il doit aussi se permettre de soutenir notre secteur edtech, donc de technologie éducative sur lequel on a beaucoup de solutions très performantes, j'en citais une tout à l'heure qui a gagné un grand prix international et donc permettre de mettre ces solutions dans les mains des enseignants et des élèves, c'est tout à fait la stratégie que l'on s'emploie à décliner. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains. sujet de zéro artificialisation nette qui nous anime beaucoup dans cet hémicycle. Et un jour, il faudra vous interroger d'ailleurs sur IA et sols vivants. Autrement dit, comment pourrons-nous avoir un jour prochain de meilleure connaissance de notre sol et de notre sous-sol ? Je voulais vous interroger là-dessus. Dans le cadre de l'analyse de masse des données photosatélitaires compilées pour nourrir l'outil OCSGE, L'institut national de l'information géographique et forestière a donc recours à l'intelligence artificielle. Cependant, à l'heure actuelle, les performances de cet outil apparaissent comme encore largement perfectibles. y a but en effet sur certaines interprétations données qui dépendent aussi de la qualité des intrants numériques impliquant nécessairement des contrôles et vérifications des opérateurs humains. Il est également possible de signaler directement des erreurs d'interprétation dans une logique de participation, d'utilisation à l'amélioration de la qualité de la donnée. Et là, je sors de ma question écrite pour vous dire qu'il y a des conflits dans les territoires entre l'Etat et les collectivités sur ce qui a été réellement artificialisé. On n'a pas les mêmes chiffres. Donc, si vous voulez, il y a non seulement la construction du sujet, mais la gouvernance et le partage de la donnée. Donc, dès lors, quelles sont pour vous les perspectives d'amélioration de cette utilisation de l'IA par l'IGN ? On pourrait parler du CEREMA aussi, bien entendu. Quel gain peut-on espérer en termes de mise à jour des millésimes, des séries de données et comment s'assurer de la fiabilité de ces données ? Un référentiel partagé avec d'autres pays pour permettre des analyses comparatives intéressantes sur le rythme et la géographie. De l'artificialisation est une piste ? Est-ce qu'elle peut être envisagée ? On aurait aimé vous entendre sur tous ces sujets. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour cette question. C'est tout à fait un exemple d'à quel point l'IA peut apporter aussi des solutions aux enjeux écologiques qui étaient mentionnés tout à l'heure. Et donc c'est bien sûr un sujet très pertinent sur lequel on sait que la puissance de l'intelligence artificielle peut nous aider à modéliser, à comprendre, à répondre aux interrogations que vous avez soulevées. l'IGN et l'IGF font un travail déjà très important sur cette question. Ils sont à la pointe de l'utilisation de l'IA, ils développent un certain nombre de choses, il y a des limitations mais il y a quand même un effort et une volonté d'aller plus loin. Dans le cadre de France 2030, on a engagé un un plan de ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Donc on regardera plus précisément si dans le cadre de ce plan, l'IGN pourrait bénéficier d'une aide et d'un appui pour pouvoir avancer plus vite et d'être encore plus performant sur cette question parce qu'il y a des cas d'usage qui peuvent nous permettre de résoudre un certain nombre de questions importantes. Merci monsieur Blanc. Merci madame la ministre. Simplement un point d'alerte sur la gouvernance de ce sujet. C'est à dire que les élus ne n'aient pas l'impression que ce soit imposé, que ça tombe d'en haut. Parce que sur le ZAN, c'est ça le problème. La planification est mal vécue. Donc faisons-le ensemble. La parole est à madame Anne Vintalon pour le groupe Les Républicains. L'Académie de médecine a récemment rendu un rapport sur l'IA générative qui estime que son déploiement pourrait avoir un impact très positif pour aider les médecins dans leurs pratiques quotidiennes. Lié en santé est ainsi considéré comme un outil supplémentaire capable d'apporter beaucoup à plusieurs niveaux. Améliorer la qualité des soins, le suivi des patients, gagner du temps médical, optimiser les diagnostics, réorganiser notre système de santé. Les avantages sont multiples pour les soignants comme pour les patients. Alors l'IA pourrait-elle être une opportunité pour lutter contre les déserts médicaux ? Des solutions numériques peuvent apporter une réponse partielle à cette problématique. Installés depuis quelques années, les cabines de télémédecine en sont une parfaite illustration. L'IA peut améliorer les performances en téléconsultation en interprétant en direct des données captées dans ses cabines ou en guidant l'entretien avec le patient. Elle est potentiellement un outil de meilleure organisation du processus de soins et de réduction des inégalités territoriales de santé. Néanmoins, l'IA ne résout pas à elle seule la question de l'accès aux soins. Elle ne remplace ni la main du médecin, ni la parole rassurante du soignant, mais permet de les soulager dans leurs tâches répétitives et administratives. Dans le secteur de la santé, l'IA est encore en phase d'apprentissage avec un foisonnement d'initiatives autour d'équipes médicales. motivés et d'entreprises innovantes. Aussi madame la ministre, comment tendez-vous à accompagner leurs actions afin que notre système de santé ne rate pas le virage de l'IA et tire le maximum de bénéfices de cette technologie ? Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, je vous remercie pour cette question. En effet, je pense que la santé, c'est le domaine où les bénéfices de l'IA sont les plus clairs et les plus compréhensibles par toutes et tous. Et les avancées sont absolument fulgurantes. Et cela doit nous permettre de répondre à un certain nombre de défis. C'est pourquoi on a un certain nombre de projets portés par le Health Data Hub, notamment le projet Partage, qui s'inscrit dans ce contexte-là de mettre à disposition l'IAGénérative pour l'analyse des données de santé et permettre d'accélérer la recherche sur un certain nombre de cas précis. Et c'est bien sûr un projet que le ministre de la Santé est très attaché à continuer à appuyer pour développer nos propres LLAM, nos propres bases de données qui permettront de résoudre un certain nombre de défis très importants pour la santé de nos concitoyens. Sur la question de la télémédecine, aujourd'hui, chaque hôpital travaille en fonction de ses spécialités à nouer un certain nombre de partenariats pour pouvoir résoudre la problématique que vous avez citée de la disponibilité des soignants partout sur le territoire et pouvoir avoir en fonction du plan qui est le leur mettre à disposition des personnes qui doivent être soignées, des experts grâce à ces partenariats et l'utilisation de l'IA en effet pour digitaliser l'expérience de soins et donc répondre à une partie de la problématique soulevée. C'est quelque chose que l'on voit notamment à l'Institut Gustave Roussi qui a été déployé déjà maintenant depuis quelques temps et qui je crois porte ses fruits. Merci Madame la Ministre. Mme Ventallon, vous avez disponible une poignée de secondes. Oui, remercie Madame la Ministre et rappelez que le fonctionnement de l'IA doit être compris pour être mieux appréhendé, en tirer profit, mais aussi pour mesurer ses limites. Donc la formation initiale et continue soignants me paraît essentielle. Merci. Merci. Nous sommes parvenus au terme de ce débat. Pour en tirer les conclusions, je donne la parole à Mme Christine Lavarde, présidente de la délégation sénatariale à La Prospective. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle cristallise tous les défis du XXIe siècle, donc je ne vais pas reprendre ici les nombreux défis qui ont été évoqués par les uns et les autres, mais peut-être tirer cinq leçons, cinq grandes idées de ce débat et aussi des travaux qui ont nourri les les travaux de l'Opex et les travaux de la délégation à la prospective pendant presque 18 mois. Et le premier de ces constats est l'évolution extrêmement rapide. En 18 mois, nous avons pu voir comment les technologies, les innovations, les solutions proposées par l'intelligence artificielle étaient différentes et comment chaque mois qui passe, et promet des solutions toujours plus complètes. Et ces évolutions très rapides, elles nous obligent, nous en tant qu'État, en tant que puissance forte, à poursuivre nos travaux de recherche, à investir pour ne pas se laisser dévalorisées par rapport à des puissances qui elles sont très fort mais je pense ici aux Etats-Unis et aux GAFAM et aussi demain aux Chinois qui disposent d'entreprises très fortes dans ce domaine. Ces évolutions rapides elles nous obligent aussi à être agiles et je pense et vous l'avez dit et c'est le constat que nous en tirons que les conclusions doivent toujours être fondées sur l'expérimentation sur des épreuves tirées du concept tirée de l'expérience et nous avons pu voir comment par exemple la direction générale des finances publiques qui a développé les premiers outils peut être force d'exemple ensuite pour développer d'autres outils par exemple dans le domaine de la fraude. Autre sujet d'importance dès qu'on parle d'intelligence artificielle est celui de la question des données. Les données sont au coeur de l'intelligence artificielle et elles ne doivent pas demain, et ça a été dit par de très nombreux orateurs ici, être captées par des GAFAM ou par d'autres pays. C'est pourquoi nous avons besoin de développer des solutions souveraines, c'est pourquoi nous devons agir collectivement pour disposer d'un cloud européen et demain nos données de santé ne devront pas pouvoir être être hébergées par des acteurs non européens. Ces données doivent aussi être structurées si nous voulons qu'elles puissent avoir un rôle moteur, le moteur, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Et malheureusement, je dois faire le constat qu'à l'issue de nos travaux, nous constatons encore aujourd'hui un très fort un très fort manque d'interconnexion des systèmes d'information. Et ça a été dit aussi quand on a parlé du créole. Si le système d'intelligence artificielle marche, ils ont besoin de pouvoir se nourrir de données. Et aujourd'hui, on voit bien pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle nous répond avec avec du franglais. C'est parce qu'elle a lu majoritairement soit du mauvais français, soit en tout cas du français traduit de l'anglais. Et c'est pour ça que certains pays, par exemple le Japon, aujourd'hui n'arrivent pas à aller très loin, à être moteur, parce qu'en fait le Japonais n'est pas parlé beaucoup à travers le monde. Donc cette question des données elle est extrêmement importante et elle est importante aussi parce qu'avec la politique des données ouvertes elle vient remettre en cause un certain nombre de principes économiques et aujourd'hui nous avons certains des acteurs nationaux qui ont vu leur modèle économique complètement remis en cause parce que politique de données ouvertes et je pense aussi à des agents soit des opérateurs de l'état ils ne peuvent plus vendre donc ils ne peuvent plus tirer de recettes économiques ce qui fragilise l'ensemble des politiques publiques qu'ils pouvaient mener Et on a évoqué très largement cet après-midi ici la question du droit d'auteur, des droits voisins. Ce sont des sujets que nous devons traiter si demain nous voulons pouvoir continuer ce processus un peu de création qui s'auto-alimente. Et on doit aussi poser la question à l'inverse. Est-ce que demain certaines entreprises privées qui disposent de données d'intérêt national devraient pas aussi les mettre à disposition de la puissance publique dans l'idée de développer le bien commun. Je vois le temps qui passe et je sais pas si je vais pouvoir tout développer mais il y a aussi la question du développement des compétences. Vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, elle procède d'une redistribution profonde des pouvoirs. Je suis complètement d'accord avec vous et si on veut que l'Etat puisse continuer à avoir ce rôle d'Etat stratège, il faut qu'il ait les capacités de pouvoir recruter des profils spécialisés, il faut qu'il puisse puisse faire monter en compétence les agents publics et je pense ici aux agents de l'Etat mais aussi aux agents des collectivités. Et derrière tout ça, il faut aussi pouvoir repenser le travail et ça c'est des choses que nous avons pu voir au cours de nos déplacements ou au cours de nos auditions. Christian Bruyan l'a très bien dit, au-delà des compétences des agents publics, il y a aussi la question du grand public. Comment pouvoir embarquer avec nous les citoyens dans cette appropriation de l'intelligence artificielle ? Il est très important d'avoir une acculturation, de démystifier et en même temps d'informer sur les dangers et les opportunités de cette technologie. Et aujourd'hui, on l'a vu, pour nous, premier pas à faire c'est bien celui de l'enseignement de l'éducation nationale où aujourd'hui les enseignants sont finalement dans une situation de faiblesse par rapport à leurs élèves qui eux pour certains sont nés avec ces outils d'intelligence artificielle et c'est très important parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle pour pouvoir se développer elle a besoin d'être dans un climat de confiance et nous avons parlé aussi cet après midi du cadre éthique et juste parce que j'ai déjà dépassé le temps et que le Président est très bienveillant, mais j'avais peut-être deux mots de conclusion à dire pour que l'intelligence artificielle puisse se développer. On l'a dit, elle doit être proportionnée, c'est-à-dire que la question de la frugalité est extrêmement importante, et Ghislaine Séné et Ludovic Hayes sont bien revenus sur cette question. Effectivement, liberté mais frugalité, il faut informer les uns et les autres sur sur le coût. Il y avait un livre très intéressant qui s'appelait « L'enfer numérique », et aujourd'hui tout le monde envoie des émaux icônes, mais on oublie le coût numérique de l'envoi de ces émaux icônes. et surtout l'intelligence artificielle. Pour être utile, elle doit démontrer sa pertinence et donc sa valeur ajoutée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de coût à ouvrir un dictionnaire pour sortir une définition plutôt qu'à utiliser l'intelligence artificielle. Vous avez épuisé ma bienveillance, chers collègues. Merci. Je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème comment relancer le frais de ferroviaire. Je vous rappelle que dans la demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaqui. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes, Monsieur le Ministre. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie pour une minute. Monsieur le Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, vous les connaissez bien, une fois que chacun d'entre eux aura retrouvé sa place dans l'hémicycle. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, monsieur Alexandre Masquin, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe CRCEK a considéré opportun qu'un échange puisse avoir lieu sur cette question fondamentale de l'avenir du frais de ferroviaire. Celui-ci porte en effet des enjeux forts en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de sécurité, mais aussi de développement économique. Or, la part modale de marchandises transportée par le rail n'est que de 10%. Aujourd'hui, nous le voyons bien, l'enjeu est donc de taille. Rappelons que c'est en 1823 que la première concession de chemin de fer pour le transport de marchandises est accordée en France. La part du fret ferroviaire augmente ensuite, pas à pas, avec l'extension du réseau sur l'ensemble du territoire national atteignant 73% de la part modale en 1948. Un vrai maillage territorial organisé, optimisé, efficace existait alors. Il y a eu ensuite, et notamment depuis les années 70, une conjonction d'éléments comme de choix politiques qui ont malheureusement amené fortement la capacité du rail au profit du tout routier. Les logiques de rentabilité court-termiste l'ont ainsi et malheureusement emporté. Le trafic routier ne cesse de progresser quand dans le même temps, Le réseau ferré n'est plus aussi bien entretenu, les investissements ne sont plus au rendez-vous, les lignes se délabrent et les installations en branché sont fermées et nous le payons encore aujourd'hui. Le tonnage transporté décline de 75 milliards de tonnes kilomètres en 1974 à 55 en 1998 et 40 en 2005. En 2021, ce chiffre chute à 35 milliards de tonnes kilomètres. La part modale du frais de Ferroviaire est de 10% en France, je l'ai dit, contre 18% en Allemagne, 32% en Autriche, 35% en Suisse, pour ne citer que quelques exemples. Alors que le transport routier, quant à lui, représente encore 87% du transport de marchandises. Ces dernières décennies, le service public de transport de marchandises a été régulièrement attaqué. Plan d'économie massif, démantèlement du groupe SNCF, ouverture à la concurrence, fermeture de gares de triage et de lignes de fret, abandon des raccordements d'entreprises au réseau, suppression de postes, ce sont 10 000 emplois qui ont été supprimés en 10 ans. La libéralisation de la politique européenne des transports dès les années 90, avec une dérégalation massive du transport routier de marchandises, a sacrifié purement et simplement le rail. A cela s'ajoute le pacte ferroviaire de 2018 qui fragmente le service public du rail ou le plan de discontinuité qui fragilise le transport public de marchandises et sur lequel l'inter-syndical demande si légitimement un moratoire. Pour autant, aujourd'hui, Beaucoup s'accordent sur le développement du fret ferroviaire. La Convention citoyenne pour le climat de 2020 proposait le doublement de la part modale du fret d'ici à 2030. L'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 plaide également et fortement pour le développement du fret ferroviaire. À l'heure où les questions de dérèglement climatique imposent de prendre des mesures fortes, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de transport audacieuse. Parlons clair. Investir dans le fret qui est le transport le moins polluant et de loin n'apparaît pas illusoire. Bien au contraire, un train, ce sont 50 camions en moins sur les routes. Choisir d'utiliser le rail permet le développement du tissu économique, qu'il soit agricole, industriel ou logistique, avec l'implantation d'activités mieux réparties sur l'ensemble du territoire national. Il permet de désenclaver certains territoires tout en les redynamisant par une activité pérenne. Je pense à la gare de triage de Sommin dans le nord, pas loin de chez moi, dont l'activité se fait en pointillée, alors même que le potentiel est là. Les cheminots sont mobilisés, les élus locaux sont au rendez-vous et la population est particulièrement attachée à ce site. La gare de triage de Sommin demande ainsi être revitalisée plutôt qu'abandonnée. D'autant plus lorsqu'on sait que le canal Seynor passera à quelques encablures, que l'ancienne base aérienne de Cambrai se développe et que le Dakarquois va accueillir prochainement de nouvelles activités de grande ampleur. Permettez-moi une parenthèse quand je parle de Dunkerquois pour avoir une pensée. Pour ces 600 salariés d'ArcelorMittal, dont 181 à Dunkerque, dont le poste risque d'être supprimé d'un trait de plume sans aucune considération, toutes ont de but. Cette entreprise qui a obtenu 300 millions d'euros d'aide de l'État en 2023, cette entreprise qui verse 300 à 400 millions d'euros de dividendes chaque année, je pense si nécessaire que nous soyons mobilisés sur cette question majeure. Je ferme la parenthèse. La relance du fret ne passera que par des investissements conséquents, bien loin des politiques d'austérité de ces dernières années. Une loi pluriannuelle de financement des infrastructures s'avère être un enjeu crucial. Il faut rénover et densifier le réseau. Il faut rendre le rail beaucoup plus attractif, plus performant que le transport routier, qui lui bénéficie d'avantages fiscaux, qui lui bénéficie d'aides financières disproportionnées et de l'absence de contribution au financement du réseau routier par les transporteurs, contrairement aux opérateurs aux opérateurs ferroviaires. Il faut également convaincre les industriels par une fiscalité environnementale favorisant le report modal de la route vers le rail. Comme il est essentiel et urgent de repenser le modèle de financement des transports, la Conférence nationale sur le financement des mobilités, ambition France Transport, lancée en mai prochain, devra concrétiser cet objectif. En matière de financement, plusieurs pistes pourraient être explorées. Il y en a une que nous soumettons au débat et à la réflexion et je pense qu'elle pourrait nous réunir, celle du fléchage des produits des concessions autoroutières en soutien aux frettes. Rappelons que les sociétés d'autoroute ont récolté 40 milliards d'euros de plus que ce qui était prévu et on parle même de surentabilité. Ces chiffres ont d'ailleurs interpellé sur l'ensemble de ces bancs et il y a eu en 2020 une commission d'enquête sénatoriale sur ce sujet. Il n'apparaît donc pas chimérique qu'une partie de ces bénéfices puissent être affectés au développement du rail. Enfin, permettez-moi, avant de conclure, de saluer très chaleureusement les cheminots, eux qui sont bien trop souvent caricaturés. Je veux rappeler ici leur engagement sincère. désintéressés au service de l'intérêt général, au service des usagers et de la sécurité. Vous l'aurez compris, nous soutenons avec force le développement du fret ferroviaire que nous considérons être un enjeu stratégique et structurant. Il peut et doit jouer un rôle majeur et être un atout essentiel pour l'ambitieuse et nécessaire relance industrielle et agricole de notre pays pour aujourd'hui et pour demain. Il n'y a pas 100 000 solutions. Il faut surtout changer de paradigme, investir, donner du sens à la politique du fret et en faire enfin, monsieur le ministre, un bien commun national. Pour ce faire, la balle est entre vos mains. Je vous remercie. Merci. Avant la balle, la parole à monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président Mandeli, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord Monsieur le Sénateur de vous remercier pour l'organisation de ce débat, remercier votre groupe, c'est pour moi l'occasion de venir au Sénat et vous savez que c'est un... c'est toujours un plaisir que de revenir dans cette magnifique assemblée et puis c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur puisque nous avons eu l'occasion pendant des années d'en discuter dans notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Moi ce que je souhaiterais très brièvement vous dire pour répondre à votre propos et on aura l'occasion de le faire probablement à travers les les différentes questions questions qui seront posées par nos collègues. Vous avez évoqué le sujet de l'ouverture à la concurrence. Moi j'aimerais rappeler que ce secteur du fret ferroviaire a été ouvert à la concurrence, vous l'avez dit en 2006, en application des textes européens. Vous citez l'Allemagne en exemple sur ce sujet. Je vous rappelle que l'Allemagne est également ouverte à la concurrence. Donc vous voyez qu'on peut réussir en fret ferroviaire tout en étant ouvert à la concurrence. plus que l'idée du difficulté du fret ferroviaire depuis plusieurs années, l'idée de l'ouverture à la concurrence, je pense que c'est plutôt l'abandon, vous l'avez dit, du fret pendant plusieurs décennies au profit de la route et du transport de voyageurs. Je fais ce même constat et plusieurs crises marquantes ont accéléré cette des industrialisations également à la fin des années 2000 parce que c'est intimement également lié aux difficultés industrielles dans notre pays. Je rappelle que la part modale du frais de ferroviaire a symétriquement connu le même déclin que la part de l'industrie dans l'économie française. Ces 20 dernières années, vous remarquerez les corrélations entre ces deux trajectoires. La part de l'industrie dans notre économie est passée de 16,2% en 1995 à 10,1% en 2017. par la même occasion, la part modale du frais de ferroviaire de 16,8% en 1995 à 10,8% en 2017. C'est intimement lié. Je compléterai mon propos tout à l'heure, monsieur le Président, si vous me permettez.

social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je veux remercier nos collègues communistes pour ce débat, qui arrive après la publication à Mars, la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, dénommée Ulysse fret. Espérons que sous ce titre enchanteur, nous retrouvions le chemin du rail, car pour le moment, c'est entre Sharid et Silla que ce secteur se débat. Nous le savons, le transport de fret ferroviaire est au plus bas. Les chiffres confirment que l'activité est en berne quand le transport routier se taille la part de Lyon, à près de 90% des tonnes kilomètres. Pour le fret ferroviaire, nous sommes ainsi passés sous la barre des 10%, du transport de marchandises. En Nouvelle-Aquitaine, le dernier CPER, donc Contra-Plate à région, mentionne une part bondale excessivement faible de l'ordre de 2,3 %. Si l'étude de vos services note que 2023 fut une année particulièrement marquée par une forte baisse imputable aux mouvements sociaux et aux prix élevés de l'électricité, elle démontre une tendance lourde que nous n'arrivons pas à redresser, y compris dans le transport combiné rail-route. Cette situation est un crève-coeur pour tous Français attachés au maillage du territoire et aux infrastructures que nous voyons dépérir et sous-utiliser. Surtout, on a à peine à comprendre ce démantèlement d'un outil majeur pour la décarbonation de nos échanges commerciaux et pour la sécurisation du transport routier. Parallèlement, le Parlement européen a voté une révision de la directive relative aux poids et dimensions visant à permettre la circulation de méga-camions. C'est déconcertant qu'un tel gigantisme routier soit poussé par la représentation européenne. Alors, on se demande comment pourrons-nous atteindre le doublement du trafic d'ici à 2030, pourtant acté dans la loi climat et résilience de 2021, à peine quatre ans plus tard, nous chutons. Mais certainement, Monsieur le Ministre, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer ? La stratégie nationale qui s'étale sur une période de dix ans évoque la mise en place d'actions à gain rapide. Pourriez-vous nous préciser les actions d'ores et déjà identifiées ? Le gouvernement annonçait un plan d'investissement de 4 milliards d'euros jusqu'en 2032, donc 900 millions pour l'État, en faveur du fret ferroviaire, la moitié passant par les CPEE que j'ai cité tout à l'heure. Le problème soulevé par la stratégie elle-même d'un CPEE voté ne permet souvent pas d'identifier les lignes concernées par de potentielles modifications. En outre, sans investissement, la pérennité de ligne capillaire n'excède pas 10 ans. D'autres projets plus emblématiques, je ne vais pas les citer, comme l'autoroute ferroviaire Cherbourg-Mougeard dans les Pyrénées, sont bien spécifiés, identifiés. Je tiens à saluer également dans un autre registre l'intégration de projets de frette fluviale, mais ce n'est pas l'objet, comme on a pu faire à Damazan, un sujet qui mériterait, monsieur le ministre, un débat à lui tout seul. Alors, M. le Ministre, pourriez-nous nous préciser où en sont les accords de programmation des abonnants au CPER, au contrat de l'Etat région, disposeront-nous bientôt d'une visibilité ? Et enfin, nous avions des sujets préoccupants dans le Sud-Ouest avec la création de la ligne GPSO entre Bordeaux et Toulouse. Nos citoyens s'en souviennent et et s'en souviendront longtemps, car elle contribue financièrement et c'est par juste titre. Nous avons un tracé qui avance aujourd'hui, mais ce n'est pas le débat non plus, nous avons un tracé qui avance aujourd'hui sans véritable réflexion sur le fret. Je crois, Monsieur le Ministre, qu'il est temps de mettre tout le monde autour de la table, et notamment nos entreprises, pour se rapprocher de leurs besoins en termes de frette et d'infrastructures de stockage. Vous le savez, le Lotte-Garonne et les départements voisins sont des départements producteurs de matières agricoles, mais également fabricants de matériaux de construction. On dispose d'atouts pour développer le frais de ferroviaire. Je pense à la ligne Agence Hoche, Agence Périgueux, pour lesquels j'ai déjà sensibilisé. Les projets viables sont d'ores et déjà sur la table. Et bien sûr, cela pourrait permettre de les engorger certaines départementales, notamment les Rennes Et enfin, dernière question. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que l'État prendra sa part dans la réouverture de ces lignes et ainsi contribuer au désenclavement de cette part du territoire et à faire de nos trois villes principales, Agen, Marmande et Villeneuve, des carrefour ferrovia

c'est terrible avec toutes les questions qui me sont posées je suis un peu frustré alors je vais simplement rappeler peut-être au sénateur Massé on en parlera peut-être sur d'autres questions concernant la position sur les mégatrucks lui dire que je suis également défavorable aux mégatrucks parce que entre autres ça fera sa frais perte 25% de d'activité aux frais de ferroviaire, très probablement. Je sais que d'autres sont d'un avis différent ici. ici. C'est pas à vous Jacques Fernic, je connais votre position sur le sujet. Moi je souscris à votre analyse M. le Sénateur concernant l'année 2023 qui a effectivement été marquée par des défis importants. Pour le secteur du fret cependant je note avec satisfaction que ça va un petit peu mieux, qu'on retrouve des couleurs en 2024 avec 33,1 milliards de tonnes kilomètres transportés cette année et le fret ferrovia rebondi de 12,1% par rapport à 2023. On est dans une dynamique qui est plus positive. Notre objectif est clair, il faut maintenir cette dynamique ascendante au cours des dix prochaines années. Vous l'avez rappelé, on avait fixé un objectif au sein de la commission de Jean-François Longereau et on garde cet objectif en tête. Pour y parvenir, il est essentiel que le secteur du fret ferroviaire continue à s'activer. Vous l'avez dit à travers la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, stratégie qui comprend 72 mesures concrètes que l'on essaie de mettre en place progressivement et avec une vraie dynamique et puis vous dire que le rôle de l'État sera bien entendu de sécuriser les financements dans le temps. On a parlé de la conférence de financement qui va nous réunir à partir du 5 mai prochain et la loi de finance 2025 prévoit aussi une enveloppe globale d'aide à l'exploitation des services de frais de ferroviaire et transports combinés. J'aimerais le rappeler quand même de 370 millions d'euros par les temps qui courent. C'est un arbitrage assez il est crucial que les régions également continuent à s'engager et puis vous vouliez une bonne nouvelle je vais vous en donner pour vous en exclusivité le service d'autoroute ferroviaire entre Cherbourg Cherbourg et Mouguère va pouvoir démarrer dans les prochaines semaines on vient d'avoir l'accord de la commission européenne bonne nouvelle pour le développement de ce secteur par un armateur privé merci monsieur le ministre pour le groupe union centrice la parole est à monsieur Jean-François Longiot président de la commission aménagement du territoire développement durable

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la loi climat et résilience du 22 août 2021 a fixé un objectif de doublement de la part modale du frais de ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur des marchandises d'ici 2030. Cette disposition, introduite dans le texte par un amendement du rapporteur de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable, un jeune sénateur prometteur, un certain Philippe Tabarot, est essentiel pour assurer la décarbonation du secteur des transports. Le transport de marchandises est en effet à l'origine de 13% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Depuis lors, le fret a fait face à une série de vents contraires. Grève sur les retraites en 2023, crise de l'énergie et inflation, effondrement du tunnel de la Morienne. L'année 2023 a été ainsi marquée par une forme de rapport modal inversé au profit de la route. La part modale du frais de ferroviaire est alors tombée à 8,9% contre 10% en 2022. La ligne de la Morienne a enfin rouvert le 31 mars dernier. J'espère donc que ces difficultés et difficultés conjoncturelles sont derrière nous. Monsieur le Ministre, pourriez-vous indiquer si le trafic a retrouvé une trajectoire de croissance l'année passée ? Quelles sont les perspectives pour l'année 2025 ? Il nous reste maintenant à nous attaquer à des enjeux structurels pour faire l'objet, fixé par la loi climat résilience, une réalité. Je pense en particulier au vieillissement du réseau ferroviaire, qui amène un ralentissement des circulations et une pénurie de sillons et eaux difficultés rencontrées par l'activité en vagons isolés. Le plan Ulysse fret réalisé par l'État, SNCF réseau et Alliance 4F soulignent que compte tenu de l'âge moyen élevé des lignes utilisées par le fret, il est urgent de mener des investissements, investissements sur le réseau pour éviter une baisse du trafic qui serait inéluctable sans changement de cap. Il prévoit donc d'accélérer les investissements au faveur du fret ferroviaire ? pour un total de 4,5 milliards d'euros entre 2023 et 2035 concernant notamment le renouvellement des voies de services frais, les équipements de tri à la gravité. L'indispensable pour le marché du wagon isolé, les terminaux du fret, les outils de développement du transport combiné et l'augmentation de la capacité du réseau ferroviaire en faveur du fret. Quel devrait être l'impact de ces investissements sur le volume du trafic ? L'objectif de doublément de la part modale du fret ferroviaire est-il encore atteignable d'ici 2030 ? Ces travaux pourraient-ils avoir un impact temporaire négatif sur le trafic ? Plus largement, les travaux sur le réseau ont souvent lieu la nuit pour ne pas pénaliser excessivement la circulation des trains de voyageurs. Comment faire en sorte de concilier la nécessité d'intervenir sur un réseau vieillissant et l'exigence de ne pas causer une interruption de trafic de forte ampleur dont le fret est souvent la première victime. Par ailleurs, la circulation de trains de voyageurs génère des ressources liées au pH ferroviaire, pH ferroviaire plus élevé que celle des trains de fret. Dans un contexte de manque de moyens sur le réseau, le gestionnaire d'infrastructure n'est donc pas incité à développer le fret. Comment répondre à cette difficulté ? Enfin, il est indispensable que les investissements programmés en faveur du fret soient effectivement réalisés. La Conférence nationale de financement des transports prévoit à ce propos un atelier consacré à et au verdissement du transport de marchandises. Avez-vous déjà étudié la nouvelle source de financement que vous envisagez de soumettre aux acteurs de la conférence de financement ? Pensez-vous que l'écotaxe poiloure qui sera bientôt mise en œuvre en Alsace pourrait être étendue à d'autres territoires et fléchée vers le financement des transports ? Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, que certains poids lourds, et ça a été dit tout à l'heure, contournent les autoroutes et que, effectivement, en adaptant et en utilisant des voies inadaptées à leur transit, comme la RN 83 dans le Doubs, ce qui dégrade l'état de la route est source de danger pour les usagers. Développer le fer de ferroviaire permettrait de diminuer le nombre de camions sur les routes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. 23 a été mauvaise pour un certain nombre de raisons, notamment la crise énergétique. Et puis, on a rendu hommage aux cheminots auxquels je m'associe. Il me doit de rappeler quand même que les mouvements sociaux, aussi justifiés soit-il, cher ami, aussi justifiés soit-il, ont fait du mal aux chiffres de l'année 2023. difficilement le nier. Pour autant, pour répondre aux questions du président Longiot, je souhaite lui dire que concernant les travaux, SNCF Réseau souhaite faire un effort tout particulier pour que le fret ne soit pas relégué Il est pleinement intégré dans la planification des travaux et je citerai d'ailleurs l'exemple des travaux qui vont se dérouler concrètement sur une ligne dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, la ligne Paris, Limoges, Toulouse, dire que contrairement aux pratiques antérieures, ces travaux seront réalisés en journée et cette décision vise à minimiser l'impact sur le trafic de fret. Vous dire également sur le sujet que vous avez abordé des périages ferroviaires, qu'à la différence des péages concernant le transport de voyageurs, les péages ferroviaires français demeurent parmi les plus bas d'Europe sur le fret. Et je dis bien sur le fret. 1,08 par train kilomètre contre 2 € en moyenne européenne. Nous travaillons également à l'optimisation des sillons via les plateformes services et infrastructures en intégrant les problématiques de travaux de nuit comme je viens de le dire. Et j'ai donc 15 secondes pour vous dire que concernant le sujet de l'éco-tax, un sujet que vous suivez tout particulièrement, vous savez qu'il est possible maintenant dans les régions frontalières grâce au travail de votre commission. On va avoir l'expérimentation de nos amis du Grand Est. et de la communauté européenne d'Alsace. Mais je me dois de dire à certaines personnes ici qu'il est bien dommage qu'à l'époque, une certaine Ségolène royale soit revenue en arrière sur la question de l'écotaxe. C'était 500 millions d'euros de recettes par an et donc 5 milliards, c'est exactement la somme que nous cherchons aujourd'hui. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Claude Vareas pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste, Kanaki. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis le vote dans cet hémicycle de la proposition de résolution de mon groupe déposé le 7 décembre 2022 traitant du développement du transport ferroviaire, ce sujet pourtant central pour nos mobilités, notre économie et la transition écologique est resté le parent pauvre de nos débats. Pas tout à fait néanmoins puisque nous avons eu à débattre de la sécurité dans les transports ou pour restreindre le droit de grève et stigmatiser les salariés du ferroviaire. Je les salue ces syndicalistes cheminots présents ce soir dans la tribune qui défendent de sans relâche les droits des salariés de la SNCF, des usagers et le service public de transport ferroviaire afin qu'ils retrouvent la place stratégique dont le pays a besoin. C'est de cette place dont nous débattons ce soir, deux ans après les annonces d'Elisabeth Borne, alors Premier ministre, qui brandissait un plan à 100 milliards d'euros d'ici 2040, tentant de faire oublier un contrat de performance particulièrement régressif. Depuis, cette nouvelle donne ferroviaire ne semble plus d'actualité pour le gouvernement, et la situation s'est aggravée. Le transport de voyageurs ne suit pas à cause du manque d'anticipation et du mauvais état du réseau. La SNCF applique la loi du marché et le manque d'offres s'adapte à la forte demande en proposant des prix exorbitants au détriment des usagers les obligeant à se rabattre vers des modes de transports plus polluants comme l'avion ou la voiture. alors que les transports constituent plus de 30% de nos émissions de CO2. L'effort public pour le développement du ferroviaire, saboté par des décennies de libéralisme, n'est pas au niveau des enjeux environnementaux et des engagements pris dans le cadre des accords de Paris. C'est particulièrement vrai pour le fait ferroviaire, puisque 24% des émissions issues des transports sont liées au poids lourd et donc au transport routier de marchandises. En 2021, dans la loi Climat et résilience, le Sénat avait introduit l'objectif louable de doubler la part modale du ferroviaire d'ici à 2030. Faute de moyens financiers pour les entretenir, les lignes capillaires qui connectent entrepôts et usines au réseau principal accusent une moyenne d'âge de 73 ans. Un quart des voies a été fermé ces six dernières années. La baisse du trafic ferroviaire est significative. moins de 19,6 % de frais conventionnels et moins 23,5 de transports combinés lorsque chez nos voisins européens le transport ferroviaire des marchandises poursuit sa croissance. Il gagne 22 % en Italie par rapport à 2019, 10 % en Allemagne, 2 % en Suisse. Le plan de discontinuité décidé par le gouvernement suite aux injonctions de la Commission européenne a porté un coup très dur au transport ferré de marchandises. Le 1er janvier 2025, Fret SNCF, démantelé en deux sociétés, a dû vendre du matériel roulant et abandonner 23 lignes, les plus rentables bien sûr, sur lesquelles Hexa Fret, le successeur de Fret SNCF, ne peut plus se positionner durant 10 ans. Un non-sens dans un pays qui veut se réindustrialiser. On nous répète qu'Exafred pourrait bénéficier d'une ouverture au capital mais qui viendra investir de l'argent dans une entreprise à qui on oblige de réduire ses parts de marché. Le manque de moyens alloués au transport ferroviaire de marchandises est une aberration à l'heure où nous devons de façon concomitante soutenir la réindustrialisation en produisant du matériel roulant, soutenir aussi les entreprises et nous serons plus attractifs en ayant un réseau de transport ferré développé, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, retrouver notre souveraineté et donc limiter la place des entreprises étrangères et les financements privés ou d'états étrangers qui les soutiennent. Je prends l'exemple de Keolis détenu à 30% par la Caisse des dépôts et placements du Québec. Nous le savons, le transport ferroviaire ne peut pas fonctionner sans un soutien public et la recherche de profits tout comme l'ouverture à la concurrence dans ce secteur sont forcément contraires à l'intérêt général. La recherche de la rentabilité maximum conduit à des suppressions d'emplois, à la dégradation des conditions de travail des salariés, à économiser sur la maintenance des infrastructures et des trains, à fermer des guichets, voire des gares si le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur souhaitée. Nous devons soutenir l'intermonalité en proposant un maillage au plus fin pour réduire la présence de camions sur les routes. Ce n'est malheureusement pas le choix fait par les gouvernements successifs. Des financements sont possibles, mon collègue l'a dit et je partage. Nous savons que les premières concessions autoroutières prennent fin en 2030. Nous défendons la renationalisation de ces autoroutes en conservant une logique de péage qui pourrait nous permettre de financer la décarbonation des transports. 1 milliard d'euros pourraient être alloués aux ferroviaires, 3,4 milliards pour les autres modes, dont la mise en place notamment des services express régionaux métropolitains. La France ne peut pas, Monsieur le Ministre, continuer à afficher des ambitions climatiques sans les traduire en actes. La relance du fret ferroviaire est une urgence, une opportunité industrielle, une exigence écologique et sociale. Merci. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Vareillas, j'aimerais vous rappeler quand même qu'un certain nombre de choses ont pu se faire ces dernières années sur cette question et notamment sur les moyens qui ont été donnés. Je rappellerai qu'il y a eu un triplement des aides à l'exploitation avec notamment la création d'une aide aux wagons isolés, le doublement des investissements de l'Etat en matière d'infrastructures. peut-être pour revenir sur cette question du plan de discontinuité du fret, je rappelle que la Commission Européenne a ouvert en janvier 2023 une procédure formelle d'examen sur certaines aides dont a bénéficié fret SNCF. Et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision du plan de discontinuité, c'est un de mes prédécesseurs et qui avait raison, parce que le risque était purement et simplement, même si vous n'en êtes pas tous convaincu, la disparition de l'activité fret SNCF avec un impact fort sur l'emploi de ses agents. Je vous rappelle que c'est l'emploi de 5000 cheminots qui était en jeu. Aujourd'hui, cette solution permet de sauvegarder ces emplois sans casse sociale. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. La discontinuité négociée reste proportionnée par rapport à une jurisprudence qui existe en la matière, celle d'Alitalia. En tout état de cause, nous avons garanti le respect de trois lignes rouges que je pense que vous partagerez aussi. préserver notre outil industriel, l'absence de licenciement et l'absence de report modal supplémentaire vers la route. Enfin, concernant la question du financement, Là aussi on est d'accord, alors peut-être pas sur la forme de la gestion des futures concessions autoroutières, mais un des objectifs, je le souhaite, de la conférence de financement qui débutera, et je continue la publicité, le 5 mai prochain à Marseille en présence du Premier Ministre et qui se déroulera sur dix semaines, j'ai souhaité, j'ai souhaité un atelier spécifique sur les quatre sur le transport de marchandises et j'espère que Nous pourrons aboutir après ces différents débats à ce qu'il y ait un fléchage très fort sur des financements sur le transport de marchandises et de préférence bien sûr qui viennent de la route et notamment des autoroutes. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Fernic pour le groupe Ecologie, Solidarité et Territoires.

du rapport de synthèse du cycle sur le frais de ferroviaire de notre commission développement durable. Ce débat est opportun, vous venez de l'évoquer, à la veille d'une conférence de financement. dont ce qui sortira particulièrement de l'Atelier 4 indiquera si oui ou non les ambitions de la France pour l'essor du frais de ferroviaire pourront être réalisées par une trajectoire adéquate d'ici 2040. Monsieur le Ministre, la volonté de votre gouvernement avec cette conférence est telle que soit établie et garantie les conditions de financement de la trajectoire d'investissement nécessaire pour l'essor du frais de ferroviaire d'ici 2040. Le débat de ce soir est aussi l'occasion de clarifier les impacts éventuels d'une loi de finances en voie d'être rabotée de façon significative, particulièrement le programme infrastructure et services de transport qui concerne notamment les actions 41 ferroviaires et 45 transports combinés. Monsieur le ministre, qu'en est-il précisément ? Le ferroviaire, notamment le fret, est-il ou non touché par ce nouveau reflux budgétaire de l'écologie ? La stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, Ulysse fret 2023-2032, subira-t-elle ce reflux ? Le milliard et demi supplémentaire par an d'ici 2027 et le plan de 4 milliards pour le fret d'ici 2032 sont-ils remis en cause ? Ce débat est également l'occasion de faire le point sur la situation présente du fret avec, on l'a dit, les mauvais résultats de 2023. qui ont remis en cause le début de tendance à la hausse qui s'amorçait depuis 2021. Il est sans doute encore trop tôt pour connaître les conséquences de la dislocation de fraîtes SNCF effectives depuis le 1er janvier, notamment y a-t-il report modal inversé ou non, mais vous avez sans doute des données récentes pour nous dire, Monsieur le Ministre, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la trajectoire fixée par la loi Climat ? Cet objectif intermédiaire de doublement, soit 18% de par modal en 2030, vous le maintenez ou vous y renoncez ? Monsieur le Ministre, chers collègues, il serait faux de considérer que l'effort à consentir pour le frais de ferrovia serait une charge, une mise sous perfusion coûteuse, parce que ce mode n'aurait pas son modèle économique. Alors certes, le wagon isolé nécessite par nature un soutien public pour être rentable. Certes, il s'agit de poursuivre le dispositif de prise en charge des péages dû par les opérateurs à SNCF réseau, qui place, vous l'avez dit, le coût de circulation des trains de fret en France nettement en dessous de la moyenne européenne. Mais ne perdons pas de vue les formidables atouts du ferroviaire qui le rendent si compétitif, au moins six fois moins de consommation d'énergie que le camion et neuf fois moins de carbone à la tonne transporté. Pour que ces avantages puissent déployer tout leur potentiel, des obstacles sérieux sont à lever. Pour bien les identifier, il faut élargir la focale au niveau européen. Les pays où la part modale du fret ferroviaire se situe entre 20 voire au delà de 30% sont ceux où les efforts sur l'infrastructure sont les plus significatifs et où il y a un effort déterminant de rééquilibrage compétitif entre la route et le rail. Le mode routier en effet ne pégère ses externalités négatives, dégradation des routes, nuisance, engorgement, accidentalité, pollution, contribution contribution forte à l'effet de serre et j'en oublie. Le pollueur n'est largement pas le payeur et cela creuse l'écart de compétitivité avec le rail. Je suis alsacien, du Grand-Est, je mesure la différence avec nos voisins européens. Notre Europe aujourd'hui, c'est le contraste entre au sud l'Espagne ou l'Italie qui ont basculé dans le tout camion, comme une bonne part de l'Europe de l'Est, et totalement différent. La Suisse, l'Allemagne ou les Pays-Bas, où le frais de ferroviaire est consistant, résulte d'investissements conséquents pour des sillons performants, des terminaux connectés, où le déséquilibre routeraille est corrigé par des taxes poids lourds significatives, on l'a déjà évoqué. Dégager ces recettes, ce serait permettre l'investissement massif nécessaire, l'investissement pour un réseau plus circulé par les modernisations CCR et ERTMS, et pour le fret que ces voies de service et l'étrillage soient maintenues et modernisées, car sans régénération de ces voies de service d'ici 10 ans, la moitié du trafic fret serait au mieux altérée, au pire arrêtée. On a manqué jusqu'ici en France de volonté franche d'augmenter les prélèvements sur le transport routier, En matière d'application de la directive eurovignette, on en reste au minimum et il faudrait actionner résolument le levier ETS et celui de la TICPE. De ce déséquilibre qui privilégie les routiers découle les autres obstacles qui s'opposent à l'essent du ferroviaire, l'insuffisante capacité d'un réseau vieilli, le déficit de la qualité de service qui privilégie le voyageur sur le fret, la pénalisation pour le fret du fait que les travaux sont réalisés de nuit et une ponctualité déficiente pour les trains de fret et enfin le déficit d'organisation avec une complémentarité entre le routier et le ferroviaire encore mal exploité alors que le potentiel du combiné est si prometteur. Enfin monsieur le ministre, comme si nous n'avions pas assez de difficultés à surmonter, Voilà que les camions très lourds de 44 tonnes en transit, voire les méga camions jusqu'à 60 tonnes et 25 mètres, menacent de leur impact désastreux et de leur concurrence. Le Sénat, par une résolution européenne dont j'ai été co-apporteur avec Pascal Gruny, vient d'affirmer clairement sa désapprobation. Cette désapprobation, vous la partagez Monsieur le Ministre, vous venez de le dire. Alors quelle perspective dans ce trilogue crucial, je crois que c'est à l'ordre du jour du Conseil de transport de juin, pour que ce projet de directive révisée ne tourne pas au détriment du fret Merci, cher collègue. La parole est à monsieur le ministre. matière d'investissement, l'État a démontré son engagement et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand vous avez parlé du budget et notamment du PLF 2020, 2025 je rappelle une nouvelle fois que c'est 370 millions d'euros par an dont une enveloppe qui a été significative sur le wagon isolé de 100 millions et j'en parle d'autant plus qu'elle est passée de 70 à 100 millions avec 30 millions d'euros de plus et je peux vous dire que dans les différents coups de rabot dont on a souvent parlé dans cette hémicycle d'avoir réussi l'an dernier à augmenter de 30 millions les sommes dédiées aux wagons isolés a été un petit exploit dont je suis particulièrement fier et j'espère que pour le PLF 2026 on restera sur cette dynamique pour tenir les engagements de la stratégie. S'agissant de la transformation de fret SNCF, les résultats sont plutôt encourageants. Exafret et Technis Opérationnel depuis janvier suivent leur trajectoire budgétaire. Une réorganisation sociale se déroule conformément aux engagements. Je les rappelle, deux tiers du personnel ont déjà retrouvé leur place au sein du groupe sans aucun licenciement économique. Les services ont été maintenus, évitant tout report vers la route. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, la signature toute récente d'un contrat d'exafraite concernant la sidérurgie de manière très significative et un contrat probablement qui sera signé prochainement également avec des céréaliers. Donc vous voyez que Exafret fonctionne et fonctionne plutôt bien.

refondre des systèmes d'information d'ASNCF réseau, mise en place d'indicateurs adaptés, mise en place de plateformes de services et d'infrastructures. Je peux sincèrement vous dire qu'il semble que plus que jamais ceux qui utilisent les services d'ASNCF réseau au niveau du transport de marchandises sont plutôt satisfaits de ce qui est fait en ce moment. par SNCF réseau pour pallier à ce qui a fait défaut ces dernières années, notamment en termes de qualité de service et donc que toutes ces mesures, je pense, tendent à rétablir cette qualité indispensable pour faire prospérer le fret et nous ramener aux engagements qu'on a pris dans la loi climat et résilience. Merci Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Jaquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Continue, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je veux à mon tour grandement remercier le groupe communiste pour ce débat qui peut sembler technique mais qui est en fait très politique tant les impacts du fret sont forts et pourtant si mal mesurés que ce soit en matière d'écologie, d'aménagement du territoire, d'économie, d'industrie, de défense, d'alimentation ou sur les enjeux sociaux. Oui, le fret ferroviaire est un vecteur essentiel de la réindustrialisation du pays et du continent. Oui, le fret ferroviaire est un maillon essentiel de notre système de défense à l'heure du retour de la guerre sur notre continent et de la nécessité de repenser notre stratégie nationale et européenne. Oui, le fret et le ferroviaire sont des outils essentiels d'aménagement durable du territoire et de lien entre les territoires. En cela, ils sont d'utilité démocratique. Oui, le fret ferroviaire est un outil indispensable face à la crise écologique. D'autres l'ont dit. Moins de camions, c'est moins de pollution. Moins de camions, c'est moins d'engorgements. Moins de camions sur les corridors européens, c'est moins de pertes de recettes pour l'État français du fait des traversées sans faire le plein de carburant sur notre sol. Moins de camions, c'est également moins d'usure de nos routes, d'autant plus qu'ils ne la payent pas. Nos routes sont presque toutes gratuites pour les usagers. Elles sont donc à la charge des contribuables. Il est particulièrement problématique que nos concitoyens payent pour des camions qui dégradent nos infrastructures, avec un rapport de 1 à 100 000, comparé aux voitures de monsieur et madame tout le monde. Et qu'en sera-t-il demain avec les mégacamiens, s'ils sont finalement autorisés à circuler dans notre pays ? Cette course au gigantisme doit cesser. Vous m'avez un peu rassuré sur ce point. Bref, vous l'aurez compris, le frais de ferroviaire, comme le fluvial quand il existe, est un des principaux vecteurs de réduction des externalités négatives du transport routier. Un gage d'efficacité et d'économie que nos amis suisses, allemands et autrichiens ont compris depuis longtemps et qui seraient particulièrement utiles à l'heure où vous recherchez 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors, assez d'action coup de poing, assez de tête à queue en matière de politique de transport, comme nous l'avons vu encore la semaine dernière avec le passeraille. Donnons une vision claire et des perspectives à un secteur d'activité qui ne peut se construire que sur le temps long. compte tenu des externalités positives du fret ferroviaire et fluvial, adaptons chez nous des solutions réglementaires qui ont fait recette ailleurs afin de les faire monter en puissance. À titre d'exemple, nos amis suisses et autrichiens ont institué des interdictions de circulation routière sur des axes dotés d'une véritable alternative ferroviaire. Et j'en viens au cœur de notre débat, M. le ministre. Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'évolution du fret ? Vous nous avez signifié que 2021 et 2022 ont vu la situation s'améliorer, mais pas en 2023. Mais qu'en est-il du nombre de flux et la volumétrie de marchandises transportées plus particulièrement ? ou en sommes-nous de la réalisation des 72 mesures de la stratégie nationale pour le développement du frais de ferroviaire de 2020, dont plusieurs jalons étaient fixés pour 2022. Sauf que ce départ est la première fois que nous pouvons en faire un véritable point d'étape, et nous la pressions. Dès lors, puisque nous sommes constitutionnellement chargés du contrôle de l'action du gouvernement, Pouvez-vous vous engager, monsieur le ministre, sur le fait de rendre compte régulièrement de l'évolution du secteur et des mesures à prendre pour le soutenir et l'aider à se développer ? Dans cette veine, comme d'autres avant moi, je ferais bien sûr avoir davantage d'informations quant à la pérennité ou non en 2026 des aides à la que nous avons rehaussée de 30 millions d'euros. Alors vous, vous l'avez précisé, que ces 100 millions Vous espériez les voir renouveler dans le prochain budget. Je l'espère également. Et on vous soutiendra. Surtout, la stratégie nationale pour le développement du frais de ferroviaire est-elle encore réalisable face aux 40 milliards d'économies d'économies que vous recherchez ? De même pour le plan Ulysse, publié il y a un mois et qui prévoit 4 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans. J'aimerais des précisions là-dessus. Je m'inquiète à ce titre de voir qu'une nouvelle fois vous souhaitez mettre à contribution les collectivités sur une politique qui est purement du ressort de l'État. En effet, après les injonctions faites au Département de Meurthe-et-Moselle et à la métropole de Nancy pour relancer une ligne d'équilibre du territoire vers Lyon, voilà que vous souhaitez intégrer le fret au contrat de plan État-Région à partir de 2027. C'est écrit noir sur blanc, page 19 de ce rapport. Par ailleurs, comment allez-vous continuer de lutter contre les mégacamiens si le fret continue de s'effriter ? Depuis le début de l'année, fret SNCF n'existe plus. Le plan de discontinuité a été mis en œuvre. Si nous continuons de penser que les gouvernements précédents n'ont pas du tout utilisé toutes les armes à leur disposition pour engager un véritable rapport de force avec la Commission européenne, C'est bien vers l'avenir qu'il faut se tourner. Concrètement, donc, quel est l'état de l'activité commerciale d'Exafret, et pouvez-vous nous rassurer quant à sa viabilité économique, puisque de nombreuses alertes ont été émises par les syndicats des professionnels du secteur en amont du plan de discontinuité ? Vous nous avez donné des premières informations. J'aimerais des précisions. Où en sommes-nous de l'ouverture potentiellement substantielle du capital d'Exafret qui était prévu par le plan de discontinuité ? Où en sommes-nous de la réattribution des 23 flux que devait obligatoirement lâcher la SNCF ? Vous avez indiqué que la route n'avait pas progressé par rapport à ça et que donc le ferroviaire tenait son rang, malgré cette discontinuité. Enfin, je ne peux conclure mon propos sans parler de la situation sociale du secteur de l'entreprise. Et j'en profite à cet endroit pour saluer l'engagement des cheminots. L'inglétude était forte en fin d'année. votre prédécesseur s'était voulu rassurant lors de ses rencontres avec les organisations syndicales, notamment concernant l'absence de plan social affiché, bien que les effectifs soient tout de même en diminution, à l'inverse du signal que nous voulons collectivement envoyer. Pour autant, le climat ne semble pas radieux, et les perspectives d'embauche dans le secteur ne sont pas au beau fixe. Comment arriver à développer le ferroviaire sans cheminots ? Il est plus que temps qu'en lien avec l'ensemble des acteurs, vous lanciez un grand plan sur l'emploi et les compétences, notamment dans le fret, parce que sans cheminots, point de train. Monsieur le ministre, nous nous sommes battus conjointement sur ces bancs pour renforcer les investissements publics sur un outil industriel stratégique pour le pays. Je forme le vœu que vous arriviez à sortir le frais de ferroviaire de l'impasse dans laquelle il semble se trouver. De même pour le fluvial, mais ce n'est pas le cœur de notre débat. Enfin, monsieur le Président, je ne peux terminer mon intervention sans émettre quelques propositions, surtout à une semaine de la grande conférence « France, avenir, transport », dont j'espère, monsieur le ministre, que vos réponses ne seront pas toutes cachées par cette perspective. Je pense utile que vous repreniez, puisqu'il faut le réviser, votre proposition de loi du 11 janvier 2022 pour mieux valoriser le fret dans le contrat de performance de SNCF-Réseau. C'était une belle proposition. Depuis quelques années, je me dis qu'il faudrait expérimenter l'obligation sur les axes des autoroutes ferroviaires de passer le transport de marchandises par le fer ou le fleuve plutôt que Seriez-vous prêts à lancer cette réflexion ? l'échec incroyable de l'écotaxe et c'est vraiment une erreur absolue. Je confirme qu'il nous faut relancer la généralisation d'une écotaxe poiloure en se mettant sur les pas de la région Grand-Est. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Vous avez deux minutes pour répondre à l'ensemble de ces questions. Quel exercice compliqué, M. le Président. Sénateur Jacquin, simplement vous dire que que je souhaite saluer votre détermination que nous avons en partage sur ce sujet. Nous en avons si souvent parlé. Vous dire, Penmel, que sur la question des méga camions, je vous ai dit ma position par rapport aux conséquences notamment que ça aurait sur nos routes, mais surtout surtout sur un report modal qui tuerait, je dirais définitivement, le fret ferroviaire avec moins 25% d'activité. Nous avons une partie à gagner. avant le mois de juin puisque la présidence européenne polonaise est plutôt défavorable au méga camion à la différence de la présidence danoise qui arrive ensuite donc on a le mois de juin pour essayer de régler cette question et je l'ai bien en tête et je mettrai toute l'énergie nécessaire pour le faire. Vous avez reparlé de la Suisse et de l'Autriche, mais là aussi, je le dis, vous l'avez rappelé, taxe fortement la route et ils n'avaient pas la chance d'avoir Ségolène Royale, donc ils ont pu mener la politique qu'ils souhaitaient au niveau de la route. Et puis, concernant la stratégie, les deux tiers des 72 72 mesures sont déjà en cours de mise en œuvre et je vous passerai les éléments nécessaires. Concernant Xafret, oui, Xafret va ouvrir son capital en 2026 comme il s'était engagé. J'ai une pensée aussi pour les 500 collaborateurs qui sont en train d'être reclassés sur l'ensemble du groupe et je crois savoir qu'il y a un accompagnement social, en tout cas c'est une demande. et je le souhaite sincèrement pour trouver une activité qui puisse les passionner dans le groupe SNCF de nouveau. Concernant la question du passeraille, vous l'avez évoqué, Le passereil c'était 12 millions d'euros. Nous préférons investir cet argent pour le fret parce qu'il y a eu peu de report modal et nous devons faire des choix. Les régions ont été vraiment peu à lente sur ce sujet mais ce n'est pas définitivement fermé. On trouvera peut-être un meilleur produit. Enfin, peut-être pour conclure un petit mot, soyons positifs sur la question du fret ferroviaire. Arrêtons d'en parler négativement. Moi j'ai reçu ces jours derniers tous les acteurs de 4F et je peux vous dire qu'ils y croient plus que jamais. Donc arrêtons d'avoir ce discours négatif, certes réaliste par rapport aux chiffres que vous avez, mais il y a une vraie envie de leur part de continuer à investir dans le frais de ferroviaire et à nous de savoir les accompagner utilement. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Jean Rochette pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires.

Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, permettez-moi d'avoir une voix non pas différente, un petit peu peut-être dissonante, mais complémentaire. Mais pour un débat qui parle du ferroviaire, avoir plusieurs voix, c'est jamais grave. C'est un petit jeu de mots. Oui, mais il est plutôt dans la thématique. Il n'est pas si mal que ça, pour le coup. À l'heure où notre pays cherche à concilier souveraineté économique et sobriété carbone, une évidence s'impose. Nous devons relancer le frais de ferroviaire, mais surtout, nous devons relancer tout l'écosystème autour du frais de ferroviaire. Parler du frais de ferroviaire seul, c'est une grave erreur. La chaîne logistique, elle ne se nourrit pas que d'une brique. Et pour qu'elle soit dynamique, performante et efficace, on doit travailler toutes les briques de la chaîne logistique. Parler du fret sans parler du reste, c'est surtout pas la solution. Et sur le temps long, le fret ferroviaire ne revivra jamais s'il est en opposition avec d'autres modes de transport. Et là, je vais revenir sur ce qui a été évoqué précédemment par mes collègues et revenir sur les propos de notre ministre. Je pense que s'opposer au mégacamion est une erreur en France. Je vous le dis comme je le pense. Je préférerais que nous réfléchissions à une expérimentation autour des mégacamiens qui servent le frais de ferroviaire. et encadrer cette expérimentation, qui pourra être uniquement à destination ou en provenance des plateformes multimodales, de manière à relancer, à compléter, à être en complémentarité avec le frais de ferroviaire plutôt que de l'interdire purement et simplement. Parce que les autres pays européens ne les interdisent pas. Et donc, on veut relancer le frais de ferroviaire avec une concurrence européenne qui, elle, pourra avoir des outils complémentaires tels que les mégacamions, Donc ils seront plus puissants d'un point de vue logistique, plus souples, plus agiles et nous on les interdit. Moi je crois qu'interdire de manière aussi brutale et avoir une position trop dogmatique n'est jamais la solution. Je pense effectivement qu'il y a des sujets qui doivent être traités autour de ces méga camions. Mais si on veut relancer le frais de ferroviaire qui est par nature la brique qui permet de transporter les plus lourds de charges dans l'organisation de la chaîne logistique, on ne peut pas se contenter de dire qu'à l'arrivée, pour le dernier kilomètre, on n'aura pas la capacité d'emporter des charges aussi lourdes et aussi volumineuses. La chaîne logistique, si on ne la traite pas de A à Z, on ne peut pas la redynamiser. Et c'est pour ça d'ailleurs que le routier est aussi puissant dans notre pays. Parce que comme elle ne fonctionne pas, c'est le routier qui prend le pas. N'opposons jamais les modes de transport. C'est la première des erreurs que nous ne devons pas faire. Et je vous le redis, avant de passer à autre chose, une expérimentation fermée autour du service du frais de ferroviaire sur les méga-camions me paraîtrait à la fois être une ouverture d'esprit écolo, parce que pour le coup, on veut aussi des camions électriques, mais si on ne veut pas alourdir le poids des camions en remplaçant le pétrole par des batteries, ça ne fonctionnera jamais. On perd sur la charge utile. Et moins en transport de marchandises, moins ça fonctionne. La complémentarité, elle est évidente. Sur le frais de ferroviaire aujourd'hui, le transport combiné, qui est la solution pour le frais de ferroviaire représente 41% du frais de ferroviaire en France. Mais le frais de ferroviaire lui seul ne représente que 10% du transport de marchandises. Donc on est en perte de vitesse totale depuis 20 ans face à nos concurrents voisins et amis pays allemands, suisses ou autrichiens qui eux ont une vision totalement différente de la nôtre. de l'usage du train, mais ils n'ont pas une opposition ferroviaire routier chez eux. Ils les font bosser ensemble C'est là que ça fonctionne. dire que les camions ne sont pas adaptés sur les grands trajets, je rejoins parfaitement, c'est le ferroviaire qui doit prendre cette place-là, mais on aura toujours le premier et le dernier kilomètre. Ensuite, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on travaille aussi sur les sillons, parce que les opérateurs aujourd'hui ont quand même du mal, quand ils arrivent à avoir une licence d'opérateurs ferroviaires, il n'y a pas que les opérateurs publics, il y a des opérateurs privés, Ils ont du mal à exploiter parce que les sillons ne sont pas de manière aussi simplement que ça a pu être été évoqué, donné par SNCF Réseau. L'objectif, c'est de moderniser et d'adapter les infrastructures, c'est une évidence, développer les plateformes multimodales et encourager la concurrence, faciliter l'accès aux rails, aux PME et aux petits opérateurs. Que nous ayons les opérateurs publics, aucun problème. Mais que nos logisticiens nationaux veuillent avoir accès aussi à des licences ferroviaires pour exploiter eux-mêmes du frais de ferroviaire sans passer par des opérateurs publics, ceci est une règle dans tous les autres pays où le frais de ferroviaire fonctionne. Et chez nous, les opérateurs privés sont en nombre trop faibles aujourd'hui. Si nous voulons développer le frais de ferroviaire, nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur des opérateurs publics. Et nous devons faciliter et accompagner les grands logiciens ou les petits qui ont la volonté de décarboner, qui ont la volonté d'avoir un accès au rail. Et puis je terminerai par... Le sujet de la réindustrialisation, bien entendu pas de réindustrialisation sans frais de ferroviaire performant puisque le frais de ferroviaire sert les industries massives. On va pas faire du travail d'épicier avec du frais de ferroviaire. Et réciproquement pas de frais de ferroviaire performant sans industries à desservir. Et là aussi il y a des sujets qui sont en connexion et en corrélation directe avec ce que nous traitons ici au Sénat, typiquement en termes d'urbanisme. Quand on crée une zédaïenne ou quand on veut aller installer un opérateur d'importance nationale en France, comment traitons-nous les sujets des terminaux ferroviaires en branché ? Au niveau urbanisme, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas penser une politique ferroviaire sans imaginer la connexion au réseau ferroviaire. Ce sont toutes ces thématiques que nous devons travailler et relancer pour relancer le frais de ferroviaire. Personnellement, j'y suis très favorable, mais nous devons aussi élargir notre spectre, notre esprit sur ces dossiers-là. Merci. M. le Président, M. le Sénateur Rochette, je vous laisse vous installer. Allez-y, faites le Président de Commission. Si le Président Longet, il est parti, on ne lui dira pas. Je partage Je partage votre position sur pratiquement tout. Mais je vous l'ai dit, sans opposer les modes de transport les uns après les autres, et c'est ma philosophie depuis que je suis engagé dans le domaine des transports, Je pense sincèrement que la complémentarité existe, mais en l'occurrence, sur ce mode bien spécifique, je pense que le coût serait fatal. En tout cas, je respecte votre position, mais je ne la partage pas. Par contre, je partage totalement votre vision sur la clé qu'est le transport combiné. C'est une solution d'avenir, vous l'avez indiqué, des chaînes multimodales vertueuses, notamment par le biais des services de transports combinés qui combinent le transport ferroviaire avec le préacheminement et l'acheminement du container par la route, permettent d'envisager un report modal. Alors c'est précisément là où on a renforcé notre engagement avec une enveloppe annuelle de pratiquement 50 millions d'euros depuis 2021 pour soutenir l'exploitation de ces services. Vous évoquez aussi la nécessité d'action concrète. Nous essayons d'y répondre. Nous avons piloté l'élaboration du schéma directeur de transports combinés, alors là qui va plus loin de 32 à 42, qui a été publié en octobre dernier. C'est un document stratégique qui dessine le maillage cohérent des plateformes sur l'ensemble du territoire. Et vous avez parlé également du raccordement direct de certains sites. au réseau ferré national nous avons obtenu de la commission européenne l'autorisation de soutenir financièrement ce qui n'est pas toujours possible ses investissements l'état ainsi que les régions qui ont décidé de financer ses projets dans le cadre du cpr des fois l'état finance des projets qui sont uniquement régionaux de temps en temps ce sont les régions qui vont sur des sujets qui sont plutôt du ressort de l'état mais je pense que c'est ça un bon partenariat entre les collectivités et peut-être vous dire sur les sillons je l'ai dit tout à l'heure mais il y a vraiment une démarche qui est vertueuse et qui est mise en oeuvre à travers les plateformes d'infrastructure et services et qui permet d'assurer une meilleure qualité de service pour réseau et d'avoir plus de visibilité sur les sillons c'est la clé d'une réussite indispensable pour pouvoir retrouver un certain nombre de clients qui se sont démotivés par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient et détournés vers d'autres modes de transport qui ont le mérite d'exister mais si on peut décarboner à travers le frais de ferroviaire ça reste quand même et avant tout une priorité. Merci monsieur le ministre. La parole est à madame Agnès Canaillet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je connais, Monsieur le Ministre, votre forte implication et votre grande expertise depuis longtemps sur ces sujets du transport ferroviaire. Et je voudrais moi aussi remercier le groupe communiste pour l'organisation de ce débat qui me permet de vous interroger sur la connexion entre le fret ferroviaire et nos ports. Là encore une nouvelle brique. En effet, en tant qu'élu du Havre, je mesure tous les jours la nécessité d'une multimodalité pour le transport de marchandises. Aujourd'hui, un conteneur qui arrive dans le port du Havre a huit chances sur dix de prendre la route, une chance et demie de passer par la Seine et une demie chance sur dix d'utiliser le rail. Le train comme mode de transport des marchandises est donc bien résiduel. Ce constat aduit malheureusement des conséquences environnementales et économiques. Il pose inévitablement la question de savoir comment garantir demain une logistique décarbonée performante et une meilleure compétitivité face aux défis climatiques et géopolitiques. Comment garantir que nos ports, par lesquels transitent plus de 325 millions de tonnes de marchandises, soient connectés à un réseau ferroviaire performant pour développer la multimodalité. En France, cela se traduit par la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire inscrit dans la loi climat et résilience qui fixe des objectifs ambitieux. Vous l'avez tous déjà annoncé cet après-midi. Cette feuille de route vise un doublement de la part modale du fret ferroviaire en France de 9% en 2019, 2019, 18% en 2030 et un objectif de 25% à horizon 2050. Il y a donc urgence pour atteindre la cible, car malheureusement cette ambition se heurte à une saturation chronique du réseau ferroviaire, conséquence directe de nos lignes obstruées, particulièrement en Normandie. C'est pourquoi la ligne nouvelle, Paris-Normandie, est tant attendue, et pas seulement par les Normands, qui sont depuis toujours exclus de la grande vitesse, mais surtout par l'ensemble des acteurs économiques et portuaires qui sont là des promesses 60 fois repoussées. Faire du Havre, le port de Paris, n'est pas une idée nouvelle. D'ailleurs, toutes les grandes puissances maritimes ont leur capital relié à un port. Et si Aropa donne corps aujourd'hui à l'Axe Seine, le lien entre la capitale et le port du Havre ne peut pas être simplement fluvial. Pensé dès 1991, porté en 2009 par le président Sarkozy, soutenu par tous les gouvernements depuis, la LNP est aujourd'hui toujours bloquée par une opposition de la région de France et par la lenteur des études préalables. Cette ligne est indispensable, non seulement pour les passagers, mais surtout pour le fret. Elle désaturerait le réseau existant, soulagerait nos autoroutes et favoriserait une dessert efficace de Paris, principal bassin de consommation, et elle étendrait aussi l'interland port-fer. Aujourd'hui, Aropa traite 80% de ses volumes dans un rayon de moins de 160 kilomètres. C'est insuffisant quand les ports du range nord atteintent eux 250 Si nous voulons réaliser, nous voulons aussi que l'Axe Seine devienne une véritable colonne vertébrale logistique nationale. Pour cela, il faut faire sauter les verrous qui bloquent la LNP. Le coût total du projet est estimé certes à 10 milliards d'euros, avec une réalisation par phase prévue à l'horizon 2040. Néanmoins, nous manquons encore de clarté de la part de l'État sur sa participation au financement et la tenue du calendrier. En attendant, d'autres leviers existent pour pallier le manque d'attractivité du fret ferroviaire. Le premier levier est d'investir massivement dans le réseau stratégique dédié aux frettes. Les lignes et les terminaux doivent être renforcés, notamment pour augmenter les maillages et les signaux. Le deuxième levier consiste à s'inspirer des bonnes pratiques européennes. Cela a déjà été dit, notamment de la Suisse, qui depuis 2016, grâce à la loi, réserve à long terme des sillons pour le fret, assurant ainsi une planification pérenne et équilibrée entre les trains de massagers et ceux de marchandises. Je me félicite car OPA, POR et SNCF réseau se soient engagés dans la recherche de solutions concrètes pour trouver des solutions sur le développement du ferroviaire. Cette recherche d'accord marque une étape importante dans le déploiement du frais de ferroviaire car elle soutient la création d'un corridor logistique et industriel décarboné à l'échelle de l'AXE en lien avec la stratégie nationale bas carbone et l'objectif de neutralité d'ici 2050. Enfin, si l'enjeu du report vers le frais de ferroviaire est avant tout celui de la massification du transport de marchandises et sa décarbonation, le coût des modes de transports combinés ne peut être évincé. Je me permets d'insister sur un point trop souvent peu évoqué et pourtant essentiel à la compétitivité du transport ferroviaire, à savoir les aides aux transports combinés, aussi appelées aides à la pince. Elles s'élèvent à 23 euros par transbordement, couvrant ainsi une partie du coût réel de l'opération. Elle permet de réduire l'écart de compétitivité entre le rail et la route. L'enveloppe budgétaire allouée dans le cadre du plan fret était d'ailleurs de 47 millions d'euros par an pour la période 2021-2024. La stratégie nationale du développement du fret ferroviaire a prévu de maintenir ce niveau d'aide jusqu'en 2027 et le président du gouvernement a pris l'engagement en novembre dernier de préserver ce soutien complémentaire jusqu'en 2050. c'est bien, mais il faut aller encore plus loin et concrètement concentrer ces aides sur les axes stratégiques. Face aux impératifs climatiques et énergétiques pour le développement du transport de marchandises, le fret doit être la solution. Nous savons tous ici que le rail est un mode de transport massifié par excellence pour tous les grands pays. L'objectif est donc clair, faire du frais de ferroviaire, non pas un supplément, mais un pilier de notre politique industrielle, environnementale et territoriale. Monsieur le Président, Madame la Ministre Canaillier, merci de me permettre de parler des grands ports maritimes. Comme vous le savez, la mobilisation des modes massifiés que sont le ferroviaire et le fluvial pour la desserte des Interland est un enjeu majeur pour les ports et en particulier pour les grands ports maritimes, massification des flux de marchandises, levier de croissance et d'attractivité pour les ports français liés avec l'optimisation de flux du transport maritime lui-même. Alors quelques chiffres. En 2023, 22,5% des prêts et post-acheminements portuaires sont réalisés sur les modes massifiés. 11,5% par le fer, 11% par le fluvial. Ce niveau se maintient stable depuis la sortie de la crise sanitaire, mais nous devons collectivement être plus ambitieux. C'est pourquoi nous avons mis en place deux stratégies nationales complémentaires, la stratégie portuaire en 2021 et la stratégie nationale du fret ferroviaire en 2022. Ces documents cadres se traduisent par des engagements financiers, 164 millions mobilisés entre 2023 et 2027 pour améliorer la décerte de la multimodalité ferroviaire et fluviale de nos ports maritimes. Concernant spécifiquement le port du Havre, qui vous est si cher à juste titre, la logistique et la multimodalité sont au cœur de son développement, premièrement sur le volet fluvial avec la réalisation de la châtière qui sera opérationnelle en 1926. Cet aménagement vise à connecter directement au fleuve le port en eaux profondes de Port-de-Mille qui accueille les principaux terminaux et conteneurs du Havre comme vous le savez renforçant considérablement l'efficacité de notre chaîne logistique. Et, deuxièmement, sur le volet ferroviaire à Ropaport il poursuit la régénération et la modernisation du réseau ferré portuaire avec notamment une opération de 25 millions d'euros pour les décès terrestres de Port-de-Mille. En parallèle, projet structurant Port Seine métropole ouest, plateforme multimodale, Viendra compléter ce dispositif d'ici 2040 avec un investissement de plus de 120 millions d'euros. Voilà madame la sénatrice, la détermination du gouvernement à faire du Havre à Homme multimodal d'excellence. LNPM, j'aurais voulu en dire plus mais j'ai conscience du caractère primordial de ce projet pour votre région normandie. A ce titre, M. Serge Castel est le nouveau délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine. Il a été nommé tout récemment et il doit poursuivre au plus vite la concertation auprès des élus. Nous allons l'installer officiellement et je présiderai le premier comité de pilotage. Merci M. le Ministre. La parole est à Mme Marie-Laure Finérat-Hort pour le groupe rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous débattons aujourd'hui d'un sujet majeur pour notre économie, pour l'environnement et pour l'avenir de notre système de transport, celui du fret ferroviaire. Nous le savons tous ici, le fret ferroviaire a connu de nombreuses difficultés en France. Entre 1990 et 2000, le trafic a resté relativement stable, autour de 52 milliards de tonnes kilomètres. Puis, à partir des années 2000, il a commencé à baisser régulièrement. La crise économique de 2008 a fortement aggravé la situation. En 2010, le trafic est ainsi tombé à 30 milliards de tonnes kilomètres et depuis, il n'a pas vraiment rebondi. La part du frais de ferroviaire dans l'ensemble du transport de marchandises a, elle aussi, chuté. Elle est passée de 20% en 1990 à environ 10,5% depuis 2006 et ne progresse plus. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs connus. D'abord, la France n'a pas une géographie industrielle favorable à un réseau ferroviaire performant. Les sites de production sont dispersés, ce qui rend difficile la concentration des flux nécessaires à la rentabilité du rail. Ensuite, la part de l'industrie dans notre économie a fortement baissé ces 20 dernières années. Enfin, de nombreux clients demandent aujourd'hui des livraisons très rapides et flexibles, ce qui favorise davantage le transport routier. Pourtant, le fret ferroviaire a de nombreux avantages. C'est un mode de transport beaucoup moins polluant que la route. Il consomme moins d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre. Un train de marchandises remplace plusieurs dizaines de camions. Cela signifie moins de bouchons, moins d'accidents, moins de pollution. Dans le contexte actuel de transition écologique, Il est essentiel de développer des modes de transports propres et le frais de ferrovia en fait partie. Il permet aussi de renforcer la résilience de nos chaînes logistiques et pourrait jouer un rôle important pour désengorger les routes et pour mieux organiser nos flux de marchandises à l'échelle du pays. Mais relancer le frais de ferroviaire demande des investissements importants. Il faut moderniser les infrastructures, remettre en service certaines lignes abandonnées, construire de nouveaux terminaux. Il faut aussi adapter le réseau aux besoins actuels, augmenter la capacité, faciliter les connexions entre rails et routes, rendre le système plus fiable. Face à ces enjeux, le gouvernement a lancé en 2021 une stratégie nationale pour le développement du frais de ferroviaire et en mars dernier a été publié le rapport ULIS, élaboré conjointement par la DGITM, du ministère des transports, SNCF réseau et Alliance 4F. Ce rapport prévoit notamment 4 milliards d'euros d'investissement sur la période 2023-2032, dont 2 milliards déjà engagés d'ici 2027. Il propose des actions concrètes comme la remise en état de 2 700 km de ligne, dites capillaires, utilisées principalement pour le fret. Près de 200 millions de roues sont également prévues pour moderniser la gestion du trafic et améliorer le partage de données. Ce programme Ulysse va dans le bon sens, mais pour qu'il soit une réussite, plusieurs conditions doivent être réunies. Et c'est en ce sens que j'aimerais vous interroger, Monsieur le Ministre, comment allez-vous garantir que ces investissements soient bien réalisés dans les délais prévus ? et assurer le suivi du plan Ulysse. Et comment le gouvernement tente-t-il garantir la pérennité des lignes de fret existantes, notamment celles menacées par des restructurations et les petites lignes avec le démantèlement de fret SNCF ? Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, merci d'avoir presque tout dit dans votre intervention et d'avoir résumé je pense une grande partie de notre débat. Le gouvernement a pleinement conscience des impacts à la fois écologiques et économiques. qu'aurait un désengagement du fret ferroviaire. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'un soutien massif et structuré au secteur, vous l'avez dit, notamment à travers la stratégie nationale pour le développement. Cette stratégie se traduit par deux engagements financiers qui, je pense, répondent à vos questions. À la fois le renforcement considérable du soutien à l'exploitation et puis deuxièmement l'effort massif sur les infrastructures et notamment la rénovation des voies si capillaires, si importantes au fret ferroviaire. cet effort doit maintenant être amplifié. Vous l'avez dit, c'est tout l'enjeu de la conférence de financement Ambition France Transport qui s'ouvre lundi, je crois que c'est le 5, en présence du Premier Ministre et encore une petite page de publicité. Je plaide depuis des années pour que les recettes des transports financent le développement de l'ensemble des transports et concernant spécifiquement le rapport dont vous avez parlé Le rapport Ulysse Fred qui a été publié en mars dernier, il constitue véritablement notre feuille de route pour la période 2023-2032. Ce document est le fruit d'une large concertation, vous l'avez dit, avec l'Etat, SNCF réseau est vraiment, et c'est là le plus important, les acteurs de la profession. Il pourra servir de base à la prochaine conférence de de financement. Enfin, sur la question des livraisons rapides que vous avez évoquées, vous avez raison de souligner qu'elles contribuent à renforcer le mode routier. Cela doit nous appeler à envisager de nouvelles évolutions pour gérer leurs conséquences. Et nous avons commencé à travailler sur ce sujet il y a un certain nombre de mois, voire même d'années, à travers l'excellent rapport de Nicole Bonnefoy et de Rémi Pointreau qui doit maintenant rentrer en application de manière très concrète et très volontariste. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Franck Dersin pour le groupe Union Centriste.

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je remercie moi aussi le groupe communiste d'avoir mis à l'ordre du jour ce débat sur la relance du fret ferroviaire, car on l'a entendu, il y a évidemment beaucoup à dire. Nous avions tous ici pour ambition que la part modale du fret ferroviaire s'approche de 25% à l'horizon 2030. d'ores et déjà acquis que cet objectif ne sera évidemment pas rempli. Pire encore, il semblerait que sur l'année 2024, la part modale du fret est même un peu régressée. Les années passent et le constat demeure. Pourquoi a-t-on tant de mal à faire progresser le transport ferré de marchandises dans notre pays alors que sa part modale est deux fois plus élevée outre Rhin et trois fois plus élevée chez nos voisins Helvet ? Quand on interroge les chargeurs, on s'aperçoit que le critère fondamental pour eux, c'est le respect des délais d'acheminement. Trop souvent, il faut le dire, le fret est devenu la variable d'ajustement du réseau avec des sillons insuffisamment qualitatifs, souvent perturbés par des travaux nocturnes. Les temps de trajet ne sont pas assez compétitifs face au mode routier, c'est clair. On peut également noter l'état général du réseau comme élément majeur d'explication. Les lignes dites secondaires, très empruntées par les trains de marchandises, souffrent d'un manque criant d'investissement et ne permettent pas de rouler à une vitesse commerciale satisfaisante. Pour ne pas nous répéter inlassablement, et comme la totalité des groupes politiques ici avaient souligné à l'occasion du projet de loi de finances un manque d'investissement de l'État dans le réseau, je vais ici faire une proposition, Monsieur le Ministre, qui pourrait nous aider à rendre notre réseau plus robuste et à infiner, faciliter les circulations de fret comme de voyageurs, de toute façon. Le système européen d'échange d'émissions carbone, l'ETS, connaît une augmentation importante de ses recettes depuis deux ans. Depuis 2024, une directive européenne oblige les États membres à flécher 100% de ses fonds vers des dépenses vertes. Une partie l'est d'ores et déjà vers l'ANA dans un objectif de rénovation de l'habitat. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas flécher une autre partie vers la régénération du réseau ferroviaire plutôt que de l'envoyer dans le budget général de l'État où il sera incapable de savoir si cet argent a bien été utilisé pour des projets favorables à l'environnement ? Ma proposition serait d'enfléchir une partie de manière inconditionnelle et pérenne à l'entretien du réseau et une autre partie en dédommagement à SNCF réseau, en contrepartie d'une baisse des péages ferroviaires sur des desserts jugés non rentables aujourd'hui afin de stimuler le nombre des circulations. Les opérateurs alternatifs pourraient apporter, grâce au payage généré, environ 600 à 900 millions d'euros de recettes annuelles supplémentaires pour le réseau d'ici 2030 Ainsi, sur une échelle de 10 ans, nous arriverions à environ 1,5 à 2 milliards d'euros par an, de recettes supplémentaires pour le réseau en se basant sur une affectation de l'ETS au moins égale à celle destinée à l'ANA, c'est-à-dire 700 millions d'euros aujourd'hui. Nous ne ferons pas de miracle avec le peu de moyens financiers actuels. Il faut faire preuve d'audace si nous voulons redresser notre réseau et ainsi redonner de la compétitivité à ce mode face à la route. Pourriez-vous donc nous indiquer, monsieur le ministre, si vous comptez défendre auprès du Premier ministre cette position et convainc enfin le gouvernement de flécher une partie de l'ETS vers le secteur ferroviaire ? Et rendez-vous tous le 5 mai à Marseille. le monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Dersin, merci pour votre intervention. Sur le constat et sur les objectifs, vous les avez donnés. vous les avez donnés. Après les objectifs, vous les avez donnés un petit peu plus haut que ce qu'on avait fixé. Vous avez parlé de 25 %. C'est un objectif extraordinaire et c'est ce que font d'autres pays européens. Mais l'idée, c'était de doubler la part. À l'époque, elle était de 9 %. Aujourd'hui, elle est d'un petit peu plus de de 10% pratiquement 11% et l'objectif était et reste de 18% pour des raisons que vous avez rappelées sur un certain nombre d'explications et plus de deux autres que je rajouterai à la fois la crise de notre industrie depuis un certain nombre d'années ainsi que la non taxation de la route mais je ne vais pas rajouter une couche pour l'ancienne ministre chère Olivier. Pour autant, vous avez parlé d'autres formes de financement. Bien sûr, je suis naturellement favorable à l'affectation de nouvelles recettes. Alors je pense qu'il y a plusieurs pistes et on en parlera dans la conférence de financement qui se tiendra le 5 mai, je ne l'ai peut-être pas dit, à Marseille en présence du Premier Ministre. Je compte aussi sur cette conférence pour faire preuve d'innovation. Et pourquoi pas de créativité pour identifier des sources pérennes de financement. on a évoqué quelques pistes notamment sur la route. Nous avons également à réfléchir comme le propose l'Alliance 4F sur un financement privé potentiel sur certains aspects. vous l'avez très justement dit, je suis favorable à l'affectation de nouvelles recettes au secteur des transports. qui touchent notamment la question des ETS, ce que je peux vous dire, mais vous l'avez rappelé, nous ne sommes pas les seuls sur le coup, mais qu'il est tout à fait logique et normal que ces sommes puissent revenir en partie au secteur des transports, en tout cas Je n'ai pas attendu la conférence de financement pour essayer d'installer cette idée au niveau des services du Premier Ministre et bien sûr de Bercy et j'espère que la conférence de financement nous permettra d'avancer sur ce sujet. En tout cas, c'est mon objectif et je sais qu'il est partagé par un certain nombre d'entre vous et notamment vous, M. le Sénateur. Merci M. le Ministre. Pour la dernière question, M. Jean-Marc Delia pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mes chers collègues, La relance du fret ferroviaire est un enjeu majeur qui focalise toutes les attentes autour de la transition écologique, de la compétitivité économique et de l'équilibre de nos territoires. En tant que petit-fils de cheminots, Ce sujet me touche particulièrement. J'ai grandi avec les récits de ces femmes et de ces hommes qui ont fait vivre notre réseau ferroviaire, souvent dans l'ombre, mais avec une passion et un dévouement sans faille. Aujourd'hui, le gouvernement affiche une ambition forte, doublée la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030, de 9 à 18 %, conformément à la loi Climat et résilience. Cette volonté réaffirmée dans la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire s'appuie sur plusieurs axes structurants et sur le programme Ulysse fret, dont la feuille de route a été précisée en mars 2025 par le ministère des transports, SNCF réseau et l'Alliance 4F. Soyons clairs, pour relancer le fret ferroviaire, il faut des actes forts, pas seulement des discours. Le premier pilier de la construction, c'est l'investissement massif avec le plan Ulysse-Fret. De quoi moderniser notre réseau, rénover nos gares de triage, créer de nouveaux terminaux de ferroutage et redonner vie à nos lignes capillaires. Ces investissements sont vitaux. Il s'agit de préparer l'avenir d'éviter la dégradation du service et de garantir que plus de la moitié du trafic fret ne soit pas menacée dans la décennie à venir. Dès 2026, 62,5 millions d'euros seront injectés chaque année, puis 75 millions d'euros par an pour entretenir et rénover nos voies de service. On ne parle pas de rustine, mais d'une vraie cure de jouvence pour notre réseau. Cette évolution nécessaire doit s'appuyer sur l'héritage d'un réseau déjà existant que des générations de cheminots ont patiemment tissé. Le deuxième pilier repose sur un soutien financier renforcé de l'État. Ce n'est plus 170 millions d'euros par an, mais 200 millions d'euros par an qui seront versés chaque année jusqu'à 2030. Ce soutien, c'est le gilet de sauvetage du secteur. alors que la rentabilité reste fragile, notamment avec la transformation de fret SNCF et la création de nouvelles entités comme Hexafret et Technis pour répondre aux exigences européennes. Cette stabilité financière offre la visibilité nécessaire aux opérateurs pour investir et innover. Le troisième pilier concerne le développement du transport combiné et de l'intermodalité. La stratégie nationale vise à tripler le volume du transport combiné en 10 ans, en modernisant les infrastructures multimodales et en améliorant l'articulation entre rails, fluviales et portuaires. En 2025, le schéma directeur des transports de semi-héromorques va donner un vrai coup d'accélérateur à cette dynamique. Le quatrième pilier porte sur l'amélioration de la qualité de service, fiabilité, ponctualité et compétitivité, les maîtres mots, On mise sur la digitalisation, l'innovation, la simplification des procédures pour les chargeurs. Grâce à Ulysse Fret, on veut offrir un service moderne, efficace, à la hauteur des attentes du marché. Cependant, les défis sont importants. La concurrence de la route reste avec sa flexibilité et ses coûts souvent imbattables. Le modèle économique du fret ferroviaire est encore fragile, plombé par des péages élevés et un manque de visibilité à long terme. Comme le disent souvent les cheminots, un train qui passe, c'est des dizaines de camions au moins sur les routes. Aujourd'hui, plus que jamais, cette maxime doit guider nos politiques. Les contraintes européennes, avec l'obligation pour fret SNCF de céder des activités rentables, fragilisent la filière et risquent de renvoyer des flux vers les routes. Enfin, la modernisation du réseau exige une planification rigoureuse pour répondre aux besoins de la logistique urbaine et des dessertes fines du territoire. Dans ce contexte, le programme Ambition France Transport, pilier de la relance, doit apporter des réponses concrètes. Investissement massif, soutien financier pérenne aux opérateurs et promotion de l'innovation et de l'intermodalité, levier indispensable pour répondre aux attentes des chargeurs et accompagner la transition écologique du secteur. Pour conclure, mes chers collègues, relancer le frais de ferroviaire, c'est comme mettre sur les rails un train plus performant. Ça demande de l'huile de coude, des investissements solides et de la technicité. mais c'est aussi un devoir envers ceux qui ont fait du rail l'épine dorsale de notre économie. Avec ambition France, ce train-là pourrait arriver jusqu'à destination. Alors, avec l'état, les collectivités, les opérateurs, chargeurs, embarquons tous ensemble dans ce train de la transition écologique avant que seuls les transports routiers ne prennent définitivement la tête du convoi. C'est à ce prix que nous réussirons la transition écologique, renforcerons la compétitivité de nos entreprises et offrirons à nos territoires un avenir logistique, durable et performant. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Délia, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux et quelque part fier de vous voir et de vous entendre sur cette tribu. Deuxièmement, vous dire que le gouvernement est persuadé de la nécessité de soutenir le développement du frais de ferroviaire. Vous l'avez très bien rappelé. Dans votre intervention, les chiffres sont éloquents. Il émet neuf fois moins d'émissions de CO2, consomme six fois moins d'énergie à la tonne kilomètre de marchandises transportées que le fret routier. Vous avez raison de souligner que la relance du fret ferroviaire nécessite à la fois de la persévérance et des investissements conséquents. C'est exactement la ligne que nous suivons avec la stratégie nationale. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là et c'est pour cette raison, vous l'avez dit également, qu'une stratégie claire et des actions partagées Pour l'ensemble des acteurs du secteur a été défini dans le cadre de la démarche Ulysse-Fret. Il nous permet enfin d'établir une priorisation, et c'est peut-être là le plus important, des investissements sur les infrastructures ferroviaires nécessaires à son développement. Cela étant dit, il faudra en effet faire preuve de patience pour obtenir des résultats concrets garantissant une augmentation significative du report de la part modale. dans le fret de ferroviaire. Comme vous le savez, le temps ferroviaire nécessite un temps long et sensible aux différents aléas. Le premier défi devant nous est de garantir le bouclage du financement de la démarche. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que le fret ferroviaire soit, et nous l'avons dit plusieurs fois, un thème à part entière de la conférence de financement que nous lançons Lundi prochain, 5 mai, à Marseille, en présence du Premier Ministre. Je souhaite que cette mobilisation des acteurs se poursuive dans ce cadre, notamment sur une base solide, celle du rapport ULIS, et que l'engagement de tous puisse in fine soutenir l'ambition que nous avons pour ce très beau secteur. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Est-ce que vous souhaitez prolonger par une conclusion, avant que je ne laisse la parole à Monsieur Jean-Pierre Corbusier ?

? Monsieur le Président. Je vais essayer de profiter pleinement de ces cinq minutes. J'avais besoin de plus de temps pour répondre à toutes les excellentes interventions de nos collègues, chères sénatrices, mesdames et messieurs les... Les sénateurs, nos débats de ce soir ont mis en évidence, je le pense, le défi concret auquel le fret de ferroviaire est aujourd'hui confronté. En regardant dans le rétroviseur, je pense que nous pouvons être fiers de la première étape réalisée ces dernières années pour soutenir ce fret de ferroviaire. Tous les acteurs ont travaillé ensemble pour faire avancer et donner une nouvelle chance à ce secteur essentiel. pour la décarbonation de nos transports. Je tiens à souligner ici le travail structurant et visionnaire de l'Alliance 4F qui a permis de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière et peut-être au moment le plus difficile. Bien sûr, l'État SNCF réseau qui accomplit un travail remarquable sur cette question du fret, les entreprises ferroviaires, le PSF et le CEREMA autour d'objectifs communs et afin de définir une stratégie concertée du développement du fret ferroviaire. Cette dynamique se poursuit et fait l'objet d'un suivi rapproché pour en garantir la mise en œuvre. Grâce à ce travail collectif, nous avons mis en place une stratégie unique au service du fret ferroviaire avec quatre axes prioritaires que je rappellerai et que nous avons largement évoqués. restaurer la viabilité des services et le modèle économique des opérateurs de frais de ferroviaire, améliorer la qualité de services d'SNCF réseau, investir dans les infras permettant le développement du frais de ferroviaire, accentuer la coordination avec le portuaire et le fluvial. Ce travail se poursuit à travers le travail approfondi d'identification à 10 ans des grandes priorités d'investissement pour le frais de ferroviaire dans le cadre du rapport Ulysse-Fret. Publié récemment. Par ailleurs, l'État soutient massivement, je l'ai dit, l'exploitation avec une enveloppe de près de 370 millions d'euros en 2025 dans une période tellement compliquée. Un effort particulier a été réservé aux wagons isolés, je l'ai dit également, dont l'aide a été augmentée de 70 à 100 millions d'euros. Je rappelle qu'il s'agit de la seule mesure en augmentation dans le budget des transports terrestres. c'est dire combien le fret est pour nous une priorité. Collectivement, nous avons réalisé un travail considérable pour surmonter les difficultés du secteur, notamment après la crise Covid, la crise de 2023. Vos interventions l'ont souligné, la question des péages, de la décerte des ports, du maillage territorial ou encore du développement du transport combiné sont autant de sujets qui nécessitent une réponse coordonnée. Ainsi, nous devons garantir la pérennité de ces investissements, continuer les efforts pour valoriser le fret face à la route ou à côté de la route et cela toujours dans un esprit de complémentarité entre les modes de transport ou encore sécuriser l'ouverture au capital d'Exafret. D'ores et déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en capacité d'annoncer de bonnes nouvelles concernant des futurs clients pour Exafret. C'est tout l'enjeu de la conférence de financement que nous lançons lundi prochain. Je ne vous dirai pas où ni à quelle heure Vous le savez déjà, j'ai voulu que le fret soit un axe apparent...

Il est un pilier central de notre politique de décarbonation et d'aménagement territorial. En investissement dans le fret, Nous investissons dans un avenir plus durable et plus résilient et plus équilibré. Le fret ferroviaire permet de réduire les émissions de CO2. Alors, on ne l'a pas dit, mais on le sait tous. Mais je le rappelle quand même qu'un train de fret représente l'équivalent de 40 camions de désaturer les routes, de soutenir le développement économique des territoires. Il est essentiel pour connecter les ports, les industries, les zones rurales, en favorisant une logistique plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Je sais pouvoir compter sur vous. Malgré les difficultés du fret, énumérées lors de ce débat, je vois également un secteur qui se réinvente, qui innove, qui ose. Merci à votre groupe de nous avoir permis de l'exprimer ce soir. Quand un train de frais de circule sur nos voies, ce n'est pas seulement 40 camions en moins sur nos routes. C'est l'avenir de notre industrie, de nos territoires qui se mettent en mouvement. Alors oui, le défi est immense, mais la France du rail a toujours su repousser ses limites. C'est ce que nous allons faire ensemble. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Pierre Corbizet pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste de Kanaki à l'origine de ce débat. Pour la conclusion. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux d'abord remercier le groupe d'avoir pensé à cette thématique ce soir et je vous dirai pourquoi la logistique m'interpelle un peu plus que d'autres. Je veux d'abord aussi remercier l'ensemble des collègues qui ont assisté à ce débat et ont pris la parole et vous remercier vous aussi, Monsieur le Ministre, de votre présence et votre participation. Tout ce que nous voulons d'entendre nous accorde sur un point. Le transport de marchandises est un sujet qui doit nous mobiliser davantage. La logistique est au cœur de notre société. Elle est indispensable pour lier les producteurs aux consommateurs dans le respect de notre environnement, c'est-à-dire en émettant le moins possible de CO2. Cela veut dire massifier les quantités, les stocker et augmenter si possible la longueur des trains de fret. Cette logistique évolue comme d'autres choses, d'ailleurs, à l'heure du tout numérique et de l'intelligence artificielle. Nous en avons débattu cet après-midi. Mais tant que nous n'aurons pas inventé la téléportation, nous devrons poser des outils modernes pour répondre à ce besoin de déplacement des marchandises. Je veux d'ailleurs évoquer sur mon territoire, même sur ma commune du Pas-de-Calais, La plateforme multimodale, trimodale, delta 3, je vous invite M. le ministre à la visiter, construite sur une ancienne friche minière, c'est-à-dire qu'au moment où on parle de la loi Tras, ce n'est pas inintéressant, bordure du canal de la Deul, qui sera bientôt en liaison avec le canal Seine-Nord-Europe, et la voie ferrée L'île Paris et l'autoroute A1. Mais quand nous avons imaginé cette plateforme il y a 25 ans, nous pensions à faire passer des permis charistes, parmi Fenwick, avec des bâtiments de logistique qui feront effet 6 mètres ou 7 mètres de haut. Mais aujourd'hui nous avons des bâtiments qui font plus de 12 mètres de haut. Et les trans-palettes Fendviks sont transformées en trans-stockeurs qui montent des palettes jusqu'à plus de 10 mètres de haut. Donc comme quoi l'évolution des marchandises, sans parler du stockage où on parlait à l'époque du picking, c'est-à-dire que la personne prenait un petit carton et allait dans tous les rayons, aujourd'hui tout cela... bien automatisée et contrôlée. Cela veut dire que nous nous sommes accordés ce soir, Monsieur le Ministre, sur le besoin de soutenir le fret, Firovière. Certains cherchent d'irresponsables pour expliquer comment fret SNCF est aujourd'hui en difficulté. Bien sûr, il y a l'Europe, on comprend un peu l'arrière-pensée de l'Union européenne. qui évoluerait dans un sillage que nous ne maîtrisons pas à l'Union européenne, est avant tout, pour moi, ce que nous en ferons. La décision de démanteler frais à TSNCF répond à une logique, celle de la marchandisation de la société. Là où il y a un besoin, il y a un marché. Et ce marché doit permettre à des entreprises privées de générer du profit. Pourtant, nous le voyons, cela mène à des dérives. Et même quand le besoin perdure, si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, alors personne ne répond à ce besoin ou différemment. Les camions sont donc préférés aux frais de ferroviaire. Il y a encore quelques mois, lorsqu'une entreprise avait un conteneur à faire transporter par SNCF fret, bien souvent il était transféré sur Géodis, qui est la filiale transport routier de la SNCF. Et oui, le Parlement européen a même proposé de les rendre encore plus gros avec les méga-camions autorisés il y a tout juste un an. Certains font semblant de ne pas voir que c'est une aberration écologique. C'est en plus une concurrence déloyale puisque les camions ne payent en réalité qu'une partie du coût de la route dont une grande partie repose sur la collectivité quand les camions ne sortent pas de l'autoroute payante et empruntent une route départementale pour avoir moins de frais de péage à payer. Par ailleurs, à la privatisation du rail, via l'ouverture de la concurrence contre un service public, ni aux frais de ferroviaire, des entreprises privées qui cibleront les lignes les plus rentables et déserteront les territoires avec le moins de parts de marché. Certains semblent ignorer que cette recherche de rentabilité empêche de répondre à un besoin et de satisfaire des usagers, alors que cela devrait être notre premier objectif. C'est là où il y a finalement deux visions distinctes dans notre hémicycle, comme au sein de votre ancienne commission, monsieur le ministre, et nous pensons qu'avec notre groupe, tout ne peut pas être soumis aux règles du marché. Le frais de ferroviaire en fait partie. Nous avons posé le débat du frais de ferroviaire en demandant comment le relancer. Il est vrai qu'avant de le relancer, il aurait fallu ne pas lui mettre des bâtons dans les roues, si j'ose dire. Et je pense notamment à la disparition de fret SNCF et à l'ouverture de la concurrence. Pour relancer le fret, nous l'avons dit, il faudra des investissements importants. Et nous serons à l'écoute des conclusions de cette grande conférence du lundi 5 mai prochain à Marseille, dénommée Ambition France Transport. j'espère que nos débats de ce soir auront ainsi servi à donner une trajectoire, des objectifs, une ambition pour laquelle il faut désormais effectivement se donner les moyens. Il faudrait plusieurs milliards par an pour le frais de ferroviaire. Pour faire face aux besoins, il y a l'ambition de doubler la part modale de frais de fureur d'ici 2032. Et nous savons où les trouver, nous, au groupe. C'est par exemple les fonds autoroutiers qu'il faut réorienter. Et je crois, M. le Ministre, que vous auriez dit être favorable pour y réfléchir. J'espère que vous êtes toujours convaincu d'être favorable pour y réfléchir. Mon groupe plaît pour renationaliser les autoroutes, c'est vrai, en conservant le produit des péages pour des investissements dans des mobilités moins polluantes, comme l'est le fret ferroviaire. Mais nous pouvons aussi cibler les profits tirés des concessions autoroutières, pour si financement, sans entendre la renationalisation. Mes chers collègues, monsieur le ministre, il est difficile de conclure ce débat, mais car tout reste à faire. Alors, après toutes les volontés positives que sont exprimées ce soir, je vous remercie de vos interventions. Espérons que les choix qui seront faits lors du prochain budget ne seront à vos côtés, monsieur le ministre, avec une loi de programmation annuelle du transport ferroviaire, pour que l'on ne pas rêver. En tout cas, les choix seront faits en ayant en tête cette volonté commune de relancer le frais de ferroviaire. Je vous remercie de votre présence. Merci. Mes chers collègues, par lettre, en date de ce jour le gouvernement demande l'inscription en deuxième point de l'ordre du jour du lundi 19 mai de la lecture sous réserve de l'ordre dépôt des conclusions de la commission mi-exparitaire sur la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale et du mercredi 21 mai de la lecture sous réserve de l'ordre dépôt des conclusions de la commission mi-exparitaire sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques. actes et données de cette demande. Nous pourrions en conséquence fixer le délai limite d'inscription des orateurs des groupes, respectivement au vendredi 16 mai au mardi 20 mai à 15 heures. Y a-t-il des oppositions ? Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance demain, mardi 29 avril à 9h30 pour les questions orales. La séance est levée.